La séance est reprise j'informe le Sénat que les des candidatures ont été publiés pour siéger au sein d'une part de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020, et d'autre part de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2018 actuellement en cours d'examen ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. La parole est à Madame Éliane Assassi pour un rappel au règlement. Oui merci madame la présidente d'avoir accepté ce rappel aurait vraiment qui s'inscrit d'ailleurs dans celui qui a été sollicité ce matin par notre collègue Nathalie Goulet Donal Trump a il y a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il a ainsi mis fin à une pratique initiée par Bill Clinton de maintenir Tel-Aviv comme capitale reconnu et siège de l'ambassade américaine en Israël malgré le Jérusalem Embassy de de 1995 cette décision constitue une véritable faute politique heureusement très largement condamnée dans le monde et en France, après une première réaction timide hier au soir, notre diplomatie a pris la mesure de la provocation du locataire de la Maison-Blanche en faisant partie de 8 pays demandant en urgence la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU c'est annoncé cette décision du président américain constitue une véritable provocation et mettent le feu aux poudres dans une région qui clairement n'a pas besoin de cela une provocation vis-à-vis des Palestiniens, tout d'abord, qui depuis des décennies, luttent pour leur intégrité territoriale reconnu par l'ONU et pour leur droit une provocation ensuite vis-à-vis des Israéliens, désireux d'arriver à un accord de paix et qui, chaque jour, lutte contre les groupes violents et ne de tous bords et de toutes nationalités, une profonde, une provocation enfin vis-à-vis de l'ensemble de la communauté internationale, dont les décisions et prises de position s'accumulent de la reconnaissance de Jérusalem comme ville internationalisé en 49 à la nécessité de conclure un accord instituant 2 états indépendants et libres en 2017 suite à l'initiative de Paris, en passant par la reconnaissance de Jérusalem Est comme occupés en 67 reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël s'est réitérer l'échec du Camp David II en 2001 de 2000 2001 éloigner encore toute perspective d'une paix durable et solide entre les Israéliens et les Palestiniens, qui ne se concrétisera que par l'instauration de 2 états indépendant dans les frontières issues de la résolution onusienne de 1967 Donald Trump a agi, on va-t-en-guerre patenté, en prenant cette décision et c'est acte insensé ne peut avoir pour conséquence qu'une nouvelle flambée de violence dont personne je crois ne sortirait vainqueur au vu de la gravité de la situation Madame la présidente, le Sénat dont l'expertise en politique internationale n'est plus à démontrer, s'honorerait de provoquer rapidement une réunion de sa commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées afin que la voix de notre chambre résonne fortement dans le débat public. Merci madame ceci donner de votre rappel au règlement. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission économie et article 54. Qu'inquiet 54 sexy F. 54 petit 54 obtiennent. Et du compte spécial prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, la parole est à Madame Frédérique Espagnac, rapporteur spécial de la commission des finances. à vous la parole. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la mission économique qui représente 1,9 milliard d'euros, est une mission très éclatée sur laquelle il est difficile de porter une appréciation d'ensemble : elle porte en effet une multitude de dispositifs en faveur des entreprises et notamment des PME dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, mais aussi les crédits des administrations, autorité administrative indépendante et opérateurs chargés de mise en 9 des diverses politiques c'est d'ailleurs cet éclatement qui explique très largement la stabilité de l'ensemble des crédits d'une année sur l'autre, je me limiterai donc à quelques remarques le ciblés sur les points qui seront retenus notre attention et celle de la commission des finances dans son ensemble, tout d'abord sur les instruments de soutien ont TPE-PME groupés au sein du programme 134, ils prennent la forme d'aides directes ou indirectes de prêts, de garanties de contribution des actions collectives de formation de promotion ou de mutualisation des moyens d'échelle d'une filière, il porte sur les secteurs très divers allant de la petite industrie aux métiers d'art en passant par les commerces de centres-villes, les services à la personne, ou encore les jeunes PME innovantes, le plus souvent il s'agit d'aides indirectes versées à des intermédiaires qui sont tout aussi nombreux opérateurs de l'État, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers de l'artisanat centres techniques, industriels, organismes de formation, etc, dans ces conditions, les arbitrages budgétaires de ces dernières années ont surtout consisté à régler du ira progressivement le format de ses multi-dispositif selon une logique de ceux-ci sont ainsi passés de 113 millions d'euros en 2015 à 80 millions d'euros en 2018, soit une baisse de 28 pourcent en 3 ans cette année prochaine la baisse devrait être de 12 pourcent l'exemple le plus significatif est celui d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, plus connu sous le nom de Fisac, dont la dotation a tellement baissé ces on en a, on en devient, à se demander pardon, si ce n'est pas comme si se fonds n'existait plus, nous, nous proposons donc tout à l'heure, un amendement à ce sujet, Madame la Ministre, ceci dit, cette logique de rabot finira bien par trouver ses limites au lieu de réduire chaque année un peu plus le budget de tels ou tels instruments sans trancher sur sa pertinence, il serait préférable d'engager une réflexion d'ensemble et de faire des choix politiques clairs et volontariste à force de ne pas choisir entre les outils, on finit par ne plus pouvoir mener une politique ambitieuse, pourriez-vous donc nous dire, Madame le Ministre, quels sont les choix du gouvernement en la matière, quels sont les dispositifs que vous entendez maintenir ainsi que ce que vous entendez allez-vous engager une rationalisation de ses moyens, tous ces dispositifs d'intervention, toutefois, ne compte que pour un tiers des crédits de la mission économie, celle-ci est également constitué pour moitié de crédit du personnel par nature assez rigide, en dépit d'efforts réels pour un 5ème 5ème des crédits de fonctionnement, les économies de fonctionnement sont elles aussi entravé par la multiplicité des structures dans le détail toutefois la situation varie je voudrais en particulier souligné que les crédits de l'INSEE, programme de 120 baisse assez peu cette année mais que cela s'explique par le surcoût ponctuels liés au déménagement d'une partie de ses services au centre statistique de Metz en voie d'achèvement après bien des difficultés et par le déménagement du siège de Montrouge en 2018 quant à l'allergène, hausse des crédits des services économiques de la DG Trésor programme 305 elle est en grande partie exogène et le et le taux de change de l'Euro qui fait mécaniquement augmenter le montant de l'indemnité versée aux fonctionnaires en poste à l'étranger, un mot pour conclure sur le plan France très Haut débit porté par le programme 343 en juillet dernier, ici même au Sénat, lors de la conférence des territoires, le président de la République a réaffirmé l'objectif d'une couverture à 100 pourcent du territoire en 2020, 2 mais sans annoncer de finalement supplémentaire, la partie de l'État reste fixé à 3,3 milliards d'euros sur les 20 milliards d'euros prévus à l'horizon 2020, dont 208 millions d'euros d'autorisations d'engagement sont prévues pour 2018 pourtant, Madame la Ministre, le plan France très Haut débit prend du retard, je ne parle pas évidemment des zones denses, comprenez zones rentables où les opérateurs investissent et où 66,2 pourcent des locaux sont d'ores et déjà je parle des réseaux d'initiative publique les RIP dans les zones non denses à ce jour, seuls 31,2 pourcent des locaux sont accès au très haut débit dont seulement 5,5 pourcent à la fibre optique dans ce contexte, et compte tenu de l'absence de nouveaux moyens financiers, pourriez-vous nous dire, Madame le Ministre, ce qu'entend faire le gouvernement en particulier comptez-vous utiliser la possibilité prévue par les textes, puis 2016, d'obtenir des engagements contraignants de la part des opérateurs, le cas échéant, assortie de sanctions financières, je vous remercie. Merci Madame le rapporteur. Monsieur Bernard Lalande, rapporteur spécial de la commission des finances. finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un mot pour commencer sur le compte de concours financiers près à des particuliers ou à des organismes privés dans le projet de loi de finances il correspondait presque exclusivement au Fonds de développement économique et social dit-elle DES bien que doté de 100 millions d'euros pour 2018, il n'est plus guère utilisé et son taux de consommation de l'ordre de 0 3 Autant dire que ce fonds n'a pas trouvé de preneur, hé bien non, pas du tout puisque une grande partie de ce fonds a été affecté d'une part au financement par l'état de la liaison Paris-CDG Express et d'autre part, un financement qui va être allouée à BPIFrance pour une hauteur de 100 millions, nous y reviendrons tout à l'heure dans le cas du financement d'une opération qui, avec le actuellement menée sur l'Iran pour en revenir à la mission économique je souhaiterais pour ma part, madame la ministre, insisté sur 2 sujets particuliers : premièrement, la politique de soutien à l'internationalisation des entreprises et notamment des PME et TPE qui sont nombreux à se lancer à l'export, la France compte quant à elle 125000 entreprises exportatrices, contre 360000 en Allemagne et 200000 en Italie. La création par le précédent gouvernement de Business France et de la BPI constituer un progrès important pour toutes ces entreprises le dispositif public de soutien à l'exportation dans son ensemble demeure défaillant, il suffit d'ailleurs de regarder les résultats de notre commerce extérieur. On a, compte tenu de la superposition bien connu dans notre pays une sur une superposition des compétences, une superposition des talents, mais jamais une superposition a fait une addition et en additionnant les talents et les compétences pourrait peut-être trouver une issue à ce déficit, qui devient structurel pour cela et je ce qui a mené une une réflexion du de la commission des finances, et donc a formulé des propositions, il y a quelques jours, le directeur général de Business France a remis ses propositions au gouvernement pour mettre l'agence au coeur d'une équipe France capable de faire travailler ensemble tous les acteurs à l'étranger comme dans les territoires où se trouvent nos potentiel exportateur en s'appuyant sur un outil innovant, un outil digital, notamment sur une plateforme en ligne unique et un véritable qui constitue un véritable système de gestion de la relation entre les usagers, madame la Ministre, pourriez-vous nous donner une première idée des suites que le gouvernement entend donner à ces propositions, une question particulière est crucial, a retenu notre attention : comment organiser le dispositif dans les territoires. Ces Business qui a su s'imposer à l'international comme un acteur incontournable, il y a une défaillance du système, dans la mesure où la connaissance de la connaissance de des entreprises, des PME et des TPE qui exportent sur les territoires, et sous l'autorité des chambres de commerce. 400 conseillers de chambres de commerce en fin de compte, sous l'autorité d'une d'une organisation d'un organisme qui a une vocation de relations avec le Business France c'est ce qu'on appelle la superposition et donc aussi bon préfère infiltrant et lorsque l'on filtre les compétences lorsque l'on filtre les talents, on arrive à un moment donné certainement à une synthèse mais aussi à des résultats qui nous amène à considérer que le déficit du commerce extérieur de la France structurellement à à regarder une avec un complètement nouveau, c'est là que les complémentarités entre Business France et les chambres de commerce

le second sujet, Madame la Ministre, que je sois qui je souhaite attirer votre attention, c'est la French Tech centrale, nous avons eu l'occasion, avec mon collègue Frédéric de visiter dans le 13ème arrondissement, la station Elf et cette station Elf a un Avantage extraordinaire, c'est qu'elle permet de réunir en un même lieu non seulement des entreprises innovantes, des Start-Up mais de réunir en même temps à une une une somme de services publics qui sont à la disposition de ces entreprises et donc de créer une légèreté, une fiabilité de l'information en Direct il y a encore quelques éléments à parfaire, mais on s'aperçoit néanmoins

peut-il émerger une disposition d'ordre général jour merci. Merci, monsieur le rapporteur, merci. La parole est à Madame Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le gouvernement nous invite à adopter une mission dont les crédits sont stables, avec une légère baisse de 1 pourcent des crédits de paiement, de fait, elle ne comporte pas de bouleversements profonds pour les entreprises, les mesures qui les affecteront l'an prochain, relevant essentiellement, choix de la première partie du présent projet de loi soit du PLFSS si bien que votre commission des affaires économiques, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission, elle a également procédé à cette occasion à l'examen des moyens mis en oeuvre par l'État pour assurer la conduite des politiques en faveur des entreprises dans le cadre des financements assurés par la mission, à ce titre, la commission a considéré que le Fisac était un instrument d'intervention qui avait fait ses preuves et qui devrait constituer un élément majeur de la stratégie de revitalisation commerciale des centres centres-villes, la commission a regretté le caractère particulièrement modique de la dotation prévue pour 2018 et sur ma proposition, s'apprêtait à la avant que les députés ne se saisisse du sujet et votent une augmentation de 2 millions d'euros malgré cela j'insiste pour rappeler que le Fisac est le dernier instrument de soutien opérationnel du budget de l'État en la matière et mérite qu'on lui accorde bien davantage, c'est pourquoi je suis totalement favorable à l'amendement de la commission des finances, qui va encore plus loin dans cette voie je précise que la commission économique souhaite ardemment que ces fonds soient majoritairement orientée sur la revitalisation des centres-villes et centre bourg votre commission s'était également inquiété de la diminution drastique des crédits d'intervention accordée aux instituts de consommation et associations de consommateurs, cette baisse de l'ordre de 40 pourcent aurait conduit le monde de la consommation dans une impasse financière immédiate, l'Assemblée nationale a finalement limité la diminution des crédits à 5 mais pour autant il est nécessaire d'engager très rapidement une réflexion de fond sur le rôle des différents acteurs de la consommation et les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics doivent apporter un soutien, enfin, malgré une augmentation des crédits budgétaires pour financer l'activité de garantie de BPIFrance cette dernière devra malheureusement revoir son offre à la baisse cela pose la question préoccupante de la pérennité d'une politique favorisant l'accès au crédit des entreprises, notamment les plus concernés, c'est-à-dire les PME et les TPE, l'existence de mécanismes de garantie de masse sur fonds publics reste essentiel il conviendra donc d'être vigilant sur les choix du gouvernement à l'avenir, je vous remercie. La parole est maintenant à madame N4. Et Noizier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, Madame la Ministre, mis, chers collègues, l'analyse du volet numérique et poste de la mission économique conclu un avis favorable, elle fait émerger 4 points, a souligné concerne la le transport de la presse, par la Poste qui apparaît toujours problématique cette activité de service public est structurellement déficitaire pour la Poste et les tarifs postaux fausse fausse visiblement la concurrence entre les différents types de presse la méthode unilatérale et sans concertation, choisie par l'État pour prendre la suite des accords dits Schwartz mais là non plus pas satisfaisante 2ème point le fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle qui devrait être mis en place en janvier prochain, géré par l'Agence nationale des fréquences, il prendra en charge les coûts de la lutte contre les brouillages de la télévision diffusée par voie hertzienne terrestre de plus en plus fréquent du fait notamment du déploiement de la 4 il conviendra donc Madame la Ministre, de doter ce fonds de façon suffisante afin de répondre aux nombreuses déficiences déjà constaté 3ème point la subvention à l'Arcep aussi satisfaisante mais l'autorité s'est vu notifier un schéma d'emploi à moins 3 7, sa situation apparaît peu compatible avec le fait de confier régulièrement de nouvelles missions à l'autorité 4ème point le plan France très au début qui devrait faire l'objet de certains ajustements dans les semaines à venir, à cette occasion, il serait souhaitable que le gouvernement établisse une trajectoire de financement au-delà de 2000 et renvoie la question de la fiscalité des opérateurs télécoms à ce jour contre incitative, j'en viens au point approfondi, il s'agit de la place du satellite dans la couverture numérique, le déploiement des technologies filière fait aujourd'hui face à des difficultés physiques et financières qui ne permettent pas d'atteindre les territoires peu dense et les habitats isolés afin de remplir les objectifs de bon au débit en 2020 et de très haut débit en 2020, 2, il convient de s'appuyer sur un bouquet technologique comprenant l'ensemble des technologies hertziennes et le satellite en fait partie, le satellite présente des avantages, il ne nécessite pas de recourir aux fonds publics pour financer l'infrastructure la fera structure, il pourrait être déployée rapidement en France mais aussi dans les territoires ultramarins et les repositionnent arable en fonction de l'avancée de la fibre un travail préalable d'identification des besoins et bien sûr nécessaire et devra être conduit en vue de bien choisir les options technologiques les plus rationnelle d'un point de vue économique enfin, alors que certains industriels envisagent de développer cette offre avec un satellite américain, il est absolument nécessaire, Madame la Ministre, de privilégier le recours à un satellite de fabrication franco-européenne l'ensemble des acteurs, constructeurs, opérateurs, fournisseurs d'accès internet doivent rechercher un accord sur ce sujet stratégique d'indépendance technologique pour la France comme pour l'Union européenne en ce sens, le plan France très haut débit doit positionner la solution satellitaire dans des conditions optimisées à savoir améliorer la commercialisation du satellite, sachant qu'aujourd'hui, un seul des grands opérateurs ce propos proposent des offres et favoriser l'information des collectivités locales comme des utilisateurs pour expliquer les progrès technologiques qui ont eu lieu aujourd'hui sur l'Internet par satellite et les enjeux autour de cette industrie but en devenir, je vous remercie. Si Madame le rapporteur, la parole est maintenant à monsieur Martial Bourquin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, Madame la Ministre, chers collègues, mon rapport pour avis porte cette année sur un axe étaient émergents et à mon enfance, à mon sens essentiel des politiques de soutien à l'industrie, à savoir le projet industrie du futur ce ce projet issu des 34 plans de la Nouvelle France Industrie industriel et l'équivalent du plan industrie 4,0 de l'Allemagne. Il vise à accompagner l'industrie française en son virage vers le numérique, avec des enjeux forts en termes de gains de productivité, de montée en gamme et certainement de relocalisation de nombreuses activités industrielles, ce projet comprend principalement 2 volets : le 1er vise à favoriser l'émergence d'une eau française solution 4,0 pour l'industrie par exemple dans le domaine de la Cobo tic de la fabrication additive c'est le volet des start-ups de la French Tech, et plus largement des politiques de soutien à l'innovation, je n'y assiste pas le second moins médiatique mais tout aussi important, vise à accompagner le déploiement des solutions techniques de l'industrie du futur dans l'ensemble du tissu industriel, toutes branches confondues orchis, les grands groupes ont pris le virage de l'industrie du futur des entreprises de plus petite taille, sont beaucoup moins mobilisé et surtout pour des raisons financières sur cet enjeu, je tiens donc à saluer le travail de conseils et d'accompagnement, réalisé avec peu de moyens, par les régions par l'Alliance Industrie du futur pour aider ces entreprises à s'engager dans cette voie 5000 PME TI bénéficier d'un accompagnement personnalisé et il faut Madame la Ministre, amplifier, c'était fort concernant l'aspect financier, toutes ont salué l'intérêt des prêts industries du futur, distribué par BPIFrance je souhaite attirer votre attention sur l'intérêt de créer un dispositif de sur-amortissement ce dispositif va a été voté au Sénat, il a maintenant à la disposition de l'Assemblée nationale et de vous, madame la ministre, s'il faut le recentrer sur l'industrie du futur et le réserver aux PME et ETI discute 11 ans une mesure générale de sur amortissement pourrait paraître coûteuses si nous sommes dans un une cible d'industrie du futur on peut donner une chance à ces PME assez et jetés de pouvoir s'équiper en digitalisation en robotique et encore gothique simplement une statistique, la France achète toujours cette fois moins de robots que l'Allemagne 2 fois moins que l'Italie ce mécanisme de suivre amortissement ciblés pourraient faire en sorte que notre industrie s'équipent réellement avec c'est industries du futur, il en va de la localisation de nos entreprises, il en va, à côté de nos grands groupes de touches c'est équipementiers qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à pouvoir s'équiper et à pouvoir se doter de ce virage extraordinaire, une nouvelle révolution industrielle, merci de votre attention. Merci monsieur le rapport. Monsieur André RSA. Rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame Madame la ministre, madame la présidente, mais, chers collègues, comme chaque année, la commission des lois, examiner les crédits du programme développement des entreprises régulation au titre de ses compétences en matière de droits des entreprises et de la consommation, je ne reviens pas sur la baisse cette année encore des crédits de paiement, cela a été dit ce programme reste fortement mis à contribution par l'effort budgétaire mais en 2018 cette baisse affectera lourdement certaines administrations en charge de ce programme, elle affecte aussi les crédits destinés à soutenir les entreprises à l'export, alors que c'est une priorité, une telle évolution ne peut bien entendu que susciter des interrogations, premièrement sur l'autorité de la concurrence, en dépit d'une hausse optique du plafond d'emplois ces crédits de fonctionnement vont diminuer de près d'un 1000000 d'euros, empêchant tout en réalité d'atteindre ce plafond, Madame la Ministre, comment justifier cette situation avec l'accroissement des fonctions des missions confiées à l'autorité, en particulier, depuis il y à peine 2 ans vis-à-vis des professions réglementées du droit à cette idée, nous voyons bien que la mise en oeuvre de la réforme de ces professions, à commencer par les notaires est assez éloignée des objectifs affichés, que ce soit sur le renouvellement de la profession ou sur la viabilité économique des nouveaux offices, deuxièmement, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, celle-ci va connaître en 2000 il 18 une forte baisse de 45 emplois et de 4,3 pourcent de ses crédits de paiement aujourd'hui déjà les agents dans les services déconcentrés ne sont plus assez nombreux pour assurer une vraie protection des consommateurs, année après année, en observant les indicateurs d'activité de cette direction, nous faisons le constat que son organisation administrative accentue les effets négatifs de la fonte des effectifs le ministre dans le cadre du plan action publique 2022 a bien proposé une réorganisation de ses services afin de rétablir la chaîne hiérarchique sur le terrain, Madame la Ministre, cela vous avez déjà été demandé tout à l'heure pour vous, pouvez-vous nous en dire plus, troisièmement, la direction générale des entreprises, là encore, nouvelle baisse des crédits et des effectifs, les services déconcentrés dans l'épaule 3 E des Directs qui n'ont déjà plus de crédits d'intervention vont en pâtir un n'en pas douter, on ne peut pas avoir durablement d'un côté, mes chers collègues, des services déconcentrés de l'État voit de j'ose dire, nécrose par l'attrition de leurs effectifs et de leurs crédits et d'un autre côté, des acteurs dynamiques qui se coordonnent mieux et qui prennent des initiatives telles par exemple Business français les CCI sur l'internationalisation, tels par exemple les régions et les compagnies consulaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre des fameuses schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en matière d'accompagnement des entreprises à la faveur de la loi notre une clarification déresponsabiliser c'est nécessaire entre l'État et les régions, l'État doit rester responsable des priorités nationales et des politiques de soutien des filières, mais le rôle d'impulsion et de coordination des régions et reconnue par tous les acteurs au niveau local, il faut désormais en tirer toutes les conséquences Business France enfin le niveau des subventions de l'État va aussi nettement baissé restreignant les capacités d'accompagnement des entreprises dans ce contexte de baisse de crédits plus marqué en 2018, la prise de conscience est faite de la nécessité de revoir singulièrement l'organisation territoriale des services de l'État en outre le dynamisme des autres acteurs redonne confiance dans une amélioration à venir de l'accompagnement de nos entreprises dans les territoires comme à l'étranger, au vu de ses perspectives et dans l'attente de leur concrétisation mais Madame la Ministre, nous posons la à Naples 2 fois et c'est la foi qui sauve la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de ce programme. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention en général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir, la parole est maintenant à Madame Noël ressent pour la République en marche. Madame Madame la présidente, Madame la Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues. Nous examinons la une mission qui est central centrale parce qu'il s'agit de l'autorisation parlementaire d'une stratégie économique concrète, efficace, capable de répondre aux défis contemporains. à travers 4 programmes, cette mission a pour ambition de favoriser l'emploi, la compétitivité des entreprises, le développement des exportations, ainsi qu'à assurer la protection des citoyens consommateurs. Dit autrement, il s'agit de l'une des pierres à l'édifice de transformation de l'environnement économique français que porte le gouvernement. Nous avons des champions nationaux qui signent des contrats en milliers d'euros mais nous avons aussi vivier d'entreprises dans nos territoires qui les font vivre. Dans l'Yonne, l'entreprise 3D qui fabrique des exosquelettes n'a rien envier technologiquement aux pépites américaine ou chinoise. Parce qu'elles dépendent moins de gros contrats, l'activité des petites et moyennes entreprises et plus stable, ce qui est plus, ce qui est important pour les territoires qui ont souffert de fermeture de grosses unités. Mais, chers collègues, beaucoup a déjà été fait pour les petites et moyennes entreprises depuis l'été, comme la création d'un code de travail numérique la primauté donnée au fond sur la forme, en cas de prise de décision, l'ouverture du dialogue social dans les petites entreprises. Le projet de loi de finances complète ces mesures. Citons par exemple la transformation du CICE en baisses de charges pérennes ou encore la baisse de l'impôt sur les sociétés. Qui concerne en tout 1er lieu les PC, les PME, puisque le taux normal d'impôt sur les sociétés, passe de 33 pourcent à 28 pourcent dès 2018 pour les 500000 premiers euros de bénéfices des entreprises. Par ailleurs, un volet important à destination des entreprises et des territoires concernés un point central pour l'attractivité de ces derniers et leur développement économique, la question du très haut débit. Lors de la conférence des territoires en juillet dernier, notre président de la République a annoncé que la couverture de notre pays en très haut débit serait une priorité. Le but est donc de poursuivre le plan France très Haut débit initié dès 2010 en ayant pour objectif de construire la totalité du territoire à l'horizon 2022. Rappelons que, selon l'agence du numérique est telle que cela a été souligné par le récent rapport des députés Laure de La Raudière et Éric Bothorel 13 13 millions de Français n'auraient pas accès à un débit Internet fixe de qualité dans certaines zones, les connexions Internet restent aléatoires, voire impossibles et n'est parfois même pas possible de téléphoner d'un portable. Sur le haut débit, seulement 50 pourcent de la population bénéficie du service du très haut débit essentiel aux entreprises. La fracture numérique entre les territoires existe bel et bien, et au XXIe siècle, nous ne pouvons laisser les utilisateurs dans cette situation d'inégalité que cela concerne l'affaire privée ou professionnelle. à l'heure où la numérisation des services se généralisent et devient même obligatoire, nous ne pourrons pas abandonner une partie de nos territoires au bord de la route, la couverture numérique est essentielle à la survie des territoires ruraux et à leur développement. Un document publié il y a quelques jours par l'Association des maires de France diffuse une carte de France éditée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Arcep : elle permet de visualiser très clairement le déploiement de la fibre optique dans notre pays, la prédominance des zones non couvertes saute aux yeux : la carte par commune est essentiellement blanche car 95 avec pourcent des communes ne sont pas concernés par la fibre. à de rares exceptions, seules les villes grandes et moyennes sont fibré et le monde rural reste presque totalement déserté, n'oublions pas l'Outre-mer où seule la réunion est assez bien pourvue, alors que les autres territoires sont presque totalement privée de fibres, on ne peut pas envisager que des professionnels souhaitant poursuivent leur activité ou s'implanter dans des zones rurales ne puissent pas bénéficier de réseaux Internet et de téléphonie mobile. Nous savons tous que le numérique est un enjeu de croissance et de compétitivité, particulièrement dans nos territoires ruraux qui se dépeuplent. Nous connaissons par ailleurs les faiblesses actuelles au niveau local, plan d'affaires trop optimiste des réseaux d'initiative publique manque de moyens des collectivités pour contrôler l'action des entreprises auxquelles elle délègue la construction, l'exploitation de leurs réseaux. Est-il réaliste de penser que la fibre optique pourra être ramené vers les zones blanches et les zones grises d'ici 2022. Soit dans 4 ans, les crédits seront-ils suffisants, la Cour des comptes a estimé récemment que le coût du plan vrai à 35 milliards d'euros au lieu de 20 milliards prévus avec un objectif tenu autour de 2030 plutôt que 2022, à certains endroits, les travaux de mise en place de la fibre ont été entamées, mais stoppée par manque de financement afin de garantir la compétitivité des entreprises installées dans une autre chose que le mal couvertes comme cela peut être le cas dans mon département de l'Yonne où la couverture est parfois aléatoire, voire inexistant, il est indispensable de s'appuyer sur un ministre technologique, c'est-à-dire ce racisme intégrant des techniques de transition. La couverture numérique doit véritablement touché tous les territoires, il est donc nécessaire d'engager des négociations de ou pour les conduire à assurer à tous un accès légal.

Alors la parole est maintenant à monsieur Fabien Gay du groupe CRC. Pour 5 minutes. Merci beaucoup.

Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur Madame et rapporteur mais chers collègues lors de la présentation de la première partie du budget, monsieur le ministre de l'économie, nous avait donné sa vision de l'économie et le fil rouge de votre budget il faut libérer le capital alors juste 2 chiffres pour illustrer mon propos, 56 milliards d'euros a été versé aux actionnaires en 2016, c'est-à-dire 13 milliards de plus qu'en 2015

on est donc loin, comme le démon de ces 2 chiffres de l'emprisonnement du capital mais puisqu'il faut le libérer, ou plutôt le débridé, vous y allez franchement, au moins, je dois vous reconnaît, de la cohérence et de la Pena cité économie fondée entre autres sur la cession d'actifs de l'État, suppression de l'ISF, réduction de l'impôt sur les sociétés, cotisations sociales Kohl sidéré comme décharge remise en cause du droit du travail, je dois vous avouer ne chose je ne suis pas un grand spécialiste de l'alpinisme, comme ça se voit, alors peut-être pourrez vous expliquer, madame la ministre, cette fameuse théorie du 1er lot cordée pour ma part, j'ai toujours préféré les sports collectifs, notamment le rugby où chacun donne en fonction de ses moyens et récolte en fonction de ses besoins, pour notre part, nous coïncideront que ce projet de loi de finale favorise les rentiers et les spéculateurs et non l'économie réelle, l'État a renoncé, en plus de sa milliards d'euros de recettes annuelles en espérant que cet argent sera réinvesti par les ménages pour développer des entreprises françaises mais cet espoir est bien légers lorsqu'on sait que rien n'oblige à investir dans notre tissu des PME et que rien n'oblige à investir en France LCI ce budget loin de soutenir massivement nos entreprises et le prolongement des politique austérité du précédent quinquennat pourtant nos entreprises ont besoin d'accès massif au crédit d'interlocuteurs étatiques fiables d'encadrement de la sous-traitance d'investissement pérenne, or l'État ne se donne pas la capacité d'intervenir en soutien et comme prix si l'enjeu est de préserver des savoir-faire et des emplois à moyen et long terme ou encore en renforcement voire une création de nouvelles filières industrielles, les crédits de cette mission illustre le désengagement de l'État, en effet, celui-ci ne place plus par des mesures volontaristes et ciblées, mais par le levier fiscal, or ce dernier ne peut pas remplacer le soutien Direct aux entreprises par la dépense publique, si, comme cela a été souligné en commission, le principal le levier d'aide aux entreprises reste de nature fiscale non budgétaires, ce que j'ai, c'est moins de mesures directes en faveur des entreprises moins de 2 milliards d'euros et près de 90 milliards de mesures fiscales, elles discriminer c'est-à-dire aveugle et à l'efficacité plus que douteuse, Avantage qui bénéficieront encore une fois aux grandes entreprises savent que l'impact en termes de création d'emplois ne soient évalués et cela même si ce sont les TPE et les PME qui font la force de notre appareil productif et qu'il faut aider à se développer dans le détail, nous déplorons maintenant depuis plusieurs années, la baisse de plusieurs de plusieurs pas aussi essentiel elle aussi le qui est encore en baisse en 2018 passe à 11 milliards d'euros en crédit de paiement se jouent pourtant un rôle essentiel dans la préservation et la modernisation du tissu commercial en zone rurale, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le centre bourg à moins de 10 ans ses moyens baisser de 83 pourcent nous saluons donc la manne demain, adopté en commission, pourtant, les crédits du Fisac à 30 millions d'euros de même nous a fait la promotion de la protection de la sécurité du consommateur, comment dès lors expliquer la baisse continue des dotations allaient donc GC CRF, comment justifier la baisse prévue initialement de 40 pourcent des crédits d'intervention pour les associations de consommateurs agréées El-Hammam demain, a été votée à l'Assemblée nationale pour réduire cette baisse annoncée à 7 pourcent Halphen pour conclure alors que notre industrie est toujours en crise, les crédits destinés au soutien à la politique industrielle recule de 12 loin de préserver notre Patrimoine industriel, il semble au contraire que le gouvernement ait fait le choix de santé sanitaire et c'est que ce soit du terme budgétaire ou patrimonial, nous regrettons réussi qu'il n'y a pas de ministère de l'industrie dans ce gouvernement, enfin la vente de fleurs industrielle à des groupes étrangers semblent s'accélérer l'État prévoyait un plan de cession d'actifs de 10 milliards d'euros à vos bourdes la nécessité de trouver des moyens pour assurer la stabilité capitalistique de nos industries, aujourd'hui il n'est plus à démontrer que les entreprises individuels et les PME font la richesse de nos territoires et permettent de lutter contre la dérive désertification il est illusoire de croire que nous pourrons faire de la France une Start-Up nation en ne soutenant que le innovation et en reléguant le savoir-faire qui ont fait la richesse de nos territoires, quoi qu'il en soit, malgré les discours, ce budget ne soutiennent ni l'innovation ni le savoir-faire ni finalement l'industrie, et comme vous l'aurez compris d'entre vous faire ce vote raconte. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre de pour le groupe, les indépendants.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la mission économie rassemble les programmes et les administrations qui ont pour objet d'encourager l'emploi, la compétitivité, les exportations de la concurrence et la protection des consommateurs, elle est composée de 4 programmes dont le récent programme plan France très Haut débit qui devrait financer la couverture intégrale du territoire en internet fixe très haut débit d'ici à 2022, cette mission doit être l'un des vecteurs, l'un des bras armé d'une nouvelle façon pour l'État d'intervenir dans l'économie, l'État français, traditionnellement état stratège doit en effet repenser son rôle dans une économie mondialisée, il doit savoir associer volontariste de politique et libération des énergies Édouard Oprah avec la logique de l'État pompier qui réagit avec éclat aux crises ponctuelles, sans être capable de dessiner une vision industrielle de long terme doit enfin accompagner les mutations du monde du travail sans laisser un seul travailleur au bord du chemin sans se résigner à la chute vertigineuse de l'emploi industriel que nous connaissons depuis quelques années. La France sans 16 usines, c'est le titre du livre de Patrick Arthus et de Marie-Paule Girard ce n'est pas seulement le signe d'un déclin industriel inexorable, il est un risque pour notre cohésion sociale et notre modèle de société cet effort industriel n'est d'ailleurs pas l'apanage de l'État, mais également des régions de la compétence de développement économique doit être mieux articuler avec celles des administrations centrales, je voudrais saluer ici l'action de Xavier Bertrand à la tête des France ses efforts constants en faveur de la reconversion des anciens territoires industriels portent leurs fruits et constitue un modèle de pragmatisme et d'efficacité sans tissu industriel robuste, il n'est pas de puissance exportatrice par exemple les excédents commerciaux titanesque de l'Allemagne sont le fruit de politiques de long terme pour renforcer le Mittelstand, le puissant réseau de PME et de TI allemande, si la France est encore le 6ème exportateur mondial de biens et services, avec près de 30 pour 100 de son produit intérieur brut, les chiffres du commerce t'extérieurs ne sont pas à la hauteur des attentes depuis quelques années, le solde des échanges de biens a baissé de près de 30 pourcent en 4 ans, le déficit commercial de la France s'est creusé en septembre 2017 de 500 millions d'euros pour atteindre 4,7 milliards d'euros, selon les chiffres des douanes sur 12 mois, le déficit cumulé de la France atteint 60,8 milliards d'euros, contre 48,1 milliards en 2016, soit un chiffre abyssal extrêmement inquiétant dans ce contexte, nous ne pouvons que regretter la diminution des crédits alloués au commerce extérieur, par exemple, vous n'avez pas augmenté Madame le Ministre, les crédits affectés à la Coface, la Business France dont les programmes d'aide à l'export sont nécessaires à l'accompagnement de nos PME à l'international, la France ne compte que 125000 entreprises exportatrices, contre 350000 en Allemagne, votre projet de budget ne prend pas en compte ce retard criant dont le comblement devrait être une priorité politique pour terminer je m'attarderai sur le plan France très haut débit, lors de la conférence des territoires du 17 juillet 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé sur l'objectif d'une couverture du territoire en haut débit d'ici à 2020 et en très haut débit d'ici à 2022, cela s'est traduit dans le projet de loi de finances pour 2018 par 200 1000 8 millions d'euros de crédits alloués au programme 343 nous estimons néanmoins que ce montant est insuffisant pour remplir les engagements du président de la République, la couverture numérique était essentielle à la survie de nos territoires à leur dynamisme et leur développement, nous souhaitons que ce budget traduise sincèrement les dépenses afférentes et que soit précisée la mise en oeuvre opérationnelle du plan France très Haut débit pour l'ensemble de ces sujets que j'ai évoquais le groupe les indépendants républiques et territoires et déçu par le manque d'ambition de cette mission et ne votera donc pas ces crédits en l'état. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Joël Labbé. Pour le groupe RDSE et pour une durée de 6 minutes chers collègues.

monsieur le ministre, Madame la Ministre excusez-moi. Mes chers collègues. J'ai tout d'abord évoqué le CICE qui reconduit encore pour cette année, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi représente à lui seul 20 20,8 milliards d'euros, soit plus de 72 pourcent du montant total de la dépense fiscale rattaché à cette mission, encore aujourd'hui, de l'aveu même du comité de suivi du CICE, il reste difficile d'évaluer les impacts réels de la mesure, toutefois, on nous annonce quelques chiffres : le comité de suivi s'accordent sur un chiffre de l'ordre de 100000 emplois préservés par la mesure entre 2013 et 2015 avec une fourchette allant de 10000 à 200000 ça manque toutefois de précision et si on part sur les 100000 ce qui permet par une simple division d'évaluer le coût par emploi de la mesure à 20000 euros par emploi par an ce qui somme toute est bien plus cher que les emplois aidés. Le seul bénéfice du CICE n'est évidemment pas l'emploi, et heureusement, nous dirons-nous, le CICE a permis de reconstituer des marges d'un certain nombre d'entreprises et, pour certaines d'investir, ce qui est une bonne chose, mais quand on y regarde de plus près, il a surtout permis à un grand nombre de rues, grandes entreprises, d'augmenter les dividendes pour leurs actionnaires, sans aucun bénéfice pour l'emploi et pour l'investissement en particulier, je voudrais citer la grande distribution 1er bénéficiaire du CICE qui ont profité de cet effet d'hommes d'aubaine pour certaines, même pour supprimer 2 des emplois, ce qui est un comble alors, chers collègues, ne serait-il pas temps de recentrer le CICE sur un certain nombre d'objectiver de secteurs dont on sait qu'il leur manque un coup de pouce pour embaucher pour investir pour innover, plutôt que de financer des dividendes pour les mesures futures qui sont en réflexion, on espère que cela sera prise en compte. Concernant les autres crédits de la mission peut souligner l'efficacité de certains mécanismes comme le Fisac reconnu par tous dans le recentrage en 2015 a permis une plus grande efficacité des dépenses, notamment concernant le commerce local en centre ville et dans les centres bourgs et particulièrement pour nos espaces ruraux, l'amendement qui porte les crédits du Fisac à 30 millions d'euros, nous le saluons nous aussi bien évidemment en ce qui concerne la fibre, l'annonce du président de la République d'une couverture numérique en très haut débit sur l'ensemble du territoire pour 2022, nous voulons y croire, nous espérons véritablement que le gouvernement tienne ses engagements sur notre département du Morbihan, il y a beaucoup beaucoup de doutes et on espère que, il faudra que la la puissance publique, ça me pose pour faire en sorte qu'on accélère les travaux, l'inquiétude est grande également au sein des associations agréées pour la protection des consommateurs, en effet, le programme 134 se voient amputés de 40 pourcent de ses crédits, ce qui pose un certain nombre de questions aussi bien sur les subventions directes que reçoivent ces associations, mais également en raison d'un crédit de de la baisse des crédits de la DGCCRF, on peut se demander comment dans ces conditions, nous allons pouvoir maintenir le même niveau de protection des consommateurs, je pense par exemple à l'application de la loi consommation et son volet d'interdiction de l'obsolescence l'obsolescence programmée ou encore du respect des normes alimentaires en ce qui concerne les résidus de pesticides qui font l'actualité, avant de conclure, je voudrais évoquer brièvement le projet industrie du futur, en effet, nous disposons d'un vivier de Start-Up technologiques dans l'ensemble des domaines prometteurs que l'homme aujourd'hui la French Tech Soutenir la structuration et le développement de cette filière est une nécessité si on veut éviter de se retrouver dans la même situation que nous vivons actuellement, concernant la situation écrasante des géants d'Internet américain, c'est pourquoi nous saluons ce projet en insistant sur les efforts que nous devons poursuivre dans les domaines de la formation professionnelle, afin d'accompagner les évolutions du marché du travail vers de nouveaux métiers qui vont rapidement et maire d'énergie dans ces domaines, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à madame Nathalie Goulet groupe Union centriste pour une durée de 6 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des finances, mes chers collègues, cette mission budgétaire me fait penser à une chanson de Barbara vous savez à chaque fois, on recommence le chemin on recommence la même chose, on recommence les mêmes explications chaque année et on ne voit pas beaucoup les marges, les marges de progrès, le rapport que vous avez dressé est accablant : superposition des structures cacophonie doublons inconséquence Business France c'est une petite éclaircie dans la nuit, pas assez, on vous proposera d'ailleurs quelques amendements au milieu, ce constat Madame le ministre, je voudrais plaider puisque vous arrivez dans dans cette maison pour la diplomatie parlementaire économiques et la coopération décentralisée, nous sommes nombreux ici à bien connaître nos territoires évidemment mais aussi à bien connaître les pays étrangers qui la Chine qui les pays du Golfe, l'Iran ou le Caucase et avoir noué pendant des années, des Liens avec les secteurs économiques et créer les les synergies nous connaissons, je l'ai dit, les territoires, nous connaissons les acteurs, nous avons les mettre en relation le service de coopération décentralisée doit être au coeur des dynamiques de notre commerce extérieur, il y a quelques années, notre collègue Jean-Claude Peyronnet, avait fait un petit inventaire il y avait 8 régions représentées au Sénat, qui entretenait dans la parfaite imperméabilité la parfaite ignorance de ce que faisaient les uns des autres, des coopérations avec la Chine sont évidemment jamais changé ni avoir de retour d'expérience, je voudrais vous citer plusieurs exemples, notamment la coopération entre Lyon et Dubaï Élisabeth Lamure connaît bien cette coopération il y a d'ailleurs beaucoup participé, c'est une coopération décentralisée qui a permis, outre l'établissement d'une ligne directe d'avion entre Lyon et et Dubaï évidemment

avait tenté de calquer sur l'ensemble des régions, le modèle de l'agence d'attractivité de l'Alsace qui est aussi une agence qui fonctionne très bien, malheureusement elle n'est pas arrivé au bout de de cette mission, c'est quand même dommage qu'on puisse pas dupliquer les opérations qui marche au lieu de toujours réinventer l'eau chaude, mais un ministre, je me suis amusée à dresser un état des lieux des outils au profit des collectivités territoriales pour asseoir leur coopération alors les autorités étatiques, bien sûr, la Commission nationale de coopération décentralisée qui a 3 missions : collecter les informations, les centralisé, ça nous a un peu dit un peu un peu indifférent, ce qu'il faut c'est c'est les diffuser et pas les centraliser, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire ensuite le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales bien suivi évidemment d'une délégation pour l'action extérieure des collectivités locales, suivie d'une mission opérationnelle transfrontalière qui a 3 missions: le dialogue avec les autorités nationales et européennes, je sais pas à qui elle parle en tous les cas, on n'a pas de rapport veiller aux intérêts des territoires transfrontaliers et délaissent porteurs de projet : premières nouvelles, mettre en réseau des acteurs d'expérience, le dernier rapport date de 2008, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils ont fait en disant ce serait pas mal d'avoir une évaluation ensuite viennent des instances de concertation politique des de coopération régionale pour l'outre-mer donc sagement mêleraient pas nos collègues de l'Outre-mer pour nous dire : l'association des maires des départements, puis le Conseil des communes et des régions d'Europe, puis des moyens financiers des cofinancements multiples et variés, un programme formidable qui s'appelle note alors je sais pas si si les très opérationnel ou pas des des programmes de coopération territoriale France-Espagne, Andorre, France, Belgique, les 2 maires le Rhin supérieur, l'Angleterre, la grande région l'espace alpin l'espace Atlantique les espaces Méditerranée etc, puis les fonds d'urgence humanitaire, les politiques de développement, le Conseil de l'Europe, les instruments de cohésion territoriale je m'arrêterai là, parce que d'abord j'ai plus le temps je voudrais aussi vous dire que, pour en finir Madame le ministre, il faudrait quand même que vous confier à des parlementaires une mission pour pouvoir vous faire un état des lieux, avoir un guichet unique, un peu d'évaluation de tous ces outils, parce que franchement diviser nos forces, c'est absolument plus acceptable dans l'état de notre économie, nous sommes franchement là dans l'inefficacité absolue dans la division des compétences et c'est quand même extrêmement dommageable, le Sénat est quand même l'endroit idéal pour la coopération décentralisée, nous connaissons nos territoires, nous connaissons les acteurs, nous sommes absolument à l'équipe de France qui doit être évidemment régi par l'ambassadeur, nous avons la France et son rayonnement partage et il serait grand temps de mettre de l'ordre dans la maison. La parole est

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, le budget 2018 de la mission économie s'inscrit dans une trajectoire qui conjuguent notamment 2 objectifs étroitement liés, le redressement économique et productif de la France et la contribution à la restauration progressive des comptes publics de la nation, c'était, il s'inscrit dans la continuité du précédent, je ne reviendrai pas sur le niveau des crédits des 4 programmes pour lesquels on constate une certaine stabilité mon propos sera plutôt cintré sur la question de la place et du rôle de l'État dans la politique industrielle dans notre pays a besoin pour retrouver leur rang et les employes qui n'aurait qu'il n'aurait jamais dû perdre sur la question majeure de la place de l'industrie dans notre production, nous partons de loin et la régression de la part de la production industrielle au cours des décennies passées, a été considérable, se traduisant par niveau de perte d'emploi de plus de 3 millions depuis 1980 après avoir cru pendant plus de 30 ans que les pays industrialisés industrialisés s'acheminer tous vers une société post-industrielle dans laquelle les activités de service supplantera les activités de production, on constate aujourd'hui l'émergence demande de hyper and Dust réelle, fondée sur la convergence de la productique du numérique et des services, les coûts très bas du transport maritime Jeannerat la spécialisation des productions et la reconfiguration des chaînes de valeur à l'échelle du monde, monde, ce contexte, la question de fond qui se pose est relative à la définition de la stratégie industrielle, que le gouvernement entend mener pour relever les grandes défi de la compétitivité et de l'emploi dans un contexte de mondialisation et donc de concurrence exacerbée, c'est l'objet du programme 3 5 stratégies économiques et fiscales et du soutien aux entreprises qui s'adapte au mode collaboratif qui prévalent désormais pour rester dans la course et cette, l'objet du programme central 4, développement des entreprises et régulation sur la question de la transformation des filières en quoi Madame la ministre, vous disquette vous distinguez-vous de la politique mise en oeuvre depuis la sortie du rapport Gallois dressant le constat donne décrochage industriel de la France politique qui s'est traduite par la même démarche dite de nouvelle français industriels décliner initialement sous la forme de 34 plans Reboux regroupées aujourd'hui à 9 solutions industrielles et une projet dit Usine du futur, sans oublier l'instinct de ce de partage que permet l'Alliance pour l'industrie du futur, quelle appréciation portez-vous sur l'écosystème qui a été mis en place dans notre pays avec les industriels eux- mêmes, mais industriels qui nous disent, quand nous les rencontrons, qu'ils ont besoin de stabilité et de visibilité à l'égard des mesures qui leur sont appliquées et qu'elle est ici la valeur ajoutée que le gouvernement entend apporter par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui produit des résultats encourageants et donc quelle place forcément nouvelles, l'État doit-il prendre dans ce contexte, doit-il se limiter au développement de politiques fiscales et d'allégement des charges comme le traduit le budget 2018 ou doit-il aller plus loin, personnellement, je crois qu'il faut aller plus loin dans le soutien à l'organisation industrielle du futur et là et à la montée en gamme de l'offre, l'État ne peut se limiter à agir sur la compétitivité coût qui n'est quand même un aspect de la problématique de la compétitivité, quelle politique de soutien à l'État entend-il aussi apporter à l'économie industrielle de nos territoires, souvent ruraux souvent structurer un pôle de compétitivité quand on constate dans ce budget, le très faible niveau de crédit que vous allez-y consacrer et que cette ligne est même en diminution de 1 1000000 d'euros à l'audition, le ministre de l'Économie a évoqué le concept d'état stratège qu'entendez-vous concrètement par cette notion à à cet égard, nous avons besoin de clarification de la doctrine du gouvernement en matière de participation de l'État au capital des entreprises oeuvrant dans des domaines affectant l'intérêt général et la souveraineté nationale, l'audition récente de monsieur le ministre de l'économie par la commission des affaires économiques à propos notamment d'Alstom et de STX nous a pas permis de comprendre où l'État veut aller, mais sa politique de participation, il ne faudrait pas qu'à terme l'État qui se veut stratège donc ce train de 120 spectateurs One commentateur de décisions prises par d'autres, au détriment de notre souvenir, la souveraineté et de nos emplois à partir de 2012, l'État s'est dotée d'une doctrine en matière d'actionnariat qui vise, je cite, pour les entreprises de jouer un rôle stratégique d'intérêt national à protéger les intérêts économiques et patrimoniaux du pays, en mettant un oeuvre les stratégies économiques, industrielles et sociales adaptées, garante de la préservation sur le territoire national des armes ploie et des compétences, cette doctrine a été conforté par l'instauration du droit de vote double qui permet de renforcer le rôle de l'État au sein des entreprises et le nouvelle gouvernance et les entreprises à participation publique a aussi vu le jour, d'autres l'état de plus de grandes de plus grande capacité d'influence dans les sociétés où ils détiennent une majorité du capital aujourd'hui la vente de 10 milliards d'euros de titres va diminuer drastiquement les actifs de l'État au bénéfice de qui aura lieu cette cession massive de titres et avec quel niveau de recettes financières pour le budget de l'État, quand on sait qu'actuellement, le rendement de ses actifs est supérieur à celui des marchés Kanoute au fonds de soutien à l'innovation qu'une partie de ses recettes de cession est censé alimenter comme le souligne le rapport pour avis de nos collègues de Châtillon élu réelle sur le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, il devrait financer l'innovation à hauteur de 2 à 300 millions d'euros, l'État a dépassé celui par ailleurs 8,5 milliards d'euros, dont 2,2 hors dépenses fiscales nous sommes pas du tout dans le même ordre de grandeur et on ne comprend pas la nécessité qu'il y aurait ainsi à céder ses 10 milliards d'euros d'actifs, on voit par cet exemple, qu'il y a une grande besoin de clarification de la doctrine de l'État en matière de participation au capital dans le cadre de la stratégie de développement économique quant à remettre à 9 le gouvernement d'autres points mériteraient d'être abordées mais je conclurai en disant que, compte tenu des incertitudes qui pèsent pour l'instant sur la stratégie du gouvernement sur la stratégie que le gouvernement a longtemps développés en matière économique, nous nous abstiendrons je vous remercie. La parole est à madame Patricia Mohr Richaud pour le groupe, les républicains pour une durée de 4 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre Mesdames, messieurs les rapporteurs du chers collègues permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par les différents rapporteurs sur la mission économie du PLF pour 2018 un sujet auquel je suis très sensible en tant que membre de la délégation sénatoriale aux entreprises présidée par notre collègue Élisabeth Lamure, sénateur du Rhône, si les crédits de la mission économie affichait une certaine stabilité, il existe néanmoins une grande disparité selon les programmes, une baisse de 7 pourcent des autorisations d'engagement du plan France très Haut débit : une augmentation de 17,5 pourcent des hommes terrorisation d'engagement du programme 134 au chapitre développement des entreprises et régulation au-delà des écritures comptables et du savante équilibre entre autorisations d'engagement et crédits de paiement, la mission économique est aussi un signal envoyé au monde de l'entreprise, je souhaitais partager avec vous 2 sujets qui me préoccupe et qui sont relatifs au programme développement des entreprises et régulation le 1er concerne le volet développement du tourisme ce chapitres pâtit d'une baisse de 67 pourcent des autorisations d'engagement et 56 pourcent des crédits de paiement, en effet, le gouvernement a décidé de supprimer tous les crédits d'intervention jusqu'à leur portée par cette action, les actions en faveur du tourisme se limiteront donc pour la mission à des dépenses fiscales liées à l'application d'un taux réduit de TVA et aux chèques vacances, la mobilisation complète du gouvernement annoncé par le 1er ministre lors du conseil interministériel du tourisme le 26 juillet à entériner l'absence d'un ministère dédié puisque c'est désormais le ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui en a la charge, un secteur qui pèse 8 pour 100 de notre PIB avec 2 millions d'emplois Directs et indirects, oui la France est la première destination touristique mondiale et nous ne pouvons que nous en féliciter, mais les actions doivent largement dépasser la promotion de la destination France à l'étranger, élu d'un territoire de montagne où le tourisme est un vecteur économique important, voire essentiel, je ne pense pas que de rattacher le tourisme au ministère des Affaires étrangères, soit un bon signal, je vous rappelle que le poids économique du tourisme en montagne représente 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont 30 pourcent de la clientèle est d'origine étrangère, nous devons mettre en oeuvre des logiques économiques qui nous permette de rendre nos territoires attractif et nos entreprises compétitives, c'est un gisement de croissance et d'emplois précieux pour notre pays, avec des emplois non délocalisables qui mérite toute notre attention, le second concerne le volet Fisac, en effet, alors que ce dispositif destiné à financer des opérations de créations de maintiennent de modernisation et d'adaptation de transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services a été réformé en 2015, les crédits prévus pour 2018 se sont largement insuffisants, comment un 1000000 d'euros pourrait-il permettre de préserver de développer le tissu d'entreprises de proximité et de répondre aux appels à projets pour Pro conduire des opérations collectives, individuelles spécifique au plan national, le Sénat s'est investi sur ce fut sujet et certaines de nos collègues du groupe de travail crever revitalisation du centre bourg et centre ville ils travaillent actuellement, en effet, la France voit nombre de ses centres villes des centres Bourse vider et mourir lentement, même si le constat est unanime et que ce phénomène était, est et continue, il n'est pas inéluctable pour autant des moyens financiers en rapport doivent-ils être consacrés, c'est pourquoi vous l'aurez compris je voterai ces articles sous réserve que des améliorer à Sion puisse être, il y a être apportée, je vous remercie. Merci, cher collègue, nous terminons par Monsieur Michel Vespa. Pour le groupe, les républicains pour une durée de 4 minutes. minutes. La présidente, madame la ministre mais, chers collègues, la mission économie porte sur un ensemble de dispositifs en faveur des entreprises, notamment des PME, des secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie ainsi que les crédits Administration, autorité administrative indépendante, opérateur chargé de la mise en oeuvre de ces diverses politiques je n'insisterai pas sur les dispositifs de soutien à l'économie concernés sur lesquels, mes collègues sont déjà largement intervenus, madame la ministre, je rejoins ma collègue certains dispositifs sont redondants et peu lisible pour les chefs d'entreprise, spécialement les petites et moyennes qui n'ont pas de services dédié à la compréhension des méandres et subtilité parfois tatillonne de l'administration en ce domaine, comme ailleurs, il y a un grand besoin de clarté et de simplification, loin d'être atteint au-delà je préfère évoquer un sujet qui me tient à coeur, celui de la transmission d'entreprise essentiel dans l'économie de notre pays dans le cas de la délégation aux entreprises créées en 2014 excellemment présidé par Élisabeth Lamure je travaille avec Claude nous depuis maintenant un an, à améliorer sensiblement le cadre législatif des transmissions et cessions d'entreprises pour tout type d'entreprise et tous secteurs, besoin j'ai dont j'ai bien mesuré l'importance, et même l'urgence ce mardi au salon, transfert de la transmission d'entreprise qui se tenait au Palais Brongniart où je suis intervenu en séance plénière, j'ai aussi entendu parmi les professionnels de la transmission, avocats, notaires experts-comptables, l'éloge de notre délégation sénatoriale et de la qualité du travail sénatorial qui me réjouit et que je veux partager ici avec tous mes collègues sénatrices et sénateurs, Madame la Ministre, permettez-moi d'évoquer le projet de loi sur l'économie préparé à Bercy dans le cadre du pain. Un mot sur la méthode, puisque l'association des parlementaires était évoquée avec un concept inédit et intérêts et intéressant de binômes, chef d'entreprise parlementaire, il semble que ces derniers n'a guère été sollicités ou alors sur certains bancs seulement j'étais moi-même demandeur, car depuis un an maintenant, nous avons produit dans le cas de la délégation aux entreprises un rapport qui débouche sur 27 propositions balayant ainsi bien aussi bien à l'aspect financier, fiscal, social, communication, animation de réseau alors faute d'avoir été consulté pour la rédaction de ce projet de loi, c'est ainsi que j'attire l'attention sur le contenu de la PPL que nous allons déposer et 12 et dont nous débattrons pour alimenter dans cet hémicycle le projet de loi du gouvernement.

il faut simplifier le cadre juridique de la transmission supprimer certaines obligations déclaratives, il faut encore s'agissant de transmission intrafamiliale modifier le pacte Dutreil instaurer un taux unique pour les droits d'enregistrement faciliter la reprise par les salariés naissance supprimant les articles 18 et 19 de la loi Hamon expérimenter certains dispositifs, notamment pour les entreprises agricoles et artisanales, redonner confiance aux chefs d'entreprise dans leur administration et notamment celle de Bercy, il y a là un très gros travail, nos entreprises ont besoin de retrouver confiance la parole et les grandes déclarations ne suffiront pas, elles attendent des actes, elles ont besoin d'être à des niveaux comparables à leurs concurrentes européennes, elles ont besoin de stabilité de confiance envers leur administration, j'espère, Madame la Ministre vous avoir convaincu de l'enjeu majeur que constitue la transmission et cessions d'entreprises dans l'économie de notre pays et nous espérons il y a être

Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, vous examiner aujourd'hui les crédits de la mission économique ainsi que ceux du compte spécial près à des particuliers ou à des organismes privés, je remercie l'ensemble des rapporteur pour la qualité de leurs observations, la mission économique porte un ensemble de dispositifs en faveur des entreprises et notamment les PME dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de l'industrie ainsi que le budget des administrations, autorité administrative indépendante et opérateurs, chargé de la mise en oeuvre de ces diverses politiques les crédits de la mission sont stables par rapport à 2017 et contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique économique du gouvernement, son objectif pour le quinquennat conformément aux engagements du président de la République devant les Français et de conduire la transformation en profondeur du modèle économique de notre pays. La dépense fiscale constitue un levier essentiel, elle est en forte augmentation en 2018, notamment le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui sera transformé en un allégement de charges à compter du 1er janvier 2019, plus largement, c'est le sens de la réorientation de l'épargne des Français vers l'investissement et l'économie productive et l'incitation donnée aux acteurs économiques et à nos concitoyens, a entrepris à prendre et à réussir à travers la mise en place de l'impôt sur la fortune immobilière du prélèvement forfaitaire unique et l'engagement sur le quinquennat de réduire l'impôt sur les sociétés de 33 pourcent aujourd'hui à 25 pourcent ces mesures pérennes, favorable à l'investissement productif ont été ont été pro-préféré aux mesures ponctuelles de sur-amortissement la réorientation de l'épargne doit in fine et soutenir l'investissement dans les entreprises pour leur permettent de faire face à leurs enjeux de modernisation et de développement, c'est par exemple le cas en matière industrielle, pour préparer l'industrie du futur, comme l'a évoqué votre rapporteur pour avis. Le gouvernement entend accompagner la vitalité, l'écosystème des Start-Up en France l'incubateur, station Elf, le plus grand E incubateur au monde avec 1000 Start-Up bénéficie, comme vous l'avez mentionné d'un pôle ou les ou les administrations sont représentés et que Gérald art inaugurera ce soir. De transformation en profondeur, il est également question au sein même de la mission économique dont plusieurs des mécanismes d'intervention en faveur des entreprises et notamment les PME, TPE sont améliorés en réponse aux observations de vos rapporteurs spéciaux je voudrais revenir sur quelques modifications importantes opéré par le PLF 2018 ces modifications de pas supprimer brutalement, telle ou telle dispositifs mais à rationaliser leur action et à les mettre au service de la politique de libération des énergies qu'entend mener le gouvernement. La rue budgétisation en 2018 des garanties bancaires accordées aux PME par BPIFrance finement, ce moment est une première modifications importantes pour 2018 la dotation budgétaire complété de la mobilisation des ressources internes de BPIFrance permettront d'assurer un niveau d'activités comparables aux années 2016, 2017, comme l'a indiqué le ministre Bruno Le Maire de vendre votre commission des vagues affaires économiques l'amélioration sensible des conditions de financement des entreprises et de leur santé, notamment des PME et TPE doit conduire à Saintes à réinterroger globalement le positionnement de l'activité garanti qui a fortement progressé de durant la crise, il convient désormais de construire un format répondant aux besoins de la reprise économique 2ème modification la poursuite de la rationalisation des dispositifs d'accompagnement des entreprises qui existent au sein des réseaux consulaires, le gouvernement s'est engagé en faveur de la baisse des prélèvements obligatoires parmi ces prélèvements : la taxe affectée pour le financement des missions de service public, réalisée par les chambres de commerce et d'industrie, votre aussi, pardon, a décidé de revenir lors de la discussion de la 1ère partie du PLF sur la diminution de 150 millions d'euros du plafond de prélèvements qui aurait permis de réduire à due concurrence, le taux de la taxe additionnelle assise sur le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée. Le gouvernement reste convaincu que les réseaux consulaires peuvent continuer à se moderniser et réduire leur appel au financement public il continuera apporter cette mesure dans cette optique, ont été engagés, comme vous le savez, des travaux permettant de déterminer le périmètre des missions de service public, effectués par les réseaux consulaires ils identifieront les pistes de nature à améliorer l'efficacité du réseau des chambres de commerce et d'industrie, je rappelle à cet égard que la dotation des fonds de péréquation et de modernisation de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau des CCI a été significativement majoré à l'Assemblée nationale, cela à amortir à la dinde, diminution des ressources affectées pour les chambres les plus fragiles financièrement. 3ème modification l'internationalisation de l'économie française vos rapporteurs spéciaux se félicite des progrès qui a permis la création de Business France il convient d'aller encore plus loin dans la simplification et l'efficacité du dispositif pour les entreprises, une réflexion en ce sens a été confiée au niveau du directeur général de Business France Christophe Lecourtier, qui vient de remettre ses conclusions au ministre de tutelle cette réforme sera guidé par la nécessité de rendre le dispositif d'accompagnement des entreprises plus lisible, plus efficace, plus simple et générateur d'économies pour l'État en France et à l'étranger, le sujet de l'articulation avec le rôle des chambres de commerce et d'industrie sera bien sûr central dans cette évolution. Bref, le PLF 2018 présente une première étape essentielle dans une démarche globale et cohérente pour renforcer le tissu des entreprises françaises. Cet effort se poursuivra à travers le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises dont Bruno Le Maire vient de lancer la consultation autour de 6 thématiques. les parle demain les parlementaires ainsi que les chefs d'entreprises qui sont étroitement associés je remercie en particulier le sénateur Young qui est mobilisée avec Éric Kayser pour animer le thème du développement international de nos entreprises, les préoccupations de Madame Nathalie Goulet quant à la coopération économique décentralisées pourraient utilement être portée à l'attention de ce binôme, j'ai bien noté que certains d'entre vous et la délégation des entreprises souhaitait aussi contribué c'est bien évidemment encore possible puisque les consultations s'engage et se poursuivent et seront encore en cours en début d'année prochaine. Vos rapporteurs ont fait part de leur attachement aux crédits d'intervention en faveur du commerce et l'artisanat, le Fisac. Le gouvernement en a tenu compte lors de la première lecture à l'Assemblée nationale en majorant de 2 millions d'euros les crédits, les crédits du Fisac, ce qui permet de stabiliser à leur niveau de 2017, les autorités les autorisations d'engagement et de majorer de près de 35 pourcent les crédits de paiement. 200 projets pourront ainsi être soutenu les stations-service dite de maillage, c'est-à-dire sans concurrent moins kilomètre constitue, pour leur part une priorité du règlement d'appels à projets depuis 2015, vous avez mentionné les actions de revitalisation des centres-villes, le Fisac a vocation à être un outil opérationnel à l'appui de notre politique en la matière. S'agissant des associations consuméristes, je voudrais rappeler l'attachement que le gouvernement porte à la protection des consommateurs, elle est assurée par l'action conjointe et complémentaire de la DGCCRF et d'autres acteurs, dont les associations de consommateurs. Pour autant, la fragmentation du monde consumériste qui nuit à sa visibilité à son efficacité, suite à la discussion de devant l'Assemblée nationale, le gouvernement a accepté de se donner un temps de réflexion en majorant les crédits de la DGCCRF alloués à ces associations de 3,1 millions d'euros. Enfin, pour terminer avec les observer de rapporteur de la mission économie regroupe en son sein le programme du plan France très haut débit, le gouvernement a souhaité accélérer ce plan essentiel pour la compétitivité mondiale de nos territoires en réaffirmant ce l'objectif d'un bon haut débit pour tous à horizon 2020 et le très haut débit pour tous à échéance 2020, 2, le gouvernement a lancé les travaux dès cet été pour s'en assurer. Des engagements devront être conclus avec les opérateurs, ils seront contraignants et donneront lieu à des sanctions pour les opérateurs qui ne joueront pas le jeu, le gouvernement a décidé de mobiliser l'ensemble des technologies disponible. Afin de ne laisser aucune habitation aucune entreprise sans solution d'Internet fixe offrant moins beau haut débit dès 2020 les réseaux de philo fibre Fibre optique mais également les solutions satellitaires nouvelle les réseaux mobiles 4 G en fait les réseaux radio le cas du satellite a été évoqué par vos rapporteur pour avis, il constitue une solution pour les zones du territoire national, difficiles d'accès comme les zones de montagne, les technologies spatiales viendront donc en appui du déploiement de la fibre optique. Je termine avec le comte de concours financiers prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. S'agissant du Fonds de développement économique et social qui finance les prêts de l'État en faveur d'entreprises en difficulté ayant des perspectives réelles de redressement sa doctrine d'emploi prévoit que les prev DES doivent permettent de compléter un tour de table, après des négociations financières avec l'ensemble des partenaires privés exposé en 2017 ce programme à disposer de 100 millions d'euros de crédit en en n'autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les montants unitaires des preuves accordée par le si peuvent être potentiellement très élevés, ils sont souvent décidée dans des situations d'urgence, liées à des crises industrielles et sociales majeures

pour ces raisons, la consommation de crédit reste volatile pour 2018 le montant des crédits proposés s'élève à 100 millions d'euros, garantissant un maintien des capacités d'intervention au niveau de 2017. La ligne nouvelle crédit export vers l'Iran, permettra aux entreprises françaises de tirer pleinement parti de l'ouverture des marchés iranien alors même que les sanctions internationales résiduelle à l'encontre de ce pays dissuade la plupart des opérateurs financiers privés d'y intervenir, les 100 millions d'euros ouvert par l'État à ce titre-permettront d'amorcer un dispositif de crédit export BPIFrance mettant par ailleurs en position de lever des financements privés dans des conditions vérifier de sécurité juridique, enfin, je termine avec le projet CDG Express qui vise à réaliser une liaison ferroviaire rapide Direct au niveau de service entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle essentiel pour améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire de Roissy à horizon 2024 ce projet contribuera au développement de l'image de la France à l'étranger et à l'attractivité économique de notre territoire, je rappelle que l'engagement de la France à mettre en servir cette liaison, a été l'un des critères et ont conduit à retenir la candidature de Paris aux JO votre haute assemblée a souhaité supprimer cette nouvelle dotation contre l'avis du de du gouvernement pour qui ce projet contenu de son caractère hors norme doit recevoir à titre très exceptionnel, un prêt de l'État à la société de projet. Merci madame la milice. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission économie figurant l'taper et nous commençons par 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune

madame la ministre, il s'agit d'un amendement qui a déposé notre collègue point trop avec un grand nombre de mes collègues du groupe, les républicains, tous les orateurs, tous les experts, tous les analystes disent le Fisac ces formidables, contrairement à bien des fonds, organisme qui existent et dont la l'efficacité est mise en doute, voilà quelque chose qui marche bien. Qui était absolument nécessaire pour la revitalisation des centres-villes des centres bourgs pour le commerce de proximité et voilà quelque chose qui marche bien et donc, par définition, on baisse crédits. C'est d'une logique implacable puisque ça marche, faisant en sorte qu'on ne puisse plus rien faire et donc l'amendement en question, il est simple on assiste depuis plusieurs années à la baisse des crédits du Fisac alors que tout le monde dit que c'est absolument nécessaire, alors nous faisons un amendement et Rémy-Cointreau afin d'amendement tout à fait extravagant, il est de dire puisque ça marche est-ce que, éventuellement, on pourrait avoir la raison de donner quelque crédit à quelque chose qui marche par rapport à des crédits souvent inutiles d'organismes, il ne sert à rien, donc voilà l'amendement est sympa, passer à 20 millions d'euros pour le Fisac c'est-à-dire globalement doublé quand on dit doublé tout de suite, on a l'impression qu'on fait des choses insensées mais doublé pour revitaliser les centres bourgs les centres-villes, c'est peut-être quelque chose qui dans le fond, dépend aussi de la haute assemblée qui représente si bien les collectivités territoriales. Merci monsieur Karoutchi la parole à madame. Espagnac pour présenter le 229 au nom de la commission des finances. son Anafe excusez-moi donc cet amendement donc qui a été votée en commission de finances vise de donc abondé à 17 millions d'euros les crédits Fisac permettant de doubler l'enveloppe actuelle entre 2010 et 2018 et la dotation de Fisac est donc passée de 64 millions d'euros à 11 millions d'euros en CP, soit une baisse de 83000 pourcent excusez-moi, ce qui est énorme, il est tout simplement pas possible de mener comme la dire monsieur Karoutchi une politique ambitieuse de lutte pour la désertification des territoires et la dévitalisation des centres villes et sur l'ensemble du territoire français, avec seulement 11 millions d'euros, la majoration sur 2 2 millions d'euros, adopté par l'Assemblée nationale n'apparaît pas à cet égard comme une réponse suffisante le présent amendement propose donc de porter les crédits Fisac à 30 millions d'euros en 2018 pour donner à cette politique les moyens de ses ambitions pour permettre à la réforme de 2014 qui repart sur une procédure d'appel à projets, de faire ses preuves qui, ce qui n'est pas le cas à ce jour, cet amendement répond aussi à une exigence de sincérité budgétaire chaque année en effet, les dépenses effectives engagées par le Fisac excède largement les crédits ouverts en loi de finances initiale pour exemple, en 2016 37,1 millions d'euros a été si contre 27,5 millions d'euros ouverts en loi de finances initiale sur ces 12 millions d'euros, 5 millions d'euros serait réservé à un fonds spécifique d'aide aux stations services de proximité, monsieur Karoutchi je précise juste ceci alors que celle-ci représente un enjeu crucial,

quelque 320 stations-service ont donc fermé, rien que pour l'année 2016, ce que nous pouvons tous constater les uns et les autres sur le territoire, or depuis la suppression de du comité professionnel de distribution des carburants en 2015, les aides aux stations services de proximité ne font plus l'objet de dispositifs dédiés à l'exception des, de de 2200 dossiers en souffrance au moment de la fermeture donc du CPDC, repris par le Fisac et dont le dernier a été clôturée en juillet 2017 afin d'assurer l'avenir des stations services de proximité, il importe donc de maintenir un dispositif spécifique géré par le Fisac notamment dédiée à la mise aux normes environnementales, remplacement des cuves aux énergies renouvelables bornes électriques station hydrogène à la diversification Relais Colis dépôt de pain, etc ou à la dépollution des stations, ne pouvons pas ne trouveront crédible serait donc transférée au programme 305 stratégie économique et fiscal, celui-ci porte la subvention versée à la Banque de France, qui est cette année en hausse alors que les gisements d'économie sont identiques, je vous remercie. Merci madame la rapporteure et maintenant l'avis de la commission sur l'amendement 185 rectifier. Merci madame la présidente, donc juste pour revenir donc sur la vie, comme je viens de le faire, nous avons voté une un amendement donc différent en commission des finances, donc c'est celui que je soutiens, je demande donc à monsieur Karoutchi au nom de de ses collègues, si possible, de le retirer au profit de l'amendement, donc 229 adoptée en commission des finances, cette solution vise comme votre amendement a doublé les fils du Fisac mais elle tient compte juste de la petite hausse des 2 millions déjà voté par les députés à l'Assemblée nationale, ceci permettrait de souligner face à l'inertie du gouvernement actuel, pour l'instant le Front commun constitué par l'Assemblée nationale et le Sénat. Merci madame la rapporteur à vie du gouvernement. Oui merci madame la présidente, merci madame la rapporteur donc, comme cela a été dit le le gouvernement lors du débat à l'Assemblée nationale a tenu compte en effet d'un certain nombre d'avis et a remis les crédits du Fisac à leur niveau de 2017 à 16 millions d'euros de d'engagement, c'est ceci s'accompagne également d'une forte hausse des crédits de paiement, ce niveau est désormais calibré pour soutenir les 200 projets qui nous semble une bonne enveloppe pour pour l'année 2018 par ailleurs, comme je l'ai indiqué les stations-service de maillage constitue toujours une priorité merci. de 2 amendements, y compris celui de la Commission. Il y a 2 demandes de prise de parole d'abord Monsieur Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs moi j'apporterai mon soutien au repos à l'amendement de monsieur pointeront pour plusieurs raisons : d'abord la 1ère c'est concernant les stations-services, le bon sens aurait voulu qu'avant d'être obligé d'utiliser des fonds publics pour réouvrir des stations-service, on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en place des normes moins drastique pour toutes les fermer, parce qu'en milieu rural, on en a plus fermé pendant 20 ans que ce qu'on a été capable de comprendre comment il fallait un. Et que je pense qu'il aurait été bien plus malin de se poser les bonnes questions de savoir comment on aurait pu préserver les stations-service local plutôt que de les fermer dans un 1er temps et remette de l'argent public pour un réouvrir souvent par le biais des communes qui sont plus occupés, obligé de se sont occupés de la gestion de tout cela, le 2ème élément, en terme d'appui à cet amendement-là c'est que nous avons fait remonter madame la Ministre, entre 2014 et 2017 près de 17 millions d'euros de leaders non consommés et quand on sait que le leader pour mieux consommer, il faut pouvoir le co-cofinancer et que dans les cofinancements

Madame la présidente, madame la ministre, bien entendu, je soutiens totalement l'amendement de monsieur trop et je suis tout à fait d'accord et ce qu'a dit monsieur Karoutchi choses marchent à mon avis il faut mieux gardés et élu du du rural et pas du tout de, de, de, de la ville, j'ai constaté chez moi et ailleurs, que le Fisac était très, très intéressant pour développer ou tout au moins pour maintenir les quelques commerces qui nous reste et puis pour les stations-service, on est en train de prendre de l'aspirine pour une grave maladie, parce que la grave maladie c'est l'énorme et surtout le prix libres et qui fait que le produit d'appel pour les supermarchés, c'est un produit d'appel, le carburant et bien entendu les petites stations ne doit pas vivre. Merci Monsieur, monsieur Bourquin la parole. Oui, madame la présidente, chers collègues, Madame la Ministre, le, le Sénat a mis en place une commission de revitalisation des centres-villes et centre bourg. Le constat est épatant. L'ensemble de nos centres-villes nous Centre Bourse dévitalisé dangereusement. Il y a des millions de m2 qui sont en préparation, d'ouverture et plusieurs questions se posent. La 1ère c'est est-ce qu'il ne faut pas un moratoire, pas un moratoire général avoir des voyant qui s'allume lorsque, il y a trop de grandes surfaces qui s'installent et qui dévitaliser les centres-villes, les centres bourgs, ça c'est le 1er point le travail de de cette commission viendra devant le Sénat dans peu de temps, mais il y a aussi des actions à mener avec les maires, les communautés de communes des communautés d'agglo pour justement faire en sorte que les opérations de revitalisation. Et ces opérations de revitalisation, elles sont sur le bâti bâti et sur les politiques de logement de peuplement des politiques de service des politiques d'équipements structurants dans les centres-villes et centre bourg et le Fisac est un levier indispensable pour mener ces politiques-là sans Fisac, ça ne sera même pas suffisant et moi j'aimerais plutôt qu'on ait une querelle pour savoir fusionnons comment les les 2 amendements parce que au dessus de la valeur de de 20 millions d'euros parce que ça ne sera pas suffisant et si l'on veut mener une politique à un haut niveau, faisons en sorte de nous retrouver et de voter que le Sénat, et ça sera un bon début pour cette mission que vous avez confié à Rémy-Cointreau et à moi-même et avec toute une série d'autres sénateurs et sénatrices, ça sera un bon début de dire on commence avec ses 20 millions d'euros et on essaye de d'inverser la tendance, il y en a qui disent que c'est fini, les centres-villes et centre bourg, nous, nous pensons qu'il ne faut pas baisser les bras et le Fisac et un de ses éléments. Merci monsieur Bourquin la parole à monsieur Oui merci madame la présidente, madame Luis moi je, je, je défendrai, je soutiendrai l'amendement de Rémy-Cointreau parce que vous savez quand on habite en dans le monde rural et que il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'activité même j'allais dire, même si encore vous avez un peu d'activité économique, industrielle, mais vous avez quand même une collectivité qui est vide, et je crois que Karoutchi l'a bien dit, il y a tellement de choses qui ne marche pas et pour lesquels on devrait regarder comment faire pour que ça marche, alors je vous en prie, arrêtons de s'occuper de ce qui marche et de mettre à la poubelle parce que et occupons-nous de ce qui va pas, je crois que le fils a quelque chose de fantastique, ça montrera aussi aux collectivités, hé bien tout l'intérêt qu'on porte au monde rural, tout l'intérêt qu'on porte au communes rurales tout l'intérêt qu'on montre à nos petites villes et tout l'intérêt aussi que l'on porte à nos anciens parce que je crois que nos anciens ne peuvent pas se déplacer comme ils le veulent, pour aller dans une autre ville, ou pour aller faire leurs courses ailleurs, alors s'il vous plaît, prenez-en qu'on ne sait, amendement qui est vraiment important et qui montrera la volonté de ce gouvernement d'accompagner les politiques que mènent les maires et les conseillers municipaux dans les territoires, merci. Merci Merci Monsieur bonjour Madame Espagnac, vous avez demandé la parole, mais est-ce que vous préférez pas d'apprendre une fois toutes les explications de vote passé. Alors je propose à monsieur Richard, de prendre la parole.

je voudrais militer en qualité d'abord de sénateurs pour cet amendement parce que, ici, nous représentons les territoires, nous représentons la ruralité nous représentons tout particulièrement aussi les collectivités locales dont c'est précisément une des compétences de pousser et de mettre en oeuvre les programmes de Redu Revit la revitalisation des bourses de revitalisation des centres-villes et de revitalisation, entre guillemets, de la ruralité, qui en a tellement besoin, il faut savoir qu'au point départ de Fisac, souvent il y a une collectivité locale, souvent il y a une petite commune qui a simplement envie de garder ses locaux commerciaux et qui précise pour relancer les opérations non seulement de revitalisation de l'artisanat, du commerce et des services, mais aussi de l'urbanisme alentour, bref une opération véritable de relance de de la revue de la revitalisation des collectivités locales, je voudrais aussi militer pour cet amendement en qualité d'ancien actuellement conseiller régional, ancien président de concert et je ne Alsace, ancien vice-président en charge de l'économie et aussi des fonds européens, je voudrais aussi dire ce qui a été dit à l'instant, à savoir que le Fisac joue le rôle détonateur pour le fond Leader mais aussi ce Fisac, encore une fois qui lie l'État joue un rôle de détonateur pour 2 leviers pour bénéficier d'aides du conseil régional derrière quelquefois des aides des conseils généraux maintenant départementaux et c'est par l'addition de ces forces naturellement que que l'on participe à un vrai projet et, enfin, je voudrais mettre mon ancienne casquette dans une vie antérieure, j'étais directeur général de la chambre des métiers d'Alsace, je peux vous dire que c'est un instrument tout à fait fondamental pour l'artisanat donc ici, on ne se rend peut-être pas suffisamment compte quand je dis ici dans les sphères qui qui qui nous parle de Fisac c'est véritablement mettre les, les, les doigts clairement dans les roues, âge de du développement artisanale, c'est de mettre les mains dans le cambouis et nous avons besoin dans les chambres de métiers, d'un outil de ce type, donc vraiment 20 millions franchement mais malgré les efforts faits par l'Assemblée nationale pour augmenter un petit peu la dotation initiale, ça me paraît franchement pas être exorbitant. Merci, Monsieur Richard, la parole est à madame Sophie Primas. Merci madame la présidente, madame la ministre, de vous demandons ici une petite rallonge sur le Fisac pour sauver le commerce de centre ville et vous avez entendu les plaidoyers de l'ensemble de mes collègues qui vont dans le même sens, moi, je voudrais vous. Vous proposez quelque chose qui coûte pas un Euro dans la loi hydrocarbure un amendement est venu imposer à l'ensemble des stations-service de France la double distribution de de carburant et de biocarburants alors ça part d'un bon sentiment, je suis désolé que les, les, les sénateurs de la République en marche ne ne soit pas là parce que, en obligeant. les stations-service de la ruralité à avoir. Une double distribution de carburants vous fermer tout de suite là. Pardon, pardon, pardon, chers collègues, certes collègues alors mon cher collègue. Au seul je vous fais avec madame la milice, porte-parole de ma demande, demandez à vos collègues de l'Assemblée nationale qui n'empêche pas l'ensemble des stations services de la ruralité à passer en double peu en double distribution de biocarburants, car vous êtes en train de faire mourir les stations-service et ensuite on demandera de l'argent Fisac pour les faire ressuscité. Oui. La présidente mais la milice, mes chers collègues, juste une minute. Sur cette opération et notamment sur les stations services, dans mon département, qui est un département extrêmement rurales, je rejoins ce qui a dit notre collègue longeant la petite commune de louer l'abbaye dans le bas du Domfront à la force des poignets et la volonté du maire a créé cette cette pompe municipale. Et je voudrais vous dire qu'en réalité c'est un effet d'entraînement parce que, une fois qu'il y a cette citation les gens viennent pour la station, ils viennent aussi pour les commerces de proximité extra, c'est-à-dire que, en réalité, c'est vraiment aussi un point d'attractivité en dehors du fait qu'on a. Absolument pas de transports en commun, je vous parle pas de de livrer par internet, quoi que ce soit, puisque de toute façon, on n'a pas de haut débit ni téléphonie mobile, donc de toute façon, il y a pas d'. Sujet mais en réalité, le fait de pouvoir fléché sur ce mariage de 2 stations de proximité, c'est vraiment extrêmement important et je pense que c'est une, c'est une vraie bonne idée pour l'attractivité du territoire, en plus de que pour l'utilité donc évidemment moi je voterai aussi l'amendement présenté par Roger Karoutchi. Merci Madame Goulet la parole à Cécile Cukierman. comme effet levier qui permet d'accéder à d'autres, à d'autres subventions à d'autres aides comme outil réel et qui reste encore janvie dire parce que il va y en avoir de moins en moins au service des élus locaux pour redynamiser dynamiser les centres, les centres villes, les centres bourgs, même si, et je vais le dire également, il n'y a pas que ça dans les politiques nécessaires à la redynamisation de nombreux centres centres-villes dans les années à venir, il y a bien évidemment besoin de d'agir sur les problématiques d'habitat et d'accueil de nouvelles populations mais en tout cas on ne peut pas fragiliser le développement économique que permet le Fisac, aujourd'hui, je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à être régulièrement d'ailleurs sollicité par beaucoup d'élus dans l'attente de réponses sur sur les demandes qu'il faut dire quand même, également, parce que même si on est dans un grand tout cuménisme 7 en cette fin d'après-midi sur cet amendement comme sur d'autres avant que bien évidemment, la problématique commerciale des des centres-villes et et des centres bourgs est aussi une réflexion que nous avons vont avoir plus globalement sur la problématique notamment du développement des centres commerciaux et compte dans un certain nombre de commissions départementales avec de nombreux élus locaux systématiquement des avis favorables sont donnés au développement à l'installation à l'agrandissement de grandes surfaces commerciales en périphérie de nos, de nos centres-villes nous ne contribuons pas quand même collectivement à redynamiser le commerce de centre ville de proximité auquel j'entends ici que nous sommes toutes et tous attachés en tout cas, nous voterons cet amendement pour abonder Fisac, même si sur cette mission comme sur d'autres, nous regrettons que la contrainte de l'exercice budgétaire au Parlement, nous nous oblige à accepter de les prendre sur de de les prendre ailleurs et donc de réfléchir à des missions à budget constant, alors que bien évidemment il faudrait pouvoir avoir une liberté un peu plus large dans l'exercice du débat budgétaire. Merci beaucoup, c'est Hermann, la parole est maintenant à Monsieur Morisset. Merci madame la présidente, madame le ministre j'ai apporté mon soutien à cet amendement pour plusieurs raisons : le 1er c'est que connaissant bien dispositif depuis plusieurs décennies, il a fait ses preuves dans nos zones rurales et je trouve dommage conviendrait effectivement l'fragilisée par une diminution des crédits ma ma 2ème raison, c'est que vous savez, madame le ministre, nos territoires, ils ont été bousculés dernièrement on a regroupé nos communautés de communes ensemble et je constate que dans beaucoup de communautés de communes, on engage une réflexion sur l'avenir de leur territoire et qu'est-ce qui leur retiennent en priorité, c'est la redynamisation des des commerces dans les centres bourgs, donc je pense que c'est une bonne raison de leur apporter aussi un soutien et puis Madame la Ministre, vous savez, 20 millions divisés par 100 départements, ça fait 200000 euros par département, vous nous dites que vous avez 200 projets sous on émet 200 projets divisé par son département ces 2 projets par département, donc je pense que 20 millions c'est même pas suffisant et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on vote cet amendement à 20 millions d'euros. Merci beaucoup, cher collègue. Alors je rends la parole maintenant à Madame Espagnac. Merci madame la présidente, je vais faire une proposition de pour aller dans le sens d'Inkermann et marcher un bouquin pour continuer sur le cuménisme plusieurs choses, non, ça peut arriver dans cette assemblée, on est plutôt et si je crois que c'est à l'honneur nos territoires de savoir nous retrouver sur ce genre de sujet, la preuve puisque nous sommes intervenus plusieurs les uns et les autres, on a tous connu dans nos petits villages, la fin du dernier commerce et j'ai envie de dire, quand enfin on arrive en réouvrir un grâce à un physique change le lien intergénérationnel, comme l'a dit Madame voulait que ça soit aussi une station d'essence, tout compte fait c'est redevienne paradoxalement le point de convergence de tous et de toutes et de la vie, surtout dans nos villages,

l'objet l'âme 2 sur le faisons pardon, seul l'amendement, donc de la commission d'immense permet d'aider sur les. Stations-service qui n'a pas été déclarés dans l'objet de du 1er amendement, ce qui poserait par rapport à tout ce que ce que vous avez souligné les uns et les autres, par rapport à la nécessité de pouvoir aider parce qu'on a dit tout à l'heure, les stations-service, ça ne serait plus possible dans ce cas-là, puisque on augmenterait le fond mais on ne pourrait plus permettre tout simplement malgré le l'augmentation du fonds la de stations-service, donc ce que je vous propose, attendez, vous allez voir, je vais dans votre sens, ce que je vous propose, c'est de monter la moment de la commission des finances sur votre somme, et donc de permettre à la fois une augmentation des crédits Fisac Emme alignant sur la proposition de monsieur Karoutchi et de permettent puisque l'objet de l'amendement de la commission des faits mais on se permet de pouvoir fessiers aussi l'utilisation sur les stations-service donc de trouver un accord commun est-ce que vous allez, d'accord, donc dans ce cas-là, nous retirons le vôtre si vous si, si vous en êtes d'accord et on permet donc en montant de venir sur votre sol et de permettre aussi de flécher les stations-service et donc de les aider, c'est vous qui voyez, c'est à eux, c'est, Alors je laisse la parole à monsieur Karoutchi. Oui, le climat facile limite c'est que par définition, la loi c'est pas de commentaire de la loi ni l'objet, c'est ce qu'il a dans le texte et par définition l'objet les motifs sont extrêmement intéressants, mais c'est pas ça qui fait la loi, ce qui fait la loi, c'est ce qu'on veut c'est pas le commentaire ou l'objet 2ème élément, il y a une chose qui me gêne un petit peu je du franchement c'est pas du tout qu'on aide les stations-service c'est un fléchage chiffrée parce que ça veut dire que sur l'augmentation en tout état de cause, on mettrait 5 millions quoi qu'il advienne sur les stations-service alors que. Notre idée, c'est plutôt de dire : laissez les collectivités décider de ce dont elles ont besoin ont besoin 6 CDD une station-service le font si c'est du commerce du centre le fond mais ne pas prendre d'office 5 millions alors que si ça se trouve, il y a pas de nécessité sur 5 millions et il y aurait plus de nécessité par ailleurs qui serait bloqués, moi je pense franchement

serait que le gouvernement ensuite à l'Assemblée nationale ne fassent pas en sorte que cette cuménisme de la haute assemblée, soit ne communisme de la Chambre des députés, mais contre nous. je. Alors avant de passer au vote, il y a une demande d'explication de vote de Madame Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, moi je pense qu'on ne peut pas philosopher sur la ruralité vouloir un développement équilibré de nos territoires et approcher chacune des politiques qui constituent nos territoires en terme de silos pour rogner le crédit comme on l'a vu hier sur le logement avec le PTZ et comme l'on voit aujourd'hui avec le Fisac aménager le territoire, je suppose, d'avoir une politique dans toutes les dimensions et dans toutes les composantes et on sait combien l'activité commerciale et la vitalité du commerce de centre ville est un élément qui structure le territoire non seulement la petite ville où la ville moyenne

que la chambre qui représente les territoires ne peut pas entendre le président de la République au congrès des maires, dire je vous ai compris je connais votre territoire fait des rêves fous oser et et se voir chaque jour ici sabrer les crédits qui permettent vraiment de garder du dynamisme dans les territoires et de ne pas avoir décroché la ruralité et qu'en matière de commerce, il vaut mieux éviter de perdre une guerre il s'agit là de faire de la prévention et je pense que le Fisac s'il sauve le dernier commerce, il permet aussi d'empêcher la dévitalisation des commerces des villes moyennes et des petites villes, parce que quand on en est à sauver le petit commerce, il est souvent beaucoup trop tard, donc, de grâce, Madame la Ministre, arrêtons d'être hors sol et Hortefeux dogmatique si nous aimons nos territoires si nous croyons à l'équité d'un développement équilibré, hé bien, de grâce, aujourd'hui, écoutez-nous. Merci Alain Gastal, monsieur Reina. Oui, Jacques Olek, je, je crois que sur le fond, il y a pas, il y a pas de difficulté simplement sur la forme, quel amendement retenons-nous selon l'ordre dans lequel il est paru,

Je vais vous dire, on l'a fait 10 fois la depuis qu'on est en mission, on s'est mis d'accord sur une partie d'amendements communs bon, heureusement, on l'a fait, chaque fois que nécessaire, donc ce qui est intéressant avec l'amendement de la commission des finances de retenir l'amendement de commissions des finances et que par nature, il regroupe tout le monde

ça peut exister l'élégance que les signataires du premier amendement se remettent sur celui de la commission des finances, oh, je vous rassure, vous êtes majoritaires il y a pas de problème et qu'on vote l'amendement de la commission des finances, c'est plutôt comme ça que l'on fait voilà après vous choisissez. Merci monsieur Raynal la parole à Madame Espagnac. dans l'état actuel ne permet plus d'aider les stations d'essence. Donc, si ce n'est pas spécifié monsieur Occident l'amendement, on ne pourra plus les aider tout simplement, donc c'est pour ça que j'aurais insiste : ce n'est pas une question de loi ou pas loi, c'est que dans la situation actuelle, le système d'attribution des aides pour les stations-service est caduque depuis le mois de juillet, donc si nous augmentons la somme et que ce n'est pas spécifié dans l'amendement nous ne pourront tout simplement plus aidés non pas infléchi à 5 ou pas 5 on ne pourront tout simplement pas aidé du tout, les stations d'essence, c'est pour ça que je me permets de reprend la parole. Donc. Je pense que là il y a eu des explications sur. Monsieur Karoutchi pour si vous prenez la parole, c'est pour retirer. Donc.

c'est que l'on dise ce que l'on crée à l'intérieur, un fonds pour les stations-service sans mettre une somme, c'est-à-dire ce qui me gêne, c'est que l'on dise il y a forcément 5 millions si, en revanche, on dit on est tous ok pour 20 millions en plus et à l'intérieur, on accepte la création d'un fonds, ce qui permet éventuellement de faire sur les stations-service sans fléché un chiffre c'est d'accord. Donc. Madame Espagnac pour explications et dire si cette modification peut-être apporter à l'objet et si j'ai bien compris. Tout à fait, donc évidemment il n'y a aucun souci, la question n'était pas de flécher telle ou telle somme, c'est de pouvoir tout simplement rendre éligible au crédit Fisac, l'aide aux stations-service de l'amendement de la commission monte sur la somme qui vous aviez proposé et donc nous trouver un consensus global qui permet d'en sortir par le haut et puis uniquement pour chacun d'entre nous, dans l'intérêt nous territoire nous sommes d'accord, monsieur Karoutchi. Alors. Pour essayer de synthétiser cet échange, hé bien s'assurer que tout le monde sera satisfait si je comprends bien, c'est l'objet le montant, nous sommes d'accord, c'est 20 millions l'objet à ce moment-là, il faudrait le modifier dans la 2ème page de l'amende de, de, là où il écrit sur c'est 17 millions d'euros. 5 millions d'euros serait à un fonds spécifique d'aide aux stations service de proximité serait créés, on met ça à la place de ces sur 7 17 millions d'euros, 5 millions un fonds spécifique d'aide aux stations service de proximité seraient c'est la phrase qui remplacera la première phase trace de ce 3ème paragraphe, on est bien d'accord. C'est 20 millions. On est d'accord, c'est indiqué, ce qui est important, c'est le fonds spécifique d'aide aux stations services de proximité. madame la prison s'il faut en fait une petite suspension de séance, on se met d'accord. Voilà la présidente si vous autorisez. Alors Madame Espagnac ne sort enfin une petite suspension pour écrire les choses proprement si voulez Madame Espagnac. On va dans le sens, donc ce qui a été proposé, c'est de dire tout simplement dans l'objet que les stations ces 2 services seront éligibles au au au au Crédit Fisac allait de crédit FISA. Donc nous sommes sur la somme proposée par monsieur Karoutchi et dans ce cadre là dans l'objet, nous mettons bien que les stations-service seront à partir de maintenant éligible au fonds Fisac. Très bien, on en reste là, on indique simplement l'éligibilité des stations-service terminé dans l'objet et donc si nous en sommes d'accord, l'amendement de monsieur Karoutchi est retiré la main et l'amendement de la commission, donc est le 229 rectifier va être maintenant soumis au vote. Et et pour cet amendement rectifier. Avec 20 millions bien sûr Il est défavorable aux 2 de toute façon. Favorable qui est contre. Qui s'abstient, cet amendement est adopté à l'une anémie. Nous passons à l'amendement 444 représentée par Madame Goulet. La présidente avec votre autorisation, je défendrai bien de 519 en même temps, images gagnerait un petit peu de temps parce qu'en réalité il y a une connexité je je vous ai indiqué brièvement tout à l'heure. Je vous ai indiqué totalement tout-à-l'heure brièvement et on en a parlé avec le rapporteur spécial, l'efficacité de de Business France et aussi le fait. Il manquait à Business France des moyens donc dans la première amendement, je vous propose des moyens financiers et dans le second, je vous propose des moyens en équivalent temps plein, c'est-à-dire des moyens humains, il est parfaitement évident aujourd'hui que les besoins et les demandes, notamment en matière de de promotion de nos entreprises sont multiples et lorsque vous avez un bureau de Business France à Moscou, qui doit couvrir l'ensemble de l'Asie centrale, voire le Caucase, les gens ont pas la possibilité d'ubiquité ils ne peuvent pas rendre les services qui sont attendus, alors qu'en réalité, les opportunités sont multiples, donc le 1er amendement, je vous propose d'abonder le fonds pour 20 millions d'euros et le second de transférer des moyens humains d'une délégation qui est en fait des des postes dont on ne connaît pas exactement l'efficacité, mais peut-être que le ministre pourra nous donner des explications sur les 664 équivalents temps plein de la direction générale du Trésor qui sont situés à l'étranger,

qui est de renforcer Business France. Madame la présidente, Madame la Ministre, nous nous partageons l'analyse qui a été faite par notre collègue néanmoins : en même temps il y a en ce moment, un rapport qui est déposé auprès du gouvernement du responsable de Business France comme nous n'en connaissons pas non plus la teneur en ont certainement qu'on la ministre nous en donnera quelques peut-être quelques éléments, nous pensons que nous devons attendre ce rapport pour savoir quelles sont les équilibres financiers proposés par le directeur de Business France avant de, de, de donner des crédits supplémentaires, néanmoins, nous sommes extrêmement, extrêmement vigilants sur cette question et nous dans un à la commission des finances propose dans un autre, par un autre amendement, de pouvoir faire un rapport beaucoup plus globale sur la position de Business France qui tiendra compte des éléments financiers que vous proposez Madame Goulet, donc moi ce que je vous propose ma chère collègue, c'est de retirer vos amendements de de reprendre tout à l'heure, les propositions qui sont faites par la commission des finances sur un rapport général dont vous avez soulevé tout à l'heure les les le besoin je vous remercie.

sur le, sur l'amendement qui qui augmente les crédits de de Business France je rappelle que, en effet, Business France est engagée dans une évolution profonde et positive de son modèle d'affaires et de financement Business France va augmenter la part de ses ressources propres des progrès importants ont déjà été réalisés puisque ces ressources sont passées de 45 à 49 pourcent de ses ressources totales en 3 ans, l'objectif de ces réformes, ça vise à toujours mieux répondre aux demandes des entreprises exportatrices évidemment et c'est : c'est l'objectif de la mission qui a été confié à Christophe Lecourtier le Nouvel, le nouveau directeur général, les propositions de réforme du dispositif de soutien à l'export que monsieur le courtier a remis à ses tutelles implique notamment la création de nouveaux outils digitaux, notamment pour mieux servir les entreprises, ce qui supposera des investissements de court terme, elle implique aussi une rationalisation des dispositifs et une meilleure articulation entre les différents intervenants du coup une évaluation du du coût des investissements doit encore être menées avec l'ensemble des acteurs au 1er rang desquels Business France en tenant compte des marges d'efficience collective qui seront dégagés par une meilleure organisation de l'ensemble du dispositif, les financements que cette réforme rendrait nécessaires seront identifiés au terme de cette réflexion aujourd'hui l'ouverture de crédit que propose le cet amendement apparaît comme prématuré. et, en outre, le le gage qui est qui est proposée sur les dépenses hors personnel de l'INSEE serait. Extrêmement douloureuse puisque les crédits de l'INSEE s'élève à 61 millions d'euros pour les autorisations d'engagement et à 52 millions d'euros pour les crédits de paiement, l'amendement reviendrait donc à amputer d'un tiers les autorisations d'engagement de Lindsay et de 40 pourcent ces crédits de paiement, ce qui est clairement insoutenable. Sur l'aspect ma salariale du programme 305 donc il s'agit, Damas Apple salariales de la direction générale du du Trésor, elles augmentent de 4 millions d'euros, entre la LFI 2017 et le PLF 2010. Suite mais cette augmentation se fonde sur les prévisions d'exécution 2017 et résume pour l'essentiel, de facteurs exogènes, notamment la variation de l'indemnité de résidence à l'étranger des à des agents expatriés qui est indexé sur le cours de l'Euro, lequel a connu une baisse en 2017 et de mesures de transfert de service. Il convient de rappeler que programme 305 supportera 24 suppressions de postes en 2018 soit 1,5 pourcent du plafond d'emplois de 2017 dont 21 à la DG Trésor 3 à la direction de la législation fiscale. Donc, pour ces raisons-là, nous souhaitons également le retrait de cet amendement, tout comme du précédent merci. Merci madame la ministre Madame Goulet vous êtes sollicité par la Commission et le gouvernement pour un retrait de vos amendements. Je comprends bien, je qui justifie le retrait moi-même régulièrement demande rapports, on attend des résultats etc, mais enfin je le dis, assez souvent, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon texte et et et on arrive finalement pas avoir de moyens en attendant, il faudra encore une année budgétaire pour avoir des moyens supplémentaires pour Business France et pendant ce temps-là, nos entreprises sont à la dérive et essaye de, de, de s'implanter à l'étranger ou en tous les cas de répondre aux besoins dans la, dans le même temps, Ubi Business France est complètement débordés et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avancer dans l'art, qui manque de moyens humains et bon j'ai bien, j'ai bien conscience que c'est que ces amendements répondront pas à cette nécessité, mais en même temps, il faut trouver une solution intermédiaire, comme on va répondre aux besoins, donc il faudra pas s'étonner l'année prochaine dans la même mission, qu'on a les mêmes résultats, donc je vais retire mais franchement, c'est un très très mauvais signal. Nous. Sont à l'amendement 562 rectifier qui est présenté par monsieur petit. Non

les membres du groupe socialiste, notamment la protection économique du consommateur est l'objet de l'article 17 du PAM 134 elle comporte des dépenses d'intervention en faveur de la Suisse national de la consommation de 15 associations de consommateurs du Centre européen des consommateurs français et du Centre de recherche pour l'Étude et l'Observatoire des conditions de vie, le Crédoc, les 15 associations nationales agréés qui siège au Conseil national de la consommation travaillant proximité au quotidien auprès des consommateurs en faveur de l'accès et au droit et à l'information juridique en droit, la consommation ainsi que pour le règlement amiable des litiges, ces associations jouer également un rôle crucial dans l'éducation et l'accompagnement du consommateur au travers des études et des analyses qu'elles produisent dans de nombreux cas, ils ont joué un rôle de lanceur d'alerte à ce titre, on peut citer leur combat contre l'obsolescence au programme où les révélations autour des médicaments comme le Levothyrox, le la dépakine le monde de la consommation est actuellement en pleine mutation, les consommateurs ont besoin d'informations, de conseil d'orientation pour faire des choix éclairés et indépendants pour aujourd'hui et pour demain sans ces associations, ce sont des missions de service public qui disparaissent sur l'ensemble du territoire national, le PLF 2018 prévoyait initialement la diminution des crédits intervention de 40 pourcent soit environ 2000 lions 200000 euros lors de l'examen à l'Assemblée nationale a permis de majorer ses crédits d'intervention de 1,9 millions d'euros, ramenant la baisse à 5 pourcent au lieu des 40 pourcent initialement prévus ces insultes stations ont déjà fait l'objet de nombreux efforts ces dernières années pour maintenir les leur activité au service des consommateurs à la suite de ces diminutions successives qui ont pu être constatées au cours de ces dernières années, toute nouvelle baisse de financement aurait pour effet irréversible. Des effets irréversibles sur l'existence et l'organisation de leur implantation de leur maillage territorial et l'émission qu'elles assurent au quotidien pour que ces structures demeurent en capacité d'accompagner les consommateurs dans les défis résultant des différentes transitions économiques, énergétiques numérique environnemental et social, il est proposé de maintenir leur subvention au niveau actuel, soit 5,4 millions d'euros, donc proposé de majorer de 300000 euros, les crédits d'intervention en faveur de la protection économique du consommateur, telle que prévue à l'article 17 du programme 134.

permettant de remédier cette baisse à seulement 5 pourcent afin de préserver les moyens et donc l'indépendance des organismes sans pour autant remettre en cause la nécessité de réaliser des économies de fonctionnement, le gouvernement avait donné un avis favorable à cette atténuation il semble donc non pardon, il semble donc nous partageons tous Parlement comme gouvernement une même préoccupation à cet égard, pardon, excusez-moi, déjà adopté par les députés, nous proposons de demander l'avis du gouvernement quant au montant de l'amendement proposé. Merci beaucoup du gouvernement Madame la ministre. Merci madame la présidente, madame rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs, en effet, ça été rappelé le gouvernement. à soutenu l'Assemblée nationale dans sa décision d'abandonner les subventions aux associations consuméristes à hauteur de 3,1 millions d'euros ceci traduit bien l'attachement que le gouvernement porte à la protection des consommateurs, indispensables pour préserver leur confiance et au bon fonctionnement des marchés mais nous considérons que, il n'est pas opportun d'aller au-delà de cette remise à niveau qui limite la baisse des subventions à seulement 5 pourcent et permet d'envoyer un signal vers une meilleure efficacité de cet écosystème donc nous suggérons le le retrait de cet amendement, sinon le rejet merci. Merci madame la ministre, la commission qui vient d'avoir l'avis du gouvernement défavorable comme le gouvernement. On a demandé l'avis du gouvernement Madame oui tout à fait, Même avec le gouvernement, donc défavorable de la commission du gouvernent et du gouvernement si retrait de l'amendement monsieur Joly, maintenez-vous votre amendement. L'amendement est maintenu, nous allons donc le mettre aux voix qui est pour cet amendement. Qui est contre. Cet amendement n'est pas adoptée qui s'abstient nous allons procéder au vote des crédits de la mission outre-mer figurant à l'État B. je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mets donc on voit les crédits de la mission. Qui est. Qui est contre. Qui s'abstient. Les crédits de la mission sont adoptés, j'appelle en discussion : les articles 57 quater c'est les amendements qui sont rattachés pour leur examen au crédits de la mission économique. Article 54 qui-ce l'amendement 227. Présenté par monsieur de Montgolfier. Mais le président place de ministre mais, chers collègues, la commission des finances vous impose de supprimer l'article 5 54 qu'inquiet, ce qui constitue le comble de l'horreur budgétaire puisque toute simplement on vous cherche à contourner un plafond en créant l'imagination est au pouvoir, une comme volontaire obligatoire des entreprises, donc de manière très concrète, l'AMF a des besoins de d'argent qui sont parfois léger, certes légitime ce qui normalement aurait dû conduire à relever son plafond de ressources, et au lieu de faire ça, hé bien on fait quoi, on supprime une contribution obligatoire via une taxe et on la remplace par une contribution volontaire obligatoire, donc vous imaginez l'imagination et donc donc il vaut bien mieux revenir à la l'essentiel c'est-à-dire concrètement considérer que si l'AMF a des besoins financiers, hé bien, il suffit de relever le plafond de l'AMF, le plafond des ressources affectées, fixé à 94 millions d'euros pour 2016 et donc je vous pose de supprimer cet article sinon on arrive à des artifices budgétaires sans limite et demain on pourrait peut-être supprimer les impôts et remplacer par des contributions publiques volontaires obligatoire des conditions voilà donc donc voyez que je pense qu'il vaut mieux mettre face et plaisanteries et a invité le gore ne m'en a donné à l'AMF les moyens dont il a besoin, en relevant le plafond d'emplois et en le fixant à la hauteur des besoins de l'AMF. Merci monsieur de Montgolfier la parole à la Commission à l'avis du gouvernement pardon. Merci madame la présidente, mais si mesdames et messieurs les sénateurs, cet amendement proposé par la commission des finances en supprimant la possibilité pour l'AMF de prélever des contributions volontaires non obligatoire priverait la messe de ressources pour faire financer des investissements exceptionnels qui contribue à l'attractivité de la place de Paris et que les acteurs concernés sont prêtes à financer, au moment où la concurrence entre places financières bat son plein dans le contexte du poste Brexit c'est un mauvais service à rendre à l'attractivité de la France, je rappelle qu'il s'agira par ces contributions de financer des projets informatiques ponctuelles et d'intérêt commun qui ne touche absolument pas aux missions régaliennes de l'AMF l'autonomie financière de l'AMF dans ses missions régaliennes, n'est pas remise en cause ce panachage entre contributions obligatoires ajustée et contributions volontaires nous paraît donc constituer la solution la plus équilibrée qui, sans remettre en cause le niveau structurel des ressources de l'AMF permettra de lui ménager les marges de manoeuvre budgétaire budgétaire dont à la ponctuellement besoin je vous remercie.

si les entreprises effet d'aubaine décide de ne pas verser leur contribution, concrètement, il y a moins de ressources, puisque les entreprises ne verse plus ce qui était normalement obligatoire Moselle sur 1300 très contente et si ensuite des entreprises ne versent pas leur contribution volontaire, hé bien il y a de fait une baisse des ressources pour l'AMF, donc on est ici dans un contournement d'un arbitrage budgétaire qui était perdue, c'est ça, il faut d'avoir gain de cause sur l'arbitrage budgétaire, hé bien on préfère contourner la décision de l'arbitrage budgétaire Anna votants ce mécanisme un peu tordu, on vous supprime un impôt et à la place, vous contribuerez volontairement, si on fait ce mécanique sur tous les Français, je pense qu'il serait d'accord supprimant les impôts en plaçant sa par des contributions volontaires,

en toute transparence, le montant de le plafond des ressources affectées à l'AMF et ça va être comme vous le souhaitez Maddaloni ce que l'AMF puisse assumer ses missions. Alors Madame la Ministre, vous souhaitez la parole en réponse de monsieur, il y a Madame Goulet avant, ou vous préférez madame Boulet, d'abord, ensuite une réponse générale Madame rouler. Madame rouler. Madame, mais la ministre, moi je voulais simplement dire. Une une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance, on allait évidemment soutenir l'amendement du rapporteur général. Merci, cher collègue, madame la ministre en réponse. Merci bien alors d'une part, une précision en effet le le le plafond et n'est pas baisser, c'est simplement une modulation qui est qui et il y a 94 millions de crédits par taxe affectée pour un besoin de 6 millions d'euros par contribution pour par les, les, les chiffres sur la table, simplement, en effet, on a besoin de ces 2 façons de financer l'AMF de telle sorte qu'on tienne la contrainte budgétaire, mais qu'on réponde à ses besoins ponctuels. Merci Merci pour ces précisions précisions Madame la ministre, monsieur Karoutchi pour explication de vote. Je suis béotien en la matière, mais je suis admiratif devant une contribution volontaire dont on sait déjà que c'est 6 millions d'euros, alors c'est une contribution volontaire fixé c'est c'est très joli, c'est une autre Monsieur Karoutchi. S'il n'y a plus d'explications de vote l'amendement présenté par Monsieur de Mongolfier au nom de la commission défieront n'annonce pas un avis défavorable du gouvernement et nous allons maintenant le mettre aux voix qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement était adopté et l'article est supprimée. après l'article 54 qu'inquiet s'nous tous, hommes à l'amendement cette 118 présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, alors cet amendement tire les conséquences de la suppression par le PLF 2000 2018 à compter du 1er janvier 2018 de la paix taxes fiscales qui alimente le fonds national de promotion et de communication de l'artisanat FNPC cette taxe fiscale affectés représente une contribution de 11 euros par an pour chaque entreprise artisanale, la suppression de cette taxe comportera 2 fois des facto la suppression du FNPC or depuis sa création en 1997, le FN PCA a contribué à installer durablement dans l'esprit du public une image positive de l'artisanat, nous souhaitons permettre une continuation des actions de communication menée et pour ceci, un mécanisme de substitution compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré il reposera sur une contribution privée porté par un organisme privé, cet amendement qui vous est proposé habilite les organisations professionnelles d'employeurs à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales merci.

c'est absolument génial, on a enfin trouvé le moyen de faire baisser le taux des prélèvements obligatoires en France, on va supprimer les impôts, les taxes affectées et on va les remplacer par des contributions volontaires obligatoires, donc moi je prendre tous les trucs, l'habillement, le cuir, le machin, tous ces trucs financés par les taxes obligatoires et à la place, je vais vous êtes des contributions volontaires obligatoires, c'est pas la fiscalité, c'est merveilleux, le taux de prélèvements obligatoires de la France va baisser, donc supprimons tous les impôts toutes les taxes et à la place, mesdames et messieurs, vous n'avez plus payer d'impôts plus près les modulateurs : vous avez pris des contribution volontaire obligatoire, donc voilà, donc bon sagesse parce que ça change strictement rien sur le fond,

là, elle sera obligée de payer, parce qu'une contribution volontaire obligatoire, donc l'imagination est au pouvoir de le seul impact de cet amendement, la ressource est exactement la même sexe abus diminue artificiellement le taux des prélèvements obligatoires en France mais ça me donne des idées, je vais en enfer sur l'habillement, le cuir, le bois, j'ai plein d'idées pour le le PLFR et vous verrez que comme ça on pourra diminuer le taux de prélèvement en France qui a des plus élevés au monde, donc sagesse. Alors nous avons donc un avis de sagesse de prix qui vient d'être précisé. Par monsieur le rapporteur général, madame la ministre voulait apporter une réponse à l'intervention

pour décider de même des actions de promotion de leur métier, donc c'est vraiment une mission qu'ils sont, qu'ils sont volontaires pour reprendre et qui, qui, me semble-t-il, peut relever l'initiative privée.

pour les artisans pour les entreprises et donc là il y a donc un nouveau fonds qui va prendre en mains un outil qui va utiliser qui va faire de la promotion pour l'artisanat, enfin il y a des chambres de métiers de l'artisanat, il y a, il y a plein d'autres choses qui font la promotion de l'artisanat, j'avoue que je comprends pas tout à fait, on est dans une complexité totale et je pense qu'en terme de choix budgétaires, il faudrait peut-être regarder tout ça. Donc s'il n'y a plus d'explications de vote, je vous propose de mettre aux voix, cet amendement, qui bénéficie d'une sagesse de la commission des finances,

Qui est contre. Qui s'abstient, l'article 54 7ème est adopté, nous arrivons à l'article 54 obtiennent. Et nous avons un amendement 228 qui est présenté par Monsieur Lalonde au nom de la commission des finances, Monsieur Merci madame la présidente, je je reviens sur le Madame la Ministre, je reviens sur Business France, et en particulier sur les différents propos qui ont été tenus par nos collègues, surtout les bons et transpartisan pour constater une chose évidente dans notre pays, il y a un déficit structurel du commerce extérieur, il y a été créé une force de frappe avec Business France à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme l'a dit excellemment notre collègue, il y a des dizaines et des dizaines de d'organismes de et et y compris d'ailleurs quelquefois dans nos propres commune nos propre département où nos propres régions, des spécialistes de l'export, voire un ou 2 quelquefois des services, chacun dans son secteur, essayant d'être le meilleur pour son territoire donc à l'extérieur, nous avons une force de frappe et à l'intérieur, une multitude de force de frappe, autant dire une dispersion, hé bien, en matière de crédit, c'est exactement la même chose, on disperse les crédits en fonction du nombre d'intervenants dans le commerce extérieur, un déficit extraordinaire structurelle, il est donc peut-être temps de se poser la question. Au travers d'un rapport il y a-t-il une relation directe entre un 1er de cordée à l'extérieur et une multitude de 1er de cordée à l'intérieur. Elle y a-t-il quelque part quelque chose à faire entre tous ces acteurs, nous croyons que oui et nous sommes donc demandeurs d'un rapport et en tout cas d'une mission qui nous permettrait d'évaluer véritablement cas quelles sont les synergies ou les inerties de tous ces gens qui interviennent et qui à la fin de la fête n'ont pour résultat d'accord que un déficit, ils ne sont pas tous responsables, il y a dans notre pays une une hypocrisie qui elle aussi est structurelle la fête les 100 entreprises les plus importantes de France avec condescendance, dit : nous allons nous préoccuper des PME ou des jetés, et on va les aider à à exporter, je rappelle quand même que les jeter et les PME, une grande majorité d'entre elles sont les sous-traitants déjà ceux des entreprises qui sont adhérentes de la autant dire en fin de compte, que l'on demande en fin de compte à son sous-traitant de dépendre de de son de l'entreprise principale pour avoir une idée de l'exportation, quand votre Chivres-Val affaire dépend de 30 ou 40 pourcent de d'une grande entreprise vous velléités à l'export passe quand même par infiltrant celui de votre donneur d'ordre et d'un autre côté, nous qui avons la préoccupation permanente des PME nous avons démultiplier un nombre d'intervenants sur nos territoires, pour leur donner des conseils, les PME et les jeter, ils sont entre les 2, la multitude de conseils et la fête conclusion des courses, nous n'avons pas une véritable politique de l'exportation pour nos grandes zones

une opération un commando réel qui aura les moyens de pouvoir porter les couleurs de la France à l'export avec des PME et des qui ne dépendront non pas non pas de la fête ou de une multitude d'organismes mais bien d'une organisation centralisée sur l'exportation, merci. Merci, monsieur le rapporteur, avis de madame la ministre, pour le gouvernement. que les évolutions qui pourraient être envisagées porteront entre autres sur une meilleure articulation de Business France avec les CCI et donc nous pouvons être d'accord avec le fait de présenter une partie de rapport sur ce sujet. Merci beaucoup, madame la ministre, je Madame Goulet a demandé la parole. Moi je vais je vais soutenir je soutiens des amendements mais mais je voudrais quand même vous dire madame la ministre, monsieur le rapporteur, que si ce rapport ne fait pas une autopsie du nombre d'intervenants dans la chaîne qui conduit à l'exportation ou aux relations économiques je, moi je connais très bien, plusieurs secteurs et je peux vous dire que le nombre d'intervenants est quand même très inversement proportionnelle à leur efficacité, je vous parle pas des consultants de-ci de-là qui parle pas la langue du pays, ni ce qui se greffe comme les ouvriers de la 25ème heure à partir du moment où ça fonctionne sans compter ceux qui interviennent pour empêcher que ça marche parce que l'idée tient pas de donc j'espère que la foi parce que cette histoire de rapport, on l'a déjà eu, moi ça fait 10 ans que je siège et ça fait 9 ans que je plaide la même chose bon, donc il faut que ce rapport soit complet, mais surtout qu'il soit suivi d'effet, donc moi j'ai voté cet amendement maintenant que je suis à la commission des finances excès mon dernier mandat, vous allez entendre parler de cette affaire. Merci Madame Goulet, pas d'autres prises de parole donc sur cet amendement, qui bénéficie d'une sagesse du gouvernement. Présenté par monsieur Lalonde donc sagesse du gouvernement qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient. L'amendement de la commission et. Adopté nous

cet article 54 obtiennent est adopté. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits du compte spécial prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés figurante à l'État,

Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit avec cet amendement, de nous mettre en cohérence avec le vote exprimé ici même il y a une semaine sur un amendement du gouvernement que nous avions rejeté amendement qui prévoyait de prêter 1 milliard 700 millions d'euros, la société qui qui va porter le projet du Charles-de-Gaulle Express, je vous rappelle qu'Charles-de-Gaulle Express est une liaison directe entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le prix du billet est évalué aujourd'hui à peu près à 27 euros l'aller simple qui s'adressent donc uniquement voyageurs internationaux, il ne s'agissait pas pour nous de remettre en cause l'intérêt de ce projet défendu par ADP mais de souligner une incohérence et d'exprimer une grande inquiétude puisque depuis plusieurs semaines, le gouvernement laisse filtrer des informations qui remettent en cause la réalisation de l'ensemble du métro du Grand Paris Express telle qu'il a été l'objet d'un accord entre toutes les parties en 2011 accord confirmé en 2013, avec un engagement également sur le calendrier, donc on remette en cause la réalisation en particulier, la ligne 17 une 18 dans les délais prévus, au prétexte que cela aurait aggravé les ratios d'endettement de notre pays et ses engagements dans le cas de ce engagements européens, on nous propose de prêter 1 milliard 700 millions donc d'aggraver ces mêmes rations à une société de projets qui ne dit par ailleurs qu'elle n'a pas besoin de cet argent de la part de l'État, qu'elle avait son plan de financement bancaire, on peut d'autant plus facilement la croire que, aujourd'hui, les taux sont encore particulièrement favorable pour la rédaction de de cette opération, donc il s'agit d'exprimer notre incompréhension d'une part la nécessité de prêter 1 milliard 700 millions n'ayant reçu aucune explication là-dessus et, d'autre part d'appeler très fortement le gouvernement à nous rassurer à répondre très vite sur la réalisation de la totalité du projet du métro du Grand Paris, étant entendu que cette confirmation devait être donné en octobre puis en novembre puis en décembre, nous attendons toujours s'est assez pense donc, je crois qu'il est utile à travers ce vote de confirmation de notre décision de la semaine dernière d'interpeller fortement le gouvernement sur ces 2 questions : pourquoi prêter 1 milliard 700 millions ce n'est pas nécessaire et, d'autre part, pourquoi envisager untel financement alors que nous ne sommes pas garanti et c'est notre volonté de l'être de la réalisation de l'ensemble du métro automatique du Grand Paris, merci.

Merci beaucoup madame la Ministre.

Madame la présidente, la ministre, tout simplement pour soutenir cet amendement du de mon collègue Bazin. Il y a une incohérence aujourd'hui. à interdire à toute la banlieue à tous les provinciaux de venir à Paris, en bloquant les circulations et en ne prévoyant et en ne prévoyant pas d'autres modalités de transport, or à l'appel que vient de faire notre collègue le sénateur Bazin par son amendement, c'est bien celui de développer les transports en commun et il nous dit, à juste titre qu'on ne voit rien venir, on ne voit que des partout dans tous les investissements et les assises ou de la mobilité se sont transformées en assassinant et en immobilité et donc cet amendement c'est un amendement effectivement d'appel car nous voulons tous que Roissy soit desservi par seul moyen de transport, mais fait aussi un effort pour les autres. Madame la ministre, madame la présidente, je je comprends bien l'amendement de mon collègue Bazin je ne voterai pas, et je veux dire pour la une fois et mes collègues, quelle que soit leur département d'Île-de-France le savent. Que le Grand Paris Express n'est pas payé par le gouvernement. Il est payé par l'Île-de-France et par les Franciliens le gouvernement le précédent nous a imposé de créer des taxes supplémentaires payés par les entreprises et les particuliers et l'État s'est totalement désengagé du financement des transports publics en Île-de-France et la réalité, c'est que le Grand Paris Express et payé par les Franciliens par la région par les collectivités par les entreprises et par l'ensemble des citoyens qui payent de taxes supplémentaires, ce qui veut dire mon cher collègue, Bazin quand réalité on peut pas dire que le financement du Grand Paris Express rajoutons pas de la dette sur l'État puisque l'État ne paye rien, c'est nous qui payons, alors moi je suis d'accord, je l'ai dit plusieurs fois, le Grand Paris Express a été sous-évalué et a été projetée sur un calendrier irréaliste, je l'ai dit 10 fois depuis 10 ans, très bien, c'est parfait, tout le monde continue, comme si la vérité c'est que pour obtenir ou les marchés pour une gare, tout le monde, entreprises, collectivités et élus, citoyens, tout le monde a participé à l'accroissement de ce qui était le tracé les dessertes du Grand Paris Express : aujourd'hui, il y a des responsabilités et moi je suis pour qu'on fasse le tour, mais je suis surtout pour qu'on remette à plat et que personne ne monte et qu'on se mette tous autour d'une table, que le gouvernement, la région, tout le monde mette le tout sur une table pour dire qu'est-ce qu'on peut faire dans quel délai avec quel financement, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie générale général et je ne sais pas comment tout ça va finir, mais sur le le Charles-de-Gaulle Express ça fait 25 ans qu'on en parle, je ne sais pas, j'étais pas très favorable au fait de le faire, tout simplement, mais à partir du moment où le Sénat comme l'Assemblée comme le gouvernement sont favorables à le faire, il faut en sortir sur le financement, le seul élément Madame la ministre, qui me gêne beaucoup, je le dis, je conclus par la Sécu plante cette décision cette délibération a été prise, y compris par le Sénat, on nous a clairement affirmé qu'il n'y aurait pas un centime de fonds publics et là il y a un vrai sujet, c'est que si on vous dit il y a pas du tout de nécessité de fonds publics pour nous dire qu'il y a 1 milliard 700 millions de prêts de l'État, il y a un petit sujet. Merci monsieur Karoutchi monsieur Lafont pour explication de vote. Je voterai la maman ne collègue bazar, je pense que l'intérêt de de cet amendement, c'est d'attirer l'attention, il s'agit pas, il l'a bien dit d'opposer un projet contre un autre, l'utilité du Charles-de-Gaulle Express s'est aussi avéré et bien sûr le Grand Paris Express, son utilité est également complètement avéré mais on est dans une situation qui est un peu complexe, un peu complexe, tout simplement parce que nous n'avons pas de réponse de l'État pour l'instant est une réponse, comme il l'a dit, qui est différée dans le temps et qui commence à pénaliser ce projet et à travers cet amendement, c'est en cela qu'il a vocation à attirer l'attention, c'est aussi de souligner qu'il serait temps que l'État répond sur la question du Grand Paris Express qui est, pour l'ensemble des élus franciliens, une priorité une priorité parce que c'est sur ce projet que nous nous sommes engagés dans nos collectivités et pour lequel il y a une mobilisation de de d'argent public, à travers notamment la taxe spéciale d'équipement, donc il ne s'agit pas d'opposer un projet contre un autre mais par condottiere l'attention sur la nécessité désormais de la part de l'État, de répondre aux incertitudes sur le Grand Paris Express née des cirques ou budgétaires qui ont été évalués identifier et quantifier pendant l'été et donc dans cette esprit moi je voterai cette amende. Merci monsieur Lafond la parole est à monsieur Baeza pour explication de vote. Merci madame la présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, juste pour 2 petits complément ce que peut plus évidemment les énoncés en 2 minutes 30, il faut savoir que ce projet de métro automatique du Grand Paris, ce n'est pas un projet uniquement un projet des habitants pour améliorer et pourtant c'est bien nécessaire, leurs conditions de transports en commun du quotidien, c'est aussi une vision du développement de la région-capitale tout à fait indispensable pour nous maintenir dans la compétition des grandes villes monde sachant que sur notre continent européen en Europe occidentale, il y a 2 villes Mondon compétition n'a pas 3 il y il y a Londres et Paris, et si on croit que le simple Brexit nous permet de nous qualifier plus facilement dans cette compétition, se tromperaient lourdement, nous avons absolument besoin de développer notre région capitale pour le bénéfice d'ailleurs de l'ensemble du territoire français, bien évidemment, donc c'est cette vision cet accord général sur le développement de la capitale, appuyer sur un réseau de transport qui est global et qui ne peut pas être détaillées, c'est pourquoi l'ensemble de du réseau doit être réalisé, ça c'est un point extrêmement important, deuxièmement et en réponse à Roger Karoutchi, bien sûr, que il n'y a pas de fonds d'État puisqu'il y a des taxes spéciales affectées et que ce sont les habitants, les entreprises de l'Île-de-France, qui payent ce réseau mais ce modèle il est robuste, il produit 550 millions d'euros de ressources annuelles, il permet donc à la SGP d'emprunter les fonds nécessaires, même si, et je partage son avis, un certain nombre de dépenses peuvent être revus à la baisse pour faciliter la réalisation globale du projet mais le modèle financier et robuste, ce qui nous ont opposés par l'État, c'est des critères d'endettement maastrichtien Colombo donc le Land Act, la dette de l'AGP étant aggloméré à celle de l'État aux yeux de l'Europe, c'est ce qu'on nous dit : je ne sais même pas si c'est totalement techniquement exact, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit mais. On ne peut pas soutenir cet argument, d'abord, je pense qu'il faut pas le retenir, mais on ne peut pas le soutenir dans un 1er temps et dans le même temps endetter le pays d'un milliard 700 millions pour faciliter un autre projet qui a toujours été vue comme nos concurrents qui a toujours été affirmée comme un projet différent, nos concurrents, donc de de la ligne 17 nord, qui va jusqu'à Roissy, sinon on a une absurdité que nous n'arrivons pas à comprendre, dernier point, encore une fois sur le marché bancaire permet de financer comme on le Charles-de-Gaulle Express sans difficulté, donc on ne comprend toujours pas pourquoi cette proposition est faite, je vous remercie. Merci Monsieur Bazin la parole à monsieur Ouzoulias. Oui, moi je voterai une nouvelle fois l'amendement de monsieur Baeza mais je, je voudrais dire que je partage certaines des objections formulées par monsieur Karoutchi je trouve que leur leur de leur de positions ne sont pas complètement antagonistes elle se elle se complètent et je partage aussi le sentiment de monsieur Karoutchi sur l'hypocrisie du gouvernement le gouvernement nous explique que les Jeux olympiques, c'est essentiel pour notre pays la France, il engage toute la nation, d'ailleurs, ce projet, pas seulement les Parisiens, pas seulement les habitants de la, de l'Île-de-France, même chose à propos du Brexit qui veut faire de la place de Paris, une place de rayonnement mondial là aussi s'engage toute la nation donc laisser croire qu'on pourra à la fois accueillir olympique développer la place de Paris sans renforcer de façon considérable, tous les transports du quotidien, c'est une illusion, c'est une illusion, il faut aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités et engage de lourds investissements, par l'emprunt pour remettent à niveau la totalité des transports du quotidien juste et je finirais là, dessus un milliard 7 c'est exactement ce qu'il faut pour remettre à niveau la ligne B du RER, c'est-à-dire créer un un tunnel dédié entre Châtelet et Gare du Nord voilà. Monsieur Roger a demandé la parole. élu de la Seine-Saint-Denis, j'avais demandé dans les dès les premiers projets du Charles-de-Gaulle Express quand même de faire que en Seine-Saint-Denis le le tracé va passer dans ce département, il y a au moins 2 arrêts, il n'y seront pas et donc les gens iront directement, on va avoir les ennuis, ça va creuser partout, ça va passer en Seine-Saint-Denis, mais les gens de la Seine-Saint-Denis ne pourront jamais le prendre pour aller à Charles-de-Gaulle et jamais, même le prendre pour éventuellement aller travailler sur la plateforme, ce qui est encore plus aberrant mais sur le reste, je suis d'accord, on a une taxe on paye et c'est l'Île-de-France qui paye et la Seine-Saint-Denis en particulier sans avoir l'Avantage d'avoir même une seule station dans notre département, parce que tout sera dans Paris intra-muros. Merci, cher collègue, s'il n'y a plus d'explications de vote. Sur cet amendement 415 présenté par Monsieur Bazin qui fait le jet d'une sagesse de la Commission. Sion et du gouvernement, je vais donc le mettre aux voix qui était pour l'amendement.

parce que cet amendement a pour objectif de d'augmenter. Les fonds destinés à l'Iran à la au sein de la BPI il y a un effort considérable qui est fait puisque le fond est abondée de 200 millions d'euros, je vous propose de la bombe de façon complémentaire parce que, aujourd'hui, il y a un volant d'affaires extrêmement importants, j'ai organisé dans mon département, à destination de l'Iran, le 1er la première exportations de bovins vivants. Et je les fais toutes seules, avec un des contacts en Iran sans les ambassades sans le commerce extérieur semble ministre. Faire de l'agriculture, où on sait jamais si par hasard vous n'avez pas les lobbies s'des uns et des autres qui sont là pour faire en sorte que les choses ne fonctionnent pas aujourd'hui le plus gros problème pour nos entreprises qui veulent commercer avec l'Iran, c'est évidemment le secteur bancaire puisque il n'y a que 2 banques en France aujourd'hui, qui travaille avec l'Iran, les autres sont évidemment tétanisés à l'idée des sanctions américaines qui pourraient peser sur une activité dans ce dans ce pays d'où, mais manifestement les sanctions sont levées en termes techniques mais ne le sont pas encore complètement en terme ni diplomatique ni économique, donc la France a de toute façon, d'un point de vue politique et stratégique, complètement intérêt à développer les relations commerciales avec l'Iran, de façon à équilibrer les 2 rives du Golfe Persique, il faut aider nos entreprises dans ses démarches et c'est la raison pour laquelle je propose d'abonder de façon plus importante, les 100 millions que vous avez très légitimement et très intelligemment destinées à l'Iran au sein de la BPI. Merci, cher collègue, avis de la Commission, monsieur Lalonde. Madame la présidente, madame la ministre, ma chère collègue, nous avons bien entendu votre demande de majoration de 20 millions supplémentaires après les 100 millions qui ont été proposées par le gouvernement pour abonder une enveloppe spéciale de la BPI pour favoriser le développement des relations commerciales avec avec l'Iran, c'est une excellente chose, c'est un pays de 80 millions d'habitants, et donc il est important effectivement que dans le cadre de la diplomatie, entre guillemets, financière, on puisse permettre aux entreprises françaises de pénétrer sur ce marché néanmoins une première enveloppe de 100 millions ne permet un effet de levier intéressant et je pense qu'il est utile, en tout cas c'est la position de la commission des finances de considérer que ce sont 1000000 sont aujourd'hui suffisant regardez quel sera l'effet de levier avec les entreprises avant de la abonder de 20 millions supplémentaires, donc je vous propose de le retirer ou ça sera un avis défavorable de la commission merci. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la ministre pour la vie du gouvernement. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, en effet, le le programme 869 à bien le l'objet. Dédé la BPI a amorcé une activité de crédit export vers l'Iran afin de pallier l'absence de financeur privé pour nos entreprises exportatrices vers ce pays, nous pensons que ce système va se mettre en place avec des financeurs privés mais qu'il faut amorcer la pompe grâce à la BPI donc ce 1er près de 100 millions permettra la BPI de montrer que cette activité est réalisable dans de bonnes conditions et dans le respect des sanctions internationales à cet égard, les 100 millions d'euros nous semble suffisant pour faire cet amorçage encourager les investisseurs internationaux à prendre le relais, le nombre, le volume de prêts que BP sera en capacité de réaliser dans les dans les années qui viennent, est assez incertain ce stade et il est peu probable qu'en 2018 il y a besoin de plus de 100 millions, c'est c'est pourquoi nous proposons également le retrait merci. Merci madame la ministre Madame Goulet. Et je vais, je vais me retirer mais je voulais je voulais attirer l'attention du gouvernement sur le fait : un, il faut absolument que la BPI communique le président de la région Normandie a fait un déplacement là-bas avec des entreprises toutes le MEDEF il y va régulièrement les ailes et les organisations agricoles aussi, il faut d'abord que la BPI puisse aussi être utilisé par les entreprises agricoles et les exportateurs de produits agricoles qui n'ont jamais été sous embargo, donc un mini puisqu'on est dans la cohérence et qu'on commence, puisque c'est la première fois que ce fonds est abondé à destination de ce pays et qu'il est ciblé, mettant aussi tout de suite de la méthode mettant aussi tout de suite de la méthode, c'est-à-dire un ciblons les, les, les entreprises qui pourront en bénéficier, ajoutons y les entreprises agricoles et l'agroalimentaire, pour lequel il n'y a jamais eu d'embargo et ensuite que la BPI fasse une communication qui soit pluri- sectorielles de façon à ce que les entreprises qui sont un peu frileuses à l'égard de l'Iran et qui ont peur des sanctions, bien qu'elle soit levées puisse puisse en bénéficier donc, encore une fois, ce sera probablement un test de de la capacité et la volonté de la BPI de de mettre un peu d'ordre et de et de méthode dans un dans que vous prenez, Madame la Ministre à Benicio donc c'est vraiment le moment de montrer ce que comment on peut travailler de façon organisée et moi je, je suivrai aussi ce dossier avec beaucoup d'intérêt, puisque j'ai beaucoup d'entreprises de Normandie qui sont évidemment très impliquée notamment les les entreprises agroalimentaires, donc je retire l'amendement merci. Merci Madame Goulet, l'amendement 394 et donc retirés, nous allons procéder Rove vote des crédits du compte spécial prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés figurant à l'état des jeunes été saisi d'aucune demande explication de vote avant l'explique l'expiration du délai limite je mets donc vous allez crédit du compte spécial qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Les crédits sont en adopter, je vous propose 5 minutes de suspensions de séance, le temps de changer d'équipe. Ministériel merci madame la ministre, nous allons donc accueillir un Madame Girardin ministre des Outre-dans 5 minutes, reprise de la séance.

La séance est reprise, madame la ministre, mes chers collègues. Par lettre en date de ce jour, monsieur François Patriat, président du groupe, la République en marche, a demandé le retrait de l'ordre du jour réservée à son groupe du mercredi 13 décembre 2000 17 du débat sur le thème la politique en faveur des étudiants et et son remplacement par un débat sur le thème : le retour des djihadistes en France acte donner de cette demande, j'informe le cénacle des candidatures pour siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaire ont été publiés ces candidatures seront ratifiés si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions : le Sénat va examiner les crédits de la mission outre-mer. Article 57 quater inquiète sexuelle et Et la parole est à monsieur Georges Patient, rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Salut. L'effort budgétaire et financier global de l'État en faveur des outre-mer s'élève en 2018 à 21,3 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 20,5 milliards en crédits de paiement cet effort correspond à 3,9 pourcent du budget général, alors que les populations ultramarines représente 4,3 de la population, ce qui m'autorise à dire que les outre-mer ne sont pas aussi budgétivore que certains peuvent le penser. Les crédits de la mission outre-mer 13 pourcent des crédits de l'État consacré aux Outremers, à travers ces 2 programmes emploi outre-mer et conditions de vie outre-mer sont à bien des égards, indispensables pour ces territoires qui souffrent d'importants handicaps structurels liés à leur éloignement de l'Hexagone à la faiblesse de leurs marchés locaux. Il a leur tissu économique composé pour l'essentiel, de très petites entreprises. L'année 2017, à mon sens particulièrement révélatrice de ses fragilités. Je pense au mouvement social survenu en Guyane qui n'est qu'un symptôme des difficultés de ce territoires mais il y allemand à l'ouragan Irma qui nous rappelle la prégnance des risques naturels auxquels sont confrontés ces collectivités. Il faut souligner d'anglais que les crédits sont maintenus au-dessus du seuil des 2 milliards d'euros, puisqu'ils s'élèveront à 2104 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2000 68 milliards d'euros en crédit de paiement à périmètre constant, il est en hausse de 3,6 pourcent en AE et de 4,3 pourcent en CP par rapport à 2017 on ne peut que s'en réjouir, en tout état de cause, il convient d'insister sur le fait que ce budget le 1er du quinquennat constitue un budget de transition. Ne présage qu'en partie des priorités futures. Pour les prochaines pour jouer, projet de loi de finances, le gouvernement s'est en effet engagé à s'appuyer sur les bleu Outre-Mer qui résultera des incidents outre-mer lancé par le gouvernement le 4 octobre 2017 afin d'ouvrir un temps d'échanges et de réflexion avec l'ensemble des ultramarins. La compensation des exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale spécifique outre-mer est le principal exemple du caractère transitoire de ce budget, selon le gouvernement, ce dispositif devrait faire l'objet d'un réexamen à l'Automne 2019 nous serons particulièrement vigilants quant à ce que cette réforme soit favorable à l'emploi outre-mer le chômage culminant encore aujourd'hui à 20 pourcent en moyenne dans ces territoires. Ce budget présente quelques motifs de satisfaction, les crédits destinés au financement des opérations contractualiser entre l'État et les collectivités d'outre-mer sont en hausse de 12 pourcent en autorisations d'engagement et de 6 pourcent en crédits de paiement, cette hausse est particulièrement bienvenue alors que de nombreux contrats en fait l'objet d'un important sous-financement des années passées. Les crédits du fonds exceptionnel dès investissements sont en augmentation de 3 pourcent on eux surtout le gouvernement s'est engagé à un maintien de sa dotation au niveau de 2018 sur l'ensemble du quinquennat. Nous avons souligné dans le rapport d'information que nous lui avons dédié l'an dernier l'utilité de cet instrument, nous serons donc là aussi particulièrement vigilant quant au respect de la promesse du gouvernement. Ce budget conforte le service militaire adapté qui atteint en 2017 objectif il fixer former 6000 jeunes ultramarins et leur permettre une insertion dans le monde professionnel, ces crédits sont en augmentation de plus de 4 pourcent et le ratio d'encadrement a été améliorée, enfin si les crédits affectés au logement sont en légère baisse les crédits de paiement des dire la construction neuve seront en augmentation, c'est donc bien conscient de l'ampleur des besoins des outre-mer mais également du fait qu'il s'agisse d'un budget de transition que nous vous proposons avec mon collègue nuit et il ne peut être présent aujourd'hui d'adopter les crédits de la mission outre-mer. Je joue ainsi le jeu, madame la ministre, comme l'a suggéré à l'époque un grand guyanais Félix Eboué. Je joue le jeu parce que le président de la République lors de son passage en Guyane, en octobre dernier, vous y étiez aussi. évoquant pour le citer les engagements budgétaires dont plus personne ne comprend même la logique et les milliards accumulés sans qu'on n'est jamais le mulet affirmait qu'il voulait en finir avec une relation asymétrique, faite de promesses non tenues. Pour ce faire, il déclarait qu'il était prêt à rouvrir des sujets constitutionnel s'il apparaît pertinent de le faire et que c'est utile. Allez, porté par un véhicule législatif unique qui fasse la synthèse de tous ces besoins de toutes les adaptations, et ce par des décisions fortes de l'été prochain. Je veux croire en ces mots présidentiels concernant tout particulièrement la Guyane mon territoire. La crise de mars dernier en effet, révélé les limites institutionnelles de notre système de gouvernance et remis l'accent sur la question de l'évolution statutaire. Celle-ci figure d'ailleurs dans les accords de Guyane, signé par le précédent gouvernement et fait l'objet d'ateliers sur la gouvernance dans les états généraux de Guyane et les Assises des Outre-mer. J'espère, Madame la Ministre, que ces mots présidentiels. Qui exprime une volonté affichée de coller aux réalités des mer ce seront suivies d'effets pour tous les ultramarins puisque ce discours présidentiel de lancement des assises était diffusé en Direct à l'instant de tous les autres, mais je vous remercie de votre attention.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelques mots donc sur ce budget que je qualifierais pour ma part de budget d'amorçage ou l'attente et quelques propositions opérationnelles dans le but d'activer les crédits dans l'Outre-mer après leur vote solennel, tout d'abord l'affichage d'une ode d'une hausse de 4 pourcent des crédits ne nous a pas totalement convaincu, ce ratio traduit non pas une augmentation pour 2018, mais plutôt un dégonflement rétroactive des crédits pour 2017 un peu boostée pour parler français, juste avant les dernières élections présidentielles pour rompre avec ces pratiques, nous approuvons, Madame la Ministre, sincérité budgétaire que vous évoquez. Nous disons que cette sincérité doit également conduire à reconnaître qu'avec les crédits stabilisés à 2 milliards depuis 7 ans les ultramarins participent à l'effort de rigueur en totalisant toutes les missions et tous les ministères, on arrive à 17,3 milliards ce chiffre augmente mais son niveau dément le préjugé sur les budgétivores que nous sommes. Le collègue Georges Patient vient de le rappeler. Ce budget proposé pour 2018 a un peu déçu car il n'est pas à la hauteur des défis, le taux de chômage ultramarins est un révélateur, on atteint le doute de la moyenne nationale, tous les équilibres économiques, sociaux et politiques, le le gouvernement est conscient et a assorti ce budget de plusieurs engagements complémentaires reconstruction financement des projets sélectionnés par les assises mer et grand plan d'investissement, la commission a donc choisi, Madame la ministre de faire confiance à cet élan positif notre principale inquiétude porte toutefois sur le logement, qui est une base fondamentale de la citoyenneté réelle un objectif raisonnable a été fixé dans la loi et Rome 150000 logements construits ou réhabilités en disant pour l'atteindre, concrètement, il faut une stratégie globale et articulé subventions, aides fiscales procédure d'agrément efficace mais aussi du foncier des normes de construction adaptée et une programmation astucieuse pour choisir les bonnes cibles, une fois n'est pas coutume, j'insiste sur l'efficacité démontrée du moteur fiscales pour favoriser le logement social et la réhabilitation je présenterai par la suite des amendements en ce sens, mais pas sur la mission outre-mer pour optimiser le financement public, il faut absolument clarifier et pacifier les procédures d'agrément, sans quoi la construction stagne et tous les autres secteurs économiques le formalisme excessif génère du découragement, surtout pour des jeunes talents ultramarins qui vont créer des richesses dans d'autres pays, j'en termine avec quelques mots sur la compétitivité ultramarine elle nécessiterait tout d'abord le maintien du CICE car l'impératif de stabilité prime les autres considérations, à défaut, il faudra résoudre le rébus des compensations notre proposition et de les cibler, de préférence sur des projets précis et à long terme, plus généralement, optimiser la dépense publique, c'est aider les territoires à financer les activités une un environnement normatif adapté, Madame la Ministre, vous pourrez compter sur le Sénat pour identifier et combattre les incohérences qui entravent encore beaucoup plus qu'on ne l'imagine, le développement de nos outre-mer je vous remercie. Merci monsieur Magra Madame Nassimah Dindar. Rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. sociales. La présidente, Madame la Ministre, mes chats collègues le budget qui nous est aujourd'hui proposé ne porte pas de mesures particulièrement marquantes dans le sens de la compétence de la commission des affaires sociales et ne peut constituer pour elles qu'un budget de transition, elle a donc émis un avis favorable à la stabilité des crédits de la mission outre-mer tout en alertant des effets de périmètre, qualifié de combinaisons de tuyauterie en clair, nous ne souhaitons pas que par décret des sommes affichées, puis être en cours d'année retirés du budget au passé sur un autre programme plus Style, celui de l'enseignement scolaire, comme cela était le cas l'an dernier le gouvernement baisse de 54 millions d'euros les dotations aux collectivités territoriales et demande à ces collectivités de faire des efforts, elles le font, mais ces collectivités a donc attendons donc plus de l'État sur le logement, les collègues mondial avant moi nous regrettons cette interruption de l'effort public alors même que les populations des outre-mer subissent des conditions de logement particulièrement dégradée ma collègue Viviane développera les effets à craindre de la baisse de la LPO et de l'APL je profite de ce moment solennel pour réitérer mes demandes à propos de la politique foncière dans les Dom, au ministre de la cohésion des territoires et demandé l'extension, hommes de la zone tendue afin de bénéficier de l'abattement de 100 pourcent la plus Value de la vente d'un terrain à bâtir pour des logements sociaux sur la problématique Foncia, toujours le statut départementaux domaniale qui persiste à la Réunion et en Guyane freine de vrais projets de développement environnemental et social ainsi à la réunion des familles peuvent ne pas bénéficier des aides publiques à l'amélioration de l'habitat, alors même que leurs conditions de logement sont reconnus comme totalement dégradé, cela n'est pas normal. Madame la Ministre loger n'est pas habiter et habiter n'est pas seulement loger, je m'explique : les gens peuvent avoir une vie très simple en gardant leurs Liens à la nature et à la terre, garder les conditions de leur enracinement et c'est pour cela pousse souvent ils peuvent déplorer les contraintes normatives appliqué dans nos régions contraint qui ne s'ancre pas dans les réalités locales nous collègue vient de l'évoquer, je ne doute pas, Madame la Ministre, un seul instant de votre détermination de votre engagement, vous connaissez mieux que moi les outre-mer et je veux vous le dire ici, oui, les assises peuvent être une opportunité de construire une politique publique cohérente et efficace afin de porter l'avenir de noter territoire. je terminerai sur les préconisations de la commission des affaires sociales qui constate une performance contrastée en matière doivent de soins dans les outre-mer avec quelques défis sanitaires importants à relever sur des maladies chroniques des addictions où la mortalité périnatale avec à Mayotte et en Guyane des enjeux qui dépassent le cadre sanitaire, nous souhaitons donc que la nouvelle stratégie santé outre-mer qui sera défini pour les prochaines années, puisse faire l'objet d'une grande concertation et d'une mobilisation forte de l'État avec les différents acteurs concernés dont les collectivités territoriales, communes et départements bien évidemment et les régions, nous souhaitons également que des expérimentations puisse être menée dans le cas de la santé du sanitaire et du social car nous sommes convaincus que les outre-mer peuvent aussi être considérée comme le laboratoire du monde qui vient, je vous remercie. Merci beaucoup madame la rapporteure, la parole est maintenant à monsieur Tony Mohamed Soilihi. Rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour la 4ème année consécutive, il me revient de vous présenter la vue budgétaire de la commission des lois sur les crédits de la mission outre-mer, prenant acte du maintien de l'effort budgétaire en faveur des territoires d'outre-mer, celle-ci a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits des résultats des incises des outre-mer que vous avez lancée en octobre dernier, Madame la Ministre, viendront certainement faire évoluer ce 1er budget dans cette attente, j'ai souhaité m'intéresser aux problématiques institutionnelles de chaque territoire ultramarin et réaliser ce travail d'état des lieux, car au cours des dernières années, le Parlement a débattu de nombreux projets ou de propositions de loi tendant à clarifier le statut institutionnel de telle ou telle collectivité ultramarine, le gouvernement annonce par ailleurs d'autres textes en la matière, au vu de l'actualité je concentre mon propos sur 2 collectivités ultramarines, la première, et bien évidemment la Nouvelle-Calédonie et les questions soulevées par l'organisation du référendum d'autodétermination, prévu en novembre 2018 et notamment la composition du corps électoral qui participera le XVIe comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui s'est réuni le 2 novembre dernier à trouver un consensus, un Mac tant de manière exceptionnelle, l'inscription d'office des personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sur la liste électorale générale préalables indispensables à leur inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation relative à l'autodétermination c'est accord implique de modifier la loi organique de 1999 un avant-projet de loi Boughanmi destiné à modifier la procédure de révision des listes électorales et traduisant cet accord politique, a reçu le 23 novembre dernier un avis favorable du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de certaines précisions, cet avant-projet de loi organique et en principe était délibérée en conseil des ministres, nous serons saisis prochainement de cette question très sensible, d'autant que la conclusion de cet accord n'a pas mis fin aux tensions politiques qui secouent la Nouvelle-Calédonie entre indépendantistes et un pendentifs et au sein de chaque mouvement j'en viens maintenant à mon second point Mayotte bien que dénommée département ce territoire mais sur le plan juridique, ni un département ni une région d'outre-mer, bien qu'ils relèvent des collectivités de l'article 73 de la Constitution, il constitue depuis 2000, une forme de collectivité unique dans l'assemblée délibérante le conseil départemental exerce les compétences d'un département et certaines compétences d'une région, les autres étant plus ou moins assumées par l'État, cette situation a des impacts en matière budgétaire non négligeable puisque Mayotte qui ne bénéficient quasiment pas de la dotation globale de fonctionnement régionales, ce que la Commission avait déjà dénoncé en 2015, pourquoi ne pas envisager une prise en compte, a minima de la double compétence de Mayotte, sur le modèle de ce qui s'applique aujourd'hui en Guyane et en Martinique, à l'approche des fêtes de fin d'année, je forme le voeu de voir régler cette question à l'occasion d'un prochain toilettage institutionnel du statut de Mayotte, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention en général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir, la parole est maintenant à Madame Éliane Assassi pour le groupe CRC pour 6 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si les chiffres des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de cette mission outre-mer sont sans nul doute capitaux, il est d'autres chiffres qu'il me paraît fondamental de rappeler en préambule ne sont pas que des petits bouts de France baignée par des mers chaudes, ce sont plus de 2,7 millions d'habitants, donc d'habitants, soit un peu plus de 4 pourcent de la population française, dont beaucoup vivent dans une situation d'inégalité intolérable par rapport à la métropole, comme le rappelait l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'égalité outre-mer la et dernière par le Parlement, je cite, en dépit des politiques publiques volontarisme par l'État et les collectivités territoriales des outre-mer, les écarts de niveau de vie constatée entre les Outre-Mer et la France hexagonale reste considérable et affecte l'égalité des droits économiques et sociaux et des opportunités économiques

l'ensemble des territoires ultramarins affiche une surmortalité marqué autour de la grossesse ainsi alors que le taux de mortalité infantile s'établit à 3 avec 5 pour 100 en France métropolitaine, il atteint 6 pourcent Martinique

autre exemple, s'agissant du travail, selon l'enquête emploi pour l'année 2016 les taux chômage constatée dans les départements d'outre-mer, a-t-elle en effet plus du double de celui relevé dans l'Hexagone,

à Mayotte, je rappelle que dans l'Hexagone, c'est 10,1 pourcent là encore, nous ne pouvons nous résigner à de telles différences l'année qui vient de s'écouler a d'ailleurs permis de rappeler à ceux qui ne se souviendrait des territoires ultramarins qu'en période de campagne électorale que nos concitoyens ne sont pas résignés aux inégalités, à la pauvreté, chacun se souvient la espère du mouvement social sans précédent qui a mobilisé les guyanaise et des Guyanais au printemps dernier et qui a trouvé un terme provisoire avec la signature d'un plan d'urgence, chiffré à 1,86 milliards d'euros, dont 250 millions pour construire 5 lycées et des collèges en 5 ans dans un tout autre domaine, les ouragans Irma et Maria qui ont provoqué le déplacement de près de 7000 personnes devraient nous faire prendre conscience de l'urgence qu'il y a agir tant pour réduire les risques que pour anticiper les migrations liées au dérèglement climatique, permettez-moi également Michard collègues de vous conseiller la lecture des avis récemment publiés par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans le cadre d'une étude sur l'effectivité des droits de l'homme dans les outre-mer dans la vie, relatif à la pauvreté et l'exclusion sociale du 2 septembre 2017 la Commission rappelle à juste titre, que les droits de l'homme sont indivisibles et que l'extrême pauvreté pauvreté constitue en elle-même une violation des droits fondamentaux, droit à un logement salubre et sûr, droit à une éducation de qualité, droit à une bonne alimentation à vivre dans un environnement sain ou encore accès à la justice et à la à la santé, ces droits ne sont bien entendu pas tous effectif en métropole et il reste beaucoup à faire, mais dans les territoires ultramarins, la situation est tout à fait alarmantes des mesures spécifiques doivent être prises immédiatement au regard de ce que je viens d'évoquer la question qui reste est celle de savoir si les crédits qui nous sont soumis, aujourd'hui, sont à la hauteur de des enjeux, la réponse est évidemment et malheureusement négative et le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera contre notre collègue Nassimah Dindar, rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, pas à juste titre de budget de transition, le gouvernement s'étant engagé à s'appuyer pour la détermination des priorités des prochains, projet de loi de finances comme pour un éventuel nouveau site de réformes sur les constats et les propositions qui ressortiront donc du Livre bleu qui sera produit à l'issue des assises de l'outre-mer ouverte le 4 octobre dernier, la situation est telle, s'agissant des outre-mer que le statu quo budgétaire dans l'attente de nouvelles orientations et de nouvelles réformes n'est pas acceptable, je vous remercie. Merci Madame Assassi, la parole est maintenant à Madame Catherine Conconne pour le groupe socialiste et républicain. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Sachez, Madame la Ministre, chère Annick Girardin, que j'ai beaucoup pensé à vous, en étudiant les crédits de votre mission. Comme vous avez dû être déçu, madame la Ministre de tout le mal vous à fin en vous autorisant untel, budget. Comme vous avez dû être déçu, vous la femme à la détermination palpable au courage affiché que j'apprécie ce courage et cette détermination de la femme des îles habitué comme tous les habitants de la dite outre-mer à la résistance et à l'audace salvatrice comme non Madame la Ministre, vous avez dû être déçu de voir autant de chapitres regroupés sous l'appellation, conditions de vie outre-mer, ramené à la baisse dans des proportions extraordinaires sacré signal donné message on ne peut plus clair, conditions de vie Outre-Mer oui, Madame la Ministre, vous baissez les lignes les plus significatives, dédié aux conditions de vie outre-mer. J'avais beau pour vla logement moi 20 millions d'euros en autorisation d'engagement et moins 3 millions d'euros accrédite paiement, ce qui représente un volume de logements mis en chantier pour réhabilitation d'à peine 200 en lieu et place des quelque 9. De 2017 quand on connaît la nature des difficultés dans ce domaine, difficultés liées à l'histoire si jeune et si tourmenté de nos territoires, comment rentrer de cette séance auprès de nos compatriotes pour avec une telle annonce, madame, monsieur, pas cette année, pour votre logement, dans le 3 fuit pas cette année, pour votre logement dans l'électricité est affreusement hors norme comment expliquer aux nombreuses entreprises de 2, 3, 4 ou 5 salariés totalement dépendant des signaux dans ce domaine que cette année, les carnets de commandes resteront définitivement voire inerte, je vous laisse imaginer les dégâts collatéraux et les charrettes de chômeurs en prévision dans des économies qui affiche déjà des chiffres qui dépassent partout les 20 comment comprendre aussi que les les crédits en baisse sur les lignes Sport, jeunesse sanitaire sociales tue le sport dans lequel mon collègue membres de mon groupe, Patrick Kanner s'était personnellement investi en mouillant le maillot dans l'optique, victoire pour annoncer des investissements. Important lié à la réhabilitation des infrastructures sportives dans des pays fournisseurs de champion, pour la France, l'emblématique Teddy Riner Jean-Marc Mormeck Dimitri Payet, Laura Flessel, aujourd'hui ministre de la République, Raphaël Varane Karembeu et j'arrête là la liste où est passé le financement de ces infrastructures, les crédits baissent aussi dans un, dans le cas des dispositifs incontournable, il y a la formation professionnelle, moins 8 millions d'euros en autorisation d'engagement et cela est moins 7 millions de Rouen, crédits de paiement, je veux parler de l'atome, vous connaissez la difficulté contenu de l'étroitesse de nos manches et impôts, voire à pouvoir mieux assurer la promotion par la formation, le président de la République annonce la formation professionnelle sera le bras armé du gouvernement pour lutter contre cette pandémie du chômage, c'est grâce à cet organisme que nos populations peuvent donc y accéder le équation Finale simple Madame la Ministre, il y aurait donc les paroles et et là c'est les actes car comment accomplir cette volonté sans y mettre les moyens. Le gouvernement a annoncé vouloir faire du tourisme du développement touristique dans nos pays une priorité très bonne intention cependant le 1er ministre a même symboliquement ouvert en personne les assises de l'Outre-mer par la télé, tourisme, le mois dernier à votre présence en notre présence, déclaré à cette occasion que les efforts doivent être munis pour améliorer le produit pour le rendre plus performant, mais comment le faire quand, ne serait-ce que sur la formation professionnelle de niveau supérieur qui nécessiterait des déplacements, les crédits sont en baisse avec l'affichage, qui aurait dû être mis dans ce bureau dans ce budget, on pourra lutter contre et disparités cruel entre haute et basse saison attirer des investisseurs, ce qui avait quitté certaines de nos territoires avec fracas, mais aussi avec perte augmenter le niveau moyen de dépense du touriste rien. J'ai moi-même convaincu que ce secteur économique peut et doit être un formidable levier et j'ce déposer un amendement pour exonérer de charges patronales, les employeurs du secteur touristique qui acceptent d'embaucher des artistes pour animer valablement leur structures qui aujourd'hui sont aussi froide que matin de décembre parisien Édouard Philippe Lafon notamment souhaité, je le rappelle, améliorer le produit, nous a-t-il dit avec fougue, alors j'espère que sur cette seule petite niche vous accepteriez de soutenir mon initiative pour les nombreux artistes de notaire féconde dans le domaine culturel et donc trop de leurs acteurs sont aujourd'hui condamnés faute de contrat à émarger au RSA oui au RSA dans le domaine culturel, sur les Terres de Césaire du bon coup Chamoiseau de Damas ou de Maryse Condé permettez-leur de travailler, de se remettre à produire, je participe à des festivals désormais morts qui pourraient être créés : savez-vous que sur un cachet de 100 euros la dépense réelle pour l'employeur et finalement de 187 euros comment vivre de son art. Quand ce formidable aucun poète le tourisme ne peut, à ce tarif, je cite de nouveau améliorer le produit, rien n'est prévu d'éloquents dans le domaine du tourisme les efforts sollicités dans l'autre assemblée du Parlement été 20 alors Madame la Ministre je compte sur votre solidarité pour faire au moins ce geste ce double geste a doublé, destination cette mesure très attendue Winner pas dans ces propos sur la République, mais permettrait de lutter contre la précarité, à la fois des acteurs mais aussi de la qualité de l'Amérique du jeu, conclut enfin je sais, Madame la Ministre, que vous me direz : les assises de l'Outre-mer, les assises de l'outre-mer, mais j'ai encore des doutes, à croire qu'il ne s'agit pas là de petits cachets de Doliprane, un autre un énième face aux douleurs qui nous ronge et qu'il faut l'avouer, Madame la Ministre, sont loin d'avoir été symboliquement prises en compte dans cette édition 2018 du budget

La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Vignon. Pour le groupe, les indépendants, pour une durée de 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la ministre, chers collègues, je voudrais vous dire pour commencer, que j'aime les outre-mer et je suis honoré de représenter le groupe auquel j'appartiens, pour présenter les observations de ce groupe sur le budget, certains me connaissent et savent l'intérêt que je porte à à vos territoires, j'y suis allée souvent et toujours avec un plaisir immense toujours avec des inquiétudes fortes mais je voulais vous saluer mais chers collègues ultramarins car vous relayez avec toujours beaucoup de dignité, les populations, vous représentez pour nous dire avec une constance responsable et légitime la situation qui vous inquiète, ce qui nous inquiète les défis de nos territoires ultramarins sont immenses, n'y a que penser un instant au paysage apocalyptique qu'on a vu récemment à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy avec les problèmes de mouvements populaires en Guyane qui ne peuvent pas ne pas nous inquiéter et partout, une forme de fatigue de consternation de sentiment d'abandon auxquelles il faut réagir nos territoires ultramarins sont, en effet, plongés dans une situation économique et sociale qui est sérieuse, cela a été dit par les mais les orateurs précédents un taux chômage élevé extrêmement élevé dans certains endroits, les jeunes qui sont pourtant les incarnations du futur de ces territoires et que vous défendez toujours avec beaucoup de de vigueur sur les plus durement touchés par le chômage sont désoeuvrés, le PIB par habitant il y atteint parfois des niveaux qui sont scandaleusement bas en Guadeloupe, Mayotte, alors qu'il se situe 3, 4 fois plus élevé en métropole, l'État a pourtant fait des efforts importants, ça n'est pas discutable pour aider ces territoires, les crédits de la présente mission outre ceci 88 programme de 29 autres missions contribuent au financement de l'accompagnement des territoires ultramarins pour un effort pour un effort total de 21 milliards à l'instar de la la rapporteure pour avis, notre groupe Renault retrait regrette cette éclatement des crédits, appelle à une unification la structure budgétaire de ces engagements depuis le mais le gouvernement, engagé une politique de rationalisation des dépenses ultramarines en matière d'exonération de cotisations sociales, celles représentent plus de la moitié des dépenses de la mission, ce qui nous conduit à saluer cette entreprise peuvent être de formidables les acteurs dans la conduite des expérimentations publiques on le, on l'a encore vu ce matin pour la la et les 2 formidables table ronde qui a mené notre collègue Magra au nom de la délégation qu'il préside, sur la biodiversité sur les opportunités et la richesse de cette biodiversité, 100 pourcent d'énergies renouvelables, laboratoire de prise en charge de personnes âgées, réforme de la politique pour tirer de la surveillance des quantité d'expérimentations ont lieu en en outre-mer et il faut les prendre en compte les prochaines assises de l'Outre-mer, Madame la Ministre, devront d'ailleurs définir avec précision une feuille de route pour avancer sur ces projets, ouvrons incarner l'espérance et devront consiste constituer un renouveau plusieurs situations appelle malheureusement une réaction rapide des pouvoirs publics conduisent à interpeller le gouvernement, comme l'a fait notre collègue Madame Assassi avec beaucoup d'détermination et que je partage sur la situation sanitaire la mortalité sainte infantile et est un véritable scandale quand on la compare à la mortalité infantile en en en métropole, un essoufflement du système hospitalier sur la peau, des problèmes migratoires à Mayotte, une situation immobilière avec une assiette a su l'insalubrité critique une situation préoccupante pour près de 150000 personnes le constat et et et souvent terribles, les engagements financiers sont insuffisants pour résoudre ces problèmes, que feront quelque 3,9 millions d'euros destinés au financement dans le domaine sanitaire et social, quand les territoires ultramarins sont au bord du gouffre comment diminuer la justice diminution des crédits de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, alors que le gouvernement promet de donner une nouvelle dynamique au déplacement dans 6 directoire et de lutter contre les inégalités territoriales comment enfin mettre en adéquation le problème du logement et la diminution des crédits de la ligne budgétaire unique en commission des affaires sociales, notre collègue Viviane Malher, rappeler que les crédits consacrés aux logements ultramarins baisseront 10 pourcent 2018 alors même que les populations ultramarines attendent un accompagnement renforcé en matière d'habitat, il faut donc envisager le recours à 2 autres outils, pourquoi pas, la défiscalisation comme mesures d'incitation à la construction de nouveaux logements, une mesure sans cependant nous nous donne espoir s'agissant du service militaire adapté, nous nous félicitons en effet que les objectifs de 2017 était était atteint et que ce budget soit sanctuarisé jusqu'en 2025, c'est un outil fondamental pour assurer le suivi l'accompagnant dès l'accompagnement des jeunes ultramarins en situation d'échec scolaire ou en grande difficulté, la poursuite de ce programme est essentielle pour l'avenir de ces territoires, madame la présidente, monsieur le président de la commission Madame les monsieur et madame les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe des Indépendants républiques et territoires s'abstiendra sur le vote des crédits de cette mission et prêtera une attention toute particulière, je l'ai dit et je le redis, aux assises de l'Outre-mer nous aiment Rion pouvoir je ne sais pas si nous pourrons y être assisté mais nous aime pouvoir y participer pour dire notre détermination, ces assises seront déterminantes pour l'avenir de notre relation et territoires du ultramarins et si certains ont parlé d'un budget de transition, nous espérons que ces assises permettront d'assurer dans de bonnes conditions, une transition intelligente et qui redonne espoir à à ce pays comme Baudelaire, je terminerai en disant cette phrase qu'il adresse à sa mère, ma puissance d'espérance et mon seul capital et actuellement, c'est la situation des soutes remercier leur puissance d'espérance dans la République, qui leur permet de croire un jour à un avenir meilleur, notre abstention et bienveillante, mais elle est aussi vigilants pour mercredi. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur. Stéphane Artano pour le groupe RDSE. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un budget traduit une vision politique, il exprime une certaine philosophie de l'action publique qui, de ce que les Français ont choisi pour présider à leur destinée, mon intention ne sera pas cet après-midi, au nom du groupe RDSE de rentrer dans le détail de la mission outre-mer je pense que beaucoup de mes collègues l'ont fait le feront après moi. Nous disposons de rapports d'ailleurs très complet sur le sujet, mon intention non est vraiment de porter le débat sur la méthode qui reste, de mon point de vue de notre point de vue, une des clés de l'action publique, ce 1er budget de la mission outre-mer défendue par vous, madame la ministre, préservé essentiel mais ne va pas au-delà. un président de collectivités, je sais aussi que rien ne se fait du jour lendemain comme l'a dit mon collègue Michel Magras en commission, c'est l'amorçage budgétaire du quinquennat et je rejoins de nombreux commentaires de collègues la hausse annoncée de 4 pourcent en fait un dégonflement sincère de 2017 jeudi sincère Madame la Ministre, car vous avez consenti un effort de sincérité budgétaire qui devra d'ailleurs être durable, et ça a été d'ailleurs noté dans le cas de discussion en commission sur auprès, par contrat, faire en sorte que cet engagement puisse être durable sur toute la durée de ce mandat, j'en viens au coeur de mon propos et je pars du constat que le budget 2018, est un budget de transition en collègues Jérôme Bignon l'a à nouveau rappelé mais qu'en est-il pour demain. Il y a 7 heures je dois bien dire reste encore assez floues, la question centrale qui se pose aujourd'hui est celle de la vision que l'État assure l'outre- mer, souhaite-t-il, et je le dis également pour les élus qui siègent dans cette instance souhaitant nous transformer les Outre- mer oui car il s'agit d'une oeuvre collective, une action politique résolue en mer passe par une vision claire de notre avenir je notre avec une constance qui me gêne d'ailleurs que si des réalités sans complexe, nous faisons toujours l'objet d'un traitement différencié par rapport à l'Hexagone il y avez-vous vu, par exemple, comme en 2009, des états généraux ont l'Hexagone je ne crois pas, le président de la République nous annonce aujourd'hui la tenue des assises dans le contour précis a été assez long à mettre en 9 à dessiner, mais les choses sont lancées, il faut s'en féliciter, en posant comme postulat que outre-mer travailler à définir son avenir, le président de la République ne porte pas une vision sur l'outre-mer, mais il demande un ultramarin de regarder vers la métropole d'exprimer nos souhaits. Finalement, à défaut de vision, l'État ne demande-t-il pas assez outre-mer doit lui livrer sur un plateau. C'est ce regard totalement inversée qui me gêne profondément aujourd'hui, pourtant la France attentat à prendre de ses outre-mer, cette absence de vision. Voire même de regard sur le sens de l'action de l'État en Outre-Mer, mer d'encore plus flagrant quand on regarde la culture est un exemple pour lustrer mon propos : nous avons tous entendu votre volonté, Madame la Ministre, de faire en sorte que la Cité des outre-mer soit une oeuvre collective, elle ne l'a peut-être pas été suffisamment et la suppression des crédits effectivement on laisse aujourd'hui penser que les engagements de François Hollande seront difficiles à tenir. Poursuivant sur la culture, comment comprendre qu'aujourd'hui par exemple, au sein de l'audiovisuel public français la disparition de la chaîne France soit une hypothèse de travail au sein du groupe France Télévisions alors même que sur le plan culturel des ponts doivent être créés entre l'outre-mer et l'Hexagone, force est de constater que la Cité des outre-mer dans l'avenir est incertain et la disparition possible de France, qui est une hypothèse de travail est une hypothèse évoquée quand même transforme ce regard de l'Hexagone vers l'outre-mer, j'ai parce qu'on va dire, est en train de briser ce regard, par ailleurs, je crois sincèrement que la politique marine doit reposer sur un socle commun également décidé par le gouvernement, tout en reconnaissant qu'évidemment, la nécessaire le nécessaire respect des réalités des territoires dans certaines problématiques sont extrêmement diversifiées. Mais la méthode à nouveau employé par l'État, c'est de laisser croire que la colonne vertébrale, quelque part du développement en outre-mer passe par les grandes consultations seulement issus de nos territoires. Seront à l'inutile non et je ne souhaite surtout pas, mais ma crainte profonde celle créé finalement une espèce d'espoir qui est s'il n'est pas traduit budgétairement dans les années qui viennent va créer l'effet inverse va démotiver les territoires démotiver les populations et les élus auront à s'expliquer devant ses populations sur le résultat de ces consultations, lors de la présentation de son rapport, mon collègue Michel Magras disait après avoir auditionné rapporteur national des assises que le but fondamental de ces assises n'était pas tant de réitérer des préconisations déjà largement connu que de faire émerger et soutenir une nouvelle génération d'entrepreneurs ultramarins d'accord à son pourcent sur cet objectif, effectivement nous aurions souhaité par contre avoir des discussions en amont pour bien comprendre ce processus et les présidents de collectivités que vous avez reçu, Madame la Ministre, voulons également dit tout ce que nous disons sur ce sujet est avant tout fait pour nourrir le débat public et faire avancer les choses dans ce processus, ou non, une certaine vision des choses, il faut aussi tenir compte de ce que les collectivités ont déjà fait en matière de réflexion sur les territoires, cette absence de vision clairement définie, du côté de l'État donne aussi sentiment parfois de manière très insatisfaits insatisfaite que toutes les actions menées le sont comme une espèce d'empilement. Sans forcément cohérence sans forcément colonne vertébrale alors que le territoire engage un processus de programmation pluriannuelle, pour conforter leur développement économique, j'espère sincèrement que ses ambitions se traduiront budgétairement pour 2019, que ce soit pour la dans l'adaptation au changement climatique ou encore le développement portuaire en Outre-mer et je sais que ce thème vous tient également à coeur Madame la ministre, le groupe RDSE votera les crédits de la mission outre-mer car nous savons dans quelles conditions, vous les avez défendu mais ce budget de transition évidemment vous engage également pour l'avenir, à pouvoir traduire au niveau du résultat des assises budgétairement dans les années qui viennent, au travers du résultat des assises, des plans de convergence des prochains contrats développement toute la cohérence que l'État souhaite y donner pour autant, si ce vote et bienveillant dans les conditions dans lesquelles vous avez défendu ce budget, il y aura évidemment un certain nombre d'abonnements qui seront présentés cet après-midi, nous étudierons avec beaucoup d'intérêt, nous demandons à ce que l'État définisse une vision claire de ce qu'il souhaite pour les Outre-mer ce regard, il doit être un regard croisé et pas seulement un regard de l'outre-mer vers la métropole et c'est toute la difficulté, vous pouvez également vous appuyez bien évidemment sur cette assemblée dont sont issus des élus de territoire mais également d'instance comme le CSA pour définir des méthodes qui permettent une meilleure compréhension du processus, je remercie. La parole est maintenant à monsieur Jean-François jours pour le groupe Union centriste pour une durée de 8 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs Mimi chers collègues. Avant d'examiner les crédits dévolus pour 2018 à la mission outre-mer je tiens à remercier messieurs les rapporteurs spéciaux de l'excellent rapport qui nous propose ainsi que Madame le rapporteur pour avis, pour les travaux et l'analyse tout aussi approfondie qu'elle a fourni au nom de la commission des affaires sociales sur les crédits de cette mission budgétaire. Pour 2018, le budget de la mission outre-mer est maintenu au-dessus du seuil de 2 milliards d'euros, il est même en hausse de 85,1 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, ce qui représente une progression louable de 3,72 Cette hausse des crédits est un 1er pas d'autant plus encourageant que la projection pluriannuelle tablent sur une hausse globale des crédits d'environ 10 pourcent d'ici la fin du quinquennat. Restera donc Madame la ministre a à transformer l'essai lors des prochains exercices budgétaires de façon et ça a été répété à plusieurs reprises ce que les ambitions affichées en début d'année, à l'occasion de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, dite loi et Rome soit véritablement concrétisé au bénéfice de nos compatriotes. Mais disons-le tout de Go la suppression par le gouvernement des 22 millions d'euros de crédits affectés à l'équivalent fond Vert véritablement une erreur alors que la COB 23 il bien de s'achever que nous sommes à quelques jours seulement du sommet sur le climat organisée par le président de la République, comment pourrions-nous, Madame la Ministre, interpréter autrement cette décision. Créé l'an dernier, ce mécanisme dédié au territoire du Pacifique commence tout juste à produire ses effets. Consolidation de berge fragilisée par la répétition des catastrophes naturelles école bioclimatique centrale hybride Lampater lampadaires photovoltaïques réseaux d'eau et d'assainissement, équipement solaire etc ces investissements environnementaux engagé sur la seule année 2017, à hauteur de 12 5 millions d'euros plaide à coup sûr pour le maintien du mécanisme nous saluons donc l'initiative transpartisane de nos collègues députés grâce à laquelle l'Assemblée nationale, est parvenu à rétablir le fonds Vert cette décision devrait permettre d'assurer le financement de projets déjà engagés pour l'année 2018 et dont le coût avoisine déjà les 20 millions d'euros je poste notamment ici, à la gestion des déchets, les déchets aux Australes à la centrale hydroélectrique de Fatou, il va ou encore aux différentes centralisme hybride des îles Tuamotu, vous l'aurez compris madame laminé, mes collègues du groupe de l'Union centriste et moyens et moi-même veillerons attentivement au maintien de ce fonds, nous le jugeons indispensable aux collectivités françaises du Pacifique, nous regrettons par ailleurs que les crédits alloués louer au titre du fond d'échange à but éducatif, culturel et sportif soit simplement reconduits et non aussi. Alors que votre ministère s'était engagé à les doubler. Et allez doubler dès l'année prochaine, le nombre de billets délivrés au titre de ce fonds destiné à provoquer à promouvoir des échanges éducatifs, culturels ou sportifs, des habitants de territoires ultramarins vers la Metropolit ouvert les pays situés dans leur environnement régional. C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement de notre collègue Gérard Poadja visant à relever de 100000 euros, les crédits alloués à ce fonds. Et, de façon à ce que puisse également se font en bénéficier à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Nous avons conscience des territoires ultramarins ne souhaite pas être exempté de l'effort commun de redressement de nos finances publiques, mais ne perdons pas Madame la Ministre, le pari que nous avons pris de faire converger ces territoires avec ceux de la métropole des motifs de satisfaction existe par ailleurs et il mérite d'être souligné. Les crédits de paiement du programme 138 intitulé emploi outre-mer cérébraux, ainsi en 2018 à plus de 1,33 milliards d'euros d'euros, soit une hausse de 4,25 pourcent par rapport à 2017. L'effort porte principalement sur l'action de soutien aux entreprises qui représentent plus de 80 pourcent des crédits du programme. Au-delà, plus de 50 pourcent des crédits prévus au sein de la mission outre-mer porteront opportunément sur des mécanismes d'exonération de cotisations sociales à destination des entreprises ultramarines. Conjuguée au maintien à 9 pourcent du tome du taux majoré du C. I. C. E pour les Outre-mer ces aides devraient favoriser la production et le développement économique de nos territoires ultramarins. Mais si elle est un outil souvent efficace : la fiscalité incitative aussi de devenir rapidement inextricable la question de son éventuelle remise à plat devra, à cet égard étrave order dans le cadre des Assises des Outre-Mer. Il en va de l'aile d'illisibilité et de l'efficacité de notre politique économique et fiscale. Toujours au titre du programme, soit 138 nous saluons la concrétisation des engagements pris sur le Sénat ou service militaire adapté qui joue un rôle précieux dans l'insertion, de nombreux jeunes quant au programme 123 intitulé Conditions de Vie outre- mer il profite aussi d'une augmentation des crédits de paiement, auteur de 4,5 pourcent la progression des crédits et néanmoins inégale et varie suivant les actions du programme concerné. La ligne budgétaire unique dont la finalité consiste, rappelons-le, à répondre aux besoins de logement social recule ainsi de 1,57 pourcent cette baisse nous inquiète d'autant plus que l'augmentation des coûts de construction se poursuit et que la elle BU supporte des reste à payer et des restes à charge toujours substantielle le changement, le logement social est un enjeu particulièrement sensible en les outre-mer nous aimerions avoir donc quelques précisions quant à la stratégie du gouvernement dans ce domaine, pourquoi avoir baissé de 20 millions d'euros, les crédits alloués à l'Action logement, la stratégie du gouvernement vis-à-vis des territoires d'outre-mer doit reposer sur ses 2 jambes. Le Genk que sont effectivement l'efficacité économique d'une part et la justice sociale, d'autre part, ces quelques questions observations faut autant de pistes de réflexion nous attend 8 ont donc Madame la Ministre, allez prendre en considération parce que dans l'ensemble, nous y sommes favorables, le groupe Union centriste adoptera dans son ensemble, les crédits de la mission outre-mer je vous remercie, merci, cher collègue. La parole est à Madame Viviane pour le groupe, les républicains.

Madame la présidente, madame la Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs mais sa collègue l'examen de la mission outre-mer du projet de loi finance pour 2018 et est l'occasion pour les élus ultramarins que nous sommes, d'insister sur les priorités d'action à déterminer pour nos territoires aussi au travers des actions des différentes programmes de ce budget, je souhaite insister sur plusieurs points qui me tiennent à coeur : SIDA : des orateurs avant moi, ont rappelé les singularités de s'outre-mer j'assisterai naturellement sur la Réunion où le taux d'chômage est un fléau chez les jeunes mais qui frappe aussi les seniors, or les seniors sont les grands oubliés de ce budget, pourtant ce public peu ou pas qualifiés, peu mobiles et très éloignés du marché du travail va voir sa situation se dégrader encore, avec la baisse drastique des contrats aidés, alors même qu'un récent arrêté préfectoral est placée au coeur des publics éligibles au contrat unique d'insertion avec le bénéfice de mesures dérogatoires en terme de durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, madame la ministre, nous nous devons d'apporter à tous les réponses qu'ils attendent pour faire tomber les obstacles qui détiennent éloigné d'un emploi et les moyens mobilisés pour votre mission devrait répondre à cet enjeu. Le 2ème point que je voulais évoquer aujourd'hui porte sur la seconde partie de votre budget il y a pour vocation à améliorer les conditions de vie outre-mer, et plus particulièrement le logement je déplore que les crédits affectés au logement sont en diminution, puisque les autorisations d'engagement de l'action numéro un du programme, un, 2, 3, baisse de 8 pourcent soit 8 millions d'euros, alors même que la demande est forte, du fait notamment de la pression des pour moi, flic de la forte proportion de familles monoparentales et des disponibilités foncières concrète et des disponibilités foncières concrète mais au-delà des chiffres, il faut penser aux familles, être propriétaire de son logement est au coeur d'un projet d'une vie l'accession à la propriété est un enjeu primordial de la politique du logement et il nous appartient, Dédé, les ménages qui le souhaitent à devenir propriétaires de leur logement, ce parcours prend une forme singulière dans nos territoires, assis à la Réunion, il est fréquent que les parents cède une partie de leurs bien aux enfants, aux petits-enfants, ces derniers doivent pouvoir continuer à être aidés à la fois par la solde intergénérationnel et grâce aux opérateurs sociaux pour construire un logement de type LES je ne peux donc, mais qui était de la baisse du décidé de 13 millions d'euros, des crédits de l'accession à la propriété, Matignon plus que 7 millions d'euros, contre 20 en 2017, ce qui pénalisera fortement les plus modestes, il faut savoir à présent à l'esprit que dans les outre-mer, cette mesure va anéantir des projets de vie en excluant de nombreux emprunteurs et va fragiliser encore plus le secteur du BTP en impactant les programmes de construction alors que seule une politique de construction soutenu améliorera les conditions de logement et d'existence des ultramarins de même je regrette la chute du budget des aides à l'immigration de l'habitat privé ainsi que la baisse des aides pour la résorption de l'habitat insalubre, alors que les populations des outre-mer sont confrontés à des conditions de logement parfois très dégradé le budget baisse de 80 pourcent c'est un choix extrêmement regrettable la 3ème point que je souhaite aborder relatifs aux enjeux du développement durable de nos territoires et de préservation de l'environnement, cela passe par un développement de 2 méthodes d'économie circulaire sur des territoires souvent insulaire, donc les différences doivent être prises en compte dans le cas des orientations nationales,

Paris cela va directement entravé le développement des méthodes vertueuse de gestion des déchets, les territoires d'outre-mer doivent pouvoir réaliser des équipements indispensables au traitement des déchets équipements adaptés au contexte insulaire et à l'éloignement chez Koissy de l'Hexagone et de l'Europe afin de créer des outils de valorisation efficace et de contribuer à l'émergence de filières de recyclage, acteur d'emplois actuellement par exemple pour la Réunion 75 pourcent des déchets ménagers produit sur le territoire réunionnais vont à l'enfouissement, mode de traitement le plus critique dans la hiérarchie et s'agissant des déchets triés 90 pourcent des déchets sont exportés pour être recyclés en Asie ou en Afrique, il est donc important, madame la ministre, de s'attacher à préserver d'une fiscalité pénalisante des territoires comme la réunion afin de leur donner le temps de rattraper le retard dans la mise en des outils multi-filières indispensable, c'est le sens de l'amendement que j'ai déposée sur la première partie du PLF 2018 et qui a été adopté par le Sénat le 25 novembre dernier je demande donc pas le vol écologique et transition énergétique. Les assises de l'outre-mer puisse permettent de poursuivre les travaux sur ce sujet, enfin concernant nos jeunes, la hausse du budget du SMA est surveiller par cette structure est utile à plus de 6000 d'entre eux, et permet une insertion des volontés terre à hauteur de 80 pourcent mais alors pourquoi, dans le même temps, baisser les financements de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. il faut avoir à présent à l'esprit les difficultés des jeunes ultramarins pour se former et s'insérer professionnellement, hors de leur département d'origine, c'est l'ouverture vers l'extérieur de nos jeunes qui va t'être affectés, j'aimerais, pour terminer, souligner la disparition de la budgétaire du financement du plan Kenner devant aider au développement des équipements sportifs en outre-mer, il s'agit pourtant d'un enjeu important pour la jeunesse ultramarines, madame la ministre, des orientations budgétaires doivent intégrer les spécificités de nos territoires, qui font face à des défis de grande ampleur, à mon sens, ce projet de budget ne reflète pas les attentes que les habitants expriment pour une meilleure prise en compte de leur mode de vie et de leurs aspirations à plus d'égalité et de justice, aussi je ne pourrai voter pour ce budget qui une baisse de la ligne budgétaire unique et des critiques de la continuité territoriale, je vous remercie. Merci madame Mallet, la parole est à monsieur Dominique Théophile pour la République en marche.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 le volet crédits de la mission outre-mer s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros, il est donc sensiblement égale au volume global de 2017 blé on peut remarquer que ce budget n'a pas significativement évolué depuis ces 6 dernières années, le contexte dans lequel s'inscrit le budget des outre-mer et celui de la maîtrise des dépenses publiques en effet la croissance en volume des crédits de la mission, prévue pour 2000 19 et 2020, est inférieur aux objectifs de croissance de l'ensemble des crédits ministériels, cette perspective contraste avec les espoirs suscités de côté par le discours de responsabilité prononcée par le président de la République a Guyane et de l'autre par la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et ses objectifs de convergence, pas autant le rappeler que les crédits budgétaires ne sont pas le seul levier pour soutenir nos territoires et les politiques publiques en outre-mer, le budget de la mission outre-mer ne représente en fait que 12 virgule 25 pourcent de l'effort global de l'État en direction des collectivités, ainsi il faut également signaler que le montant cumulé des à destiné aux territoires ultramarins toute mission confondus, est en progression de 1,26 pourcent par rapport à 2017 pour atteindre 17 milliards d'euros, à ce titre, il est satisfaisant de constater dans le document de politique transversale que les engagements budgétaires de l'État sont en hausse, je retiendrai notamment au PLF 2018, une augmentation de 13,2 pourcent pour la santé 23,2 pourcent pour la transition énergétique pour l'écologie et l'aménagement durable et enfin 3,6 pourcent pour l'enseignement scolaire, nous sommes également satisfait de voir l'autorisation d'engagement, augmenté de 10 millions d'euros au sein du programme police nationale aux citoyens français des Outremers, je voudrais dire ceci : que l'État ne se désengage pas de nos territoires sous cette mandature, ce projet de loi de finances représente un soutien aux missions régaliennes de l'État en outre-mer, il nous faut maintenant investir une mutation tournés vers un développement économique, s'appuyant sur nos atouts territoriaux à l'analyse des crédits de la mission, il est prévu une hausse de 4,5 pourcent des crédits de paiement dédiée au programme 138 emplois outre- mer, soit 54 millions d'euros de plus, cet effort est porté essentiellement sur l'action, soutien aux entreprises, garantissant la pérennité des dispositifs d'allégement et d'exonération des cotisations dont bénéficient nos entreprises le programme permet également le financement d'une navette de fret qui voit son Champ d'intervention s'élargir, parmi ces éléments positifs se trouve le renforcement des moyens pour le service militaire adapté important pour notre jeunesse ainsi globalement ce budget va dans la bonne direction, cependant, permettez-moi, Madame la ministre, d'attirer votre attention sur certains points, d'abord, nous pouvons noter une stabilisation à la baisse des crédits alloués à la continuité territoriale, plus généralement, la baisse de près de 10 millions du budget de la donne était qui, alors que la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a élargi la mission de l'opérateur, notamment le déploiement de la mobilité autour retour qui est un impératif des territoires comme le mien, qui ont une démographie vieillissante en addition, le président de la République a promis de porter à 200000 le nombre de billets d'avion et des chaque année, en second lieu, je voudrais évoquer la faible participation de l'État concernant l'enveloppe destinée au sport, d'un autre histoire les Outre-mer, terre de champion mérite bien plus, c'est là une évidence, il est donc nécessaire de revoir en profondeur l'aide apportée aux actions sportives au profit de nos territoires, madame la ministre, un effort particulier me semble indispensable, je sais aussi pouvoir compter sur la détermination de notre ministre des Sports Laura Flessel pour inverser la tendance et faire en sorte que l'outre-mer, soit à l'image de la guerre, en effet, ce 1er budget de l'actuelle majorité peut-être considéré comme une étape vers un nouveau partenariat entre l'État et les collectivités d'outre-mer qui pourra trouver une source d'inspiration dans les conclusions des assises des outre-mer si chère au chef de l'État, en conséquence, nous espérons que ces assises ne sauront pas, une fois encore, l'occasion pour l'État de repousser à plus tard les obligations envers 6 territoires qui font la richesse de la France et son rayonnement à travers le monde les récents événements en Guyane sont là pour témoigner qu'une vraie réflexion est indispensable à la mise à niveau de nos départements, la situation économique de Mayotte est l'exemple type d'une France à 2 vitesses qu'il faut absolument rectifier un Guadeloupe j'ai ici même, appelé à une bienveillance du gouvernement sur la problématique de l'eau et des investissements nécessaires à réaliser pour en tenir en finir avec ce scandale à Saint-Martin et dans le sud Basse-Terre et cyclone Irma et Mariya ont montré qu'il convient désormais d'appréhender autrement la question des matériaux du type d'habitat et du plan d'aménagement du littoral, en outre, la situation du CHU de Martinique, placée sous administration provisoire et l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre, sont un grand coup porté au système de prise en charge sanitaire déjà fragilisé dans nos régions, vous l'aurez compris les besoins sont immenses et multiplie les volontés sont présentés afficher les politiques publiques se doivent donc être plus efficiente dans cette nouvelle logique de co-partenariat avec les collectivités locales, prônée par le chef de l'État, il nous faut faire mieux avec moins, madame la Ministre, mais soyez rassurés. Soyez assuré aussi de notre soutien politique, nous voterons ce budget 2018, qui est un 1er signe encourageant : il faut maintenant que se concrétise les ambitions formalisé par la loi relative à l'égalité réelle et que les perspectives qui sortiront des assises prenne véritablement corps nos territoires en besoin de concret et notre jeunesse de perspectives. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Monsieur Victorin Lurel pour le groupe socialiste et républicain.

Madame la ministre. Mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues. Comment parler de cette mission dans ce qu'on a été soi-même ministre des Outre-Mer d'exercice difficile. Les premiers exercices budgétaires d'un quinquennat sont toujours des symboles, on le sait, il concrétise des engagements de campagne traduisent une volonté légitime d'une vision aujourd'hui le budget des Outre-Mer le symbole à mon sens d'une résignation. Le symbole d'un désengagement, celui du gouvernement et de l'État, madame la ministre. De sa tribune, je ne me présente ni un nostalgique ayant cynique ni un aigri. Parce que je connais l'exercice qui est le vôtre, parce que je me refuse à verser dans la critique systématique. Et donc stérile, mais surtout parce que je souhaite sincèrement la réussite de feu qui pour les Outre-mer. Je suis des rares parlementaires qui ont gardé le silence jusqu'ici sur l'action gouvernementale, sauf à l'occasion de l'organisation des secours à Saint-Martin l'occasion moins des données aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, j'observe, comme l'assure. Sans jamais rien voir venir, loin d'être en marche, nous sommes à l'arrêt. Dans l'attente des assises 1er acte concret et tangible pour nos territoires, c'est donc ce budget. J'ai pour habitude d'Direct, franc et responsable, même si je suis trop souvent tenu par les Liens de l'amitié. Je ne me présente pas en vue d'une action gouvernementale donc je partage par ailleurs certains choix politiques Levallois ce moment d'être honnête, en affirmant que ce budget est décevant, il reviendrait au préalable, je tiens cependant à partager ressenti, Madame la Ministre. Je revendique les mots sont une arme et que les mots, bref, au-delà de l'inaction manifeste la rhétorique de l'État et procurer devenue offensante je vous ai écouté avec attention et je sais que vous prônez désormais la frugalité comme philosophie de l'action publique outre-mer

vous qui connaissez parfaitement des Outre-mer : comment pouvez-vous vous ni et la nécessité d'un État interventionniste outre-mer comment semblait ignorer qu'au vu des Anglais et des besoins, la politique de l'État outre-mer est largement sous-dimensionné, oui, j'ai le sentiment tenace que le langage évolue et que cette évolution n'est pas anodine, elle est insignifiante, que les mots, vie chère, lutte contre l'Argentine, ont disparu du vocabulaire gouvernemental que plutôt que de parler de convergence et donc de vision de long terme avec une trajectoire concertée stabilisé et sécurisé, nous renvoyons tous les problèmes à des assises qui prennent de plus en plus la forme d'appel à projets pour les premiers corps dès connaissant votre engagement et mesurant votre poids politique, j'ai donc la triste impression que des arbitrages ont été perdus, une logique exclusivement comptable de redressement de la prétendue hubris Brice budgétaire outre-mer a présidé à l'élaboration d'un budget atrophiée, à l'ambition minimaliste en somme la frugalité comme ligne directrice d'une politique, nous ne sommes pas dupes sur les chiffres qui nous sont présentés, nous demandons simplement de la transparence et de la sincérité sur les grands équilibres financiers de ce budget, mot que je crois que vous aimez bien

une fois n'est pas coutume les affichages budgétaire nominal s'amuse d'artifices de périmètre prétendant vous inscrit dans une démarche de sincérité budgétaire vous basez la hausse de Montpellier su Une exécution budgétaire et bien acter le transfert de crédits à d'autres ministères pour un montant de 90,4 millions en et 82 millions en CP, CP, mais tout à fait sincère, vous auriez dû aller au bout de cette logique en transférant les presque 85 millions d'euros qui figurent dans la mission au budget de l'Éducation nationale au lieu de cela, vous créez même une ligne budgétaire pour la construction de d'écoles, de collèges et de lycées à Mayotte en Guyane et en Polynésie pour plus de 50 millions d'euros, je dis cela vous fait comprendre qu'encore une fois nous un budget qui se verra certainement amputé par décret d'annulation de plusieurs millions d'euros d'ici quelques mois, mais au-delà de cette baisse, ce budget est l'illustration d'une philosophie budgétaire globale portée par votre gouvernement, une philosophie du rabot, du coup, terme quittera a demandé à tous les mêmes efforts notamment, on demande aux ménages pour mieux financer les entreprises, or vous le savez, à l'identique des situations différentes est une discrimination pire lorsque je lis le rapport spécial de notre collègue Georges Patient, j'apprends que je cite sur le triennal 2018, 2020 les crédits augmenterait de 0,5 pourcent en valeur, donc il y a parlé des flatteurs, donc l'augmentation de 3 pourcent en moyenne pour les missions du budget général, moi, ce que le budget général, en volume, donc les crédits devraient connaître une baisse de 2 ce budget frugale, le 1er du Nouveau Monde pour 2000 18 mai donc la première étape d'un désengagement programmé de l'État pour nos territoires cette trajectoire mortifère de pas possible, acceptable, je rappelle que l'État s'est engagé à hauteur de plus 2 milliards en faveur de la Guyane, plus une loi pour l'égalité réelle a été voté à l'unanimité du parlement et en accord avec tous les membres du gouvernement d'alors dont vous faisiez partie et que le président de la République s'est lui-même engagé sur plusieurs milliards de Madame la Ministre, comment puis-je vous dire budget qui consacrent la baisse des crédits à la mobilité comment suis voter un budget qui réduit de plus de 300000 euros le plan séisme sur ce point, je demande la clarté, on nous dit que cette baisse est à relativiser, puisque le Front national, on en clair, il faut conclure je conclus pouvez donc nous indiquer les lignes budgétaires qui confirmerait ses arguments : comment puis-je voter un budget qui sacrifie la Cité des outre-mer, comment puis-je voter un budget qui rabote de moitié des actions sanitaires, sociales, culture je n'ai 16 comment a fait voter un budget qui met à bas la politique du logement outre-mer du perd 21 millions d'euros on a soit moins 8 5 sur ces 21 millions ce serait 16 millions pour les crédits de rénovation de l'habitat privé, nous y reviendrons certainement lors du débat Madame la Ministre, et je conclus : nous ne pouvons pas attendent la fin des Assises pour répondre à l'urgence économique et sociale qui frappe les outre-mer tous les outils existent, la loi égalité a même prévu la signature de contrat de plan, donc on n'ont pas l'échec appuyez-vous que nous sommes voilà pourront pas le voter. Merci. Alors nous terminons cette série d'interventions par monsieur gros. Là où faut. Homme. Alors pour les républicains, pour une durée de 7 minutes, chers collègues, à vous la parole. La la présidente, madame la ministre, chers collègues, je tiens à saluer l'effort de solidarité nationale à l'égard des outre-mer, surtout dans le contexte actuel défend d'efforts budgétaires beaucoup a été fait pour aider à combler le retard structurel des collectivités du bout du monde, mais reconnaissons-le aussi parti nous partions de loin et beaucoup reste à faire, le budget qui nous est présenté montre montre combien notre ministre c'est défendant sa mission qu'elle en soit remercié étant le dernier match à m'exprimer, je veux pas répéter ce qui a déjà été dit mieux que je ne saurais le faire par les différents orateurs en particulier par les rapporteurs, dont je salue avec la gratitude l'excellent travail de présentation et d'analyse, permettez-moi que je me concentre sur Wallis et tournant, je soulignerai des points éminemment positif, ce qui n'empêchera pas que je soulève quelques inquiétudes. Un effort notable a été fait en faveur de Wallis et Futuna, Madame la Ministre, ces dernières années, à commencer par un rattrapage conséquents en matière de santé, je me souviens de notre ancien collègue Jean-Yves son qui est en visite sur le territoire, il y a quelques années, qui avait dit que notre hôpital n'était même pas au niveau d'un dispensaire de brousse, aujourd'hui nous avons. Quand même, et bientôt un centre d'hémodialyse tournant.

Victorin Lurel. Qui partagent nos banques désormais au plus tôt le fauteuil dans cet hémicycle les ateliers des assises outre-mer ne tiennent pas.

Je reste très optimiste, malheureusement, les grandes vacances de l'hémisphère sud, janvier, février raccourcissent le temps précieux de réflexion commune des assises. Les stratégies sectorielles notre stratégie globale. Peuvent être complétées par les ateliers qui, dans notre esprit, viennent donc compléter la préparation de notre futur contrat de développement 2019, 2023 l'actuel contrat hier était prorogée par avenant successifs, ceux qui, malgré les 5,8 millions d'euros qu'il convient de saluer avec gratitude demeure une dilution des moyens. Ce nouveau contrat développement sera notre chantier de l'année 2018, il serait souhaitable qu'il soit complété d'un contrat entre l'État et les circonscriptions permettant à celles-ci assurent leur mission de présence et de proximité auprès de la population, laissant mal, ouais, en investissement au titre des contrats de villageois était en diminution ces dernières années, laissant insuffisante, malgré les 500000 euros prévus pour 2018

Comme le service militaire adapté doit être également encouragé en 2017, trop peu de jeunes du territoire, on peut en bénéficier en Nouvelle-Calédonie, je profite aussi de l'examen de la mission outre-mer vous interpeller madame la sur l'aide au fret qui bénéficie encore très peu au territoire. Peut-on envisager une adaptation du dispositif pour pour qu'ils contribuent au développement de Wallis-et-Futuna, peut-on avoir des précisions sur la mesure, a ajouté dans la loi égalité réelle concernant le transport des déchets. Développement, voilà le mot maître celui qui conditionnent notre avenir, celle de nos enfants le développement passera aussi par une meilleure desserte aérienne pour désenclaver le territoire rwandais, l'appel d'offres. International : Madame la Ministre, enfin le développement passe par la venue de 2 missions que nous attendons, espérons-le, ne l'y avait qui semble bloquée par l'absence, par l'absence de financement des billets d'avion, espérons que ce détail puisse être résolu notre mission visant à analyser, à étudier les ressources halieutiques de nos eaux territoriales, condition nécessaire pour 100 dans le développement du territoire et pour tout accord de pêche pensez-vous Madame la Ministre, pouvoir la financer prochainement. Je vous remercie, je voterai la mission outre-mer. Merci que la. La parole est maintenant à Madame Annick Girardin ministre des Outre-mer, madame la ministre.

Madame la présidente, messieurs les rapporteurs spéciaux mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, si tous les Français, y compris les ultramarins sont appelés à consentir des efforts pour que le budget de la nation puisse être à la hauteur de nos engagements européens, le gouvernement a fait le choix de préserver la mission outre-mer, le soutien à l'emploi et à la jeunesse, l'accompagnement des entreprises, le développement des territoires. Autant de priorités réaffirmées ici, je vous remercie pour l'ensemble de vos observations pertinentes et légitime et je vous redis que le budget que nous présentons aujourd'hui est très positif, il adhère aux mesures de redressement des finances publiques, porté avec détermination par le gouvernement. Ainsi, dans le contexte d'une réduction de 7 milliards d'euros de dépenses. Vous avez pu constater que les crédits de la mission outre-mer sont en hausse de 4 pourcent soit 85 millions d'euros on crédite dément. monsieur le sénateur Artano merci de saluer l'effort de sincérité. Oui, de sincérité parce que contrairement à ce que j'ai pu entendre, je le dis clairement cette hausse, elle n'est pas virtuel.

rétrocédés au ministère d'Éducation nationale en début de l'année 2017 ces crédits n'avait donc pas vocation à rester dans le périmètre de la mission, ils sont d'ailleurs en 2018 intègre allemand reconduit dans celui d'éducation nationale. Sur la base des crédits dont j'la responsabilité, je répète, c'est donc bien plus de 85 millions d'euros, soit 4 pourcent d'augmentation. Cette hausse de crédit consolide pour les années à venir, les fondamentaux de l'action du ministère des Outre-mer, il était très important pour moi de pouvoir donner ce 1er signal dans ce début de quinquennat non monsieur le sénateur Lurel ce budget et tout. Sauf une résignation, ce n'est pas non plus d'ailleurs, un budget d'Atlantis, mais le début d'une nouvelle impulsion. Monsieur passation monsieur oui le début d'une nouvelle impulsion, car ce n'est pas un budget qui stagne, mais c'est bien un petit ornementation j'ai entendu les inquiétudes qui ont été formulées ces dernières semaines dans la presse à l'Assemblée nationale sur les territoires, à l'occasion de mes déplacements ici même il y a quelques instants sur l'ensemble de ces ventes je tiens ici à vous rassurer et à vous apporter toutes les réponses nécessaires à la bonne compréhension de l'action de l'État, il faut dire ce que l'on fait, c'est pourquoi je souhaite m'engager résolument en dans un discours de vérité, de dignité, de transparence avec les outre-mer et ce n'est pas et je ne vais pas rentrer. Dans les jeux de posture politique avec qui que ce soit dire avec force et fierté, tout ce que nous faisons mais aussi bien sûr convenir, très honnêtement, tout ce qui va nous rester à faire, se félicitait de ce qui fonctionne. Mais aussi constaté ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, ce qui mérite d'être interrogée. Assumer tout ce qui relève de notre responsabilité, mais aussi cesser d'agir ou de décider, lorsque l'État n'a pas vocation à intervenir localement, j'insiste, les collectivités territoriales, notamment outre-mer dispose de compétences essentielles et de plus en plus large, d'ailleurs, en matière de formation professionnelle, d'insertion, de gestion des services publics fondamentaux de transport. Il ne faut pas l'oublier. Il nous appartient donc de les accompagner dans l'exercice de leurs compétences. J'ai pris des initiatives en ce sens dans le cadre de la conférence nationale des territoires en proposant notamment qu'une plateforme depuis, on a ingénierie soit développée au profit des collectivités et des élus locaux, nous devons renouer une relation de confiance réciproque avec les élus et les populations ultramarines qui attendent beaucoup et en raison de l'ensemble des décideurs publics ai j'a annoncé qu'avant la fin de l'année, un site internet sera à disposition du public afin de permettre à tous de constater les mesures prises et celles engagées dans le cadre par exemple du plan d'urgence pour la Guyane. Cette initiative, je la conçois comme une première étape vers plus de sincérité de notre part. Ceci d'ailleurs a vocation à trouver l'ensemble des dépenses en faveur de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Nous vous devant cette transparence dans tous les domaines, budget, suivi de la loi Égalité réelle engagement pris en faveur de Saint-Martin. Je souhaite bien entendu. Qu'il en aille de même pour la mise en oeuvre de la loi Égalité réelle en outre-mer, cette loi, nous la mettre en en oeuvre et j'ai demandé à mes services de se mobiliser en ce sens les choses avancent peut-être pas assez vite déjà la loi financière de cette fin d'année, porte un grand nombre de dispositions prévues dans la loi, hier près de 20 pourcent des décrets d'application ont été pris plusieurs doivent encore l'être avant la fin de l'année, je comprends votre impatience mais rappelons-nous que cette loi n'a que 9 mois et si j'ose le temps de la gestation. Aussi, je veux insister sur quelques points Madame allez le ministère des Outre-mer n'pas seul. Dans cette belle mission que le développement des territoires. Et la satisfaction des besoins essentiels des populations, c'est le cas bien sûr des politiques en faveur des seniors qui relève du ministère des solidarités l'action des autres ministères en faveur des autres maires se renforce et les chiffres du document de politiques transversales confirme ce document qui recense les crédits de 87 programmes différents, fait état d'une augmentation de 336 millions d'euros entre 2017 et 2018, soit plus de 2,2 Si le. Ne couvrent pas l'intégralité des dépenses publiques, voilà il fournit quand même une bonne vision de l'effort strictement budgétaires des différents périmètres ministériels, soit 17 milliards d'euros pour 2018 merci, monsieur le sénateur Théophile de l'avoir rappelé cet effort, j'ai souhaité qu'il soit inscrit dans la durée, la programmation des crédits outre-mer prévoit une augmentation d'environ 5 pourcent. Entre 2017 et 2020 et de 10 pourcent à l'horizon 2022 alors dans d'autres temps en promettez 12, mais en réalité, il y en avec 5 hé bien gênant 5, il y aura 5. Je sais, Monsieur le Sénateur, Languedoc, comme vos collègues vous verrez accepte que cette programmation soit respectée. Je sais que vous soutiendrez tous cette augmentation future, mais je veux dire aussi que le président de la République s'est engagé en ce sens avec une parole forte, pas de promesses non tenues trop souvent les outre-mer ont été déçus de voir les promesses de rester lettre morte parce que non financées. Président de la République s'est également clairement exprimée pour indiquer que le prochain PLFSS aurait vocation à traduire financièrement les conséquences des assises. S'y ajoute, bien sûr, les plans et les contrats de convergence prévue par la loi et robes et dans la signature doit intervenir l'année prochaine les assises nourriront le contenu bien sûr de ses réflexions et de ces discussions mais ne vont pas se substituer la convergence est cependant parfois une notion complexe et vous le savez, notion complexe à cerner je mens je n'en remets pas en cause la portée bien sûr, mais je veux aussi que nous ayons des échanges francs sur son contenu, pour ne pas être dans la jonction pour ne pas empêcher les territoires de définir des aspirations et des stratégies distinctes adaptée à chacun d'entre eux. Pour l'heure, le budget 2018 nous permet de construire une politique cohérente et volontariste, j'ai défini 3 priorités : la le développement des territoires, les engagements des contrats de plan de développement, État, collectivités, célébrant à 152 millions d'euros, soit 12 pourcent d'augmentation par rapport à l'année passée, je vous parle de route, bien sûr, de ponts, de réseaux d'eau potable de filières de gestion des déchets, car oui, Monsieur le Sénateur, passion les outre-mer ont des retards structurels importants et notamment votre territoire qu'il nous faut bien sûr c'est l'objet d'ailleurs des contrats de convergence qui sont à venir. Pas plus qu'au cours des précédentes mandatures, le fonds exceptionnel d'investissement maintenu intégralement à 40 millions d'euros n'a vocation à résumer l'effort de l'État en matière d'investissement publics au-delà des différents outils de la mission outre-mer, le président de la République s'est engagé à ce que les outre-mer bénéficient, je le rappelle, d'un milliard d'euros d'investissement au titre du grand plan d'investissement, il vous sera rendu compte régulièrement de ces crédits. 2ème priorité la jeunesse vous savez l'attachement que je porte, je veux rappeler ici l'augmentation des effectifs, comme vous l'avez fait de service militaire, du service militaire adapté 127 emplois supplémentaires sur le quinquennat va dès l'an prochain, cette semaine, même le 1er ministre s'est engagé à développer les capacités d'accueil du SMA en Nouvelle Calédonie, la jeunesse, c'est aussi le fait, il sera bien doublé l'annonce a eu lieu, bien sûr, et malheureusement après l'apparition des documents budgétaires, le nombre de trajets passera bien de 4000 à 8000 je vous rassure, Monsieur le Sénateur, alors s'agissant de la daube vous a été, vous avez été nombreux à Madické votre préoccupation. Effectivement, vous avez pu avoir un certain nombre d'interrogations, je vous ai entendu et je vous êtes confirme que l'ensemble des besoins présents et à venir seront financé et mis en oeuvre, monsieur le sénateur Théophile, vous pouvez compter sur moi. La loi et Rome a élargi les dispositifs de quantifier territoriale, ces mesures entreront progressivement en vigueur et nous serons au rendez-vous de ces enjeux essentiels pour les jeunes de nos territoires. L'emploi, enfin vous l'avez vu, plus de la moitié du budget concerne le remboursement d'exonération de charges pour les entreprises, ces dispositifs couplé au maintien en 2018 du CICE majoré à 9 pourcent en mer sont essentielles à la compétitivité des entreprises et à la préservation de l'emploi, mais au-delà de la préservation de ce dispositif, parce que les échéances, le contexte nous oblige à penser l'avenir, je veux aussi évoquer avec vous, plusieurs projets que je porte aujourd'hui la réforme des aides aux entreprises, l'économie est au coeur des assises. Sans économique, pas de perspective d'avenir, pas de cohésion sociale. Mais je l'ai dit, on ne peut pas penser l'économie d'aujourd'hui, comme on le pensait hier nos sociétés en changer, il faut préparer les Outre-mer à affronter l'avenir, clarifier, rendre lisible les dispositifs protéger et soutenir les entreprises outre-mer, elles en ont besoin mais aussi soutenir l'innovation et la recherche pour construire l'économie de demain, voilà mon ambition. Ce n'est ni un coup de rabot. L'immobilisme, ce n'est pas l'ADN de ce gouvernement et c'est surtout pas le mien. La méthode du gouvernement c'est la justice, la sincérité, c'est aussi l'audace. Je veux des outils modernes ciblées. Et je souhaite qu'il soit inscrit au budget de 2019. Cantonné de l'importance de ces sujets, le temps de la réflexion n'était pas super et c'est de réflexion certaines

autre projet, autre ambition repenser globalement la priorité que constitue la politique du logement outre-mer. Oui, madame la sénatrice dada, oui madame la sénatrice qu'connaît oui madame la sénatrice mal, j'ai entendu les critiques et inquiétudes que suscite le budget 2018, la capacité d'engagement de la LB, il a été réduite de 20 millions d'euros dans 2 domaines ciblés, l'aide à la rénovation pour les propriétaires occupants et l'aide à l'accession sociale, je ne vais pas ils aient esquivé le sujet, ce n'est pas la première fois que ces dispositifs sont rationalisées. C'était le cas en 2015 et il y a eu aucune diminution sur les territoires occupés, aucune dynamique n'a été en ce que je souhaite c'est que partout où cela est possible, les Outre-Mer bénéficient, comme l'ensemble des territoires de la République des dispositifs de droit commun, quand ils existent, il faut les utiliser, ce sera une de mes priorités en 2018, mais le choix que j'ai fait et que j'assume si la construction neuve 400 logements supplémentaires par an à compter de l'année prochaine et des crédits de paiement en augmentation de 28 millions d'euros sur cette ligne. Bon choix, c'est aussi la réhabilitation des logements insalubres. Le PLF 2018. Le concrétise pas un Euro d'économies sur cette ligne, maintien du fonds Barnier pour la démolition de l'habitat informel dans les Dom, maintien de dispositifs fiscaux avantageux pour les propriétaires occupants. Mais vous avez raison Monsieur madras Madame Dindar. Il faut pouvoir aller encore plus loin, je suis d'accord aussi que notre capacité à construire n'est pas qu'une question budgétaire. Foncier norme agrément programmation adaptée. Tous ces chantiers, je les ai pris à bras le corps, dans le cas de la stratégie nationale pour le logement. 3ème ambition : faire des autres des. Précurseur dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, les 17 Objectifs de développement durable et plus particulièrement l'adaptation défis aux effets du changement climatique, pourquoi j'insiste, ce soir, sur ces 17 Objectifs de développement durable, la France est engagée en 2015 on y trouve la santé, on y trouve l'éducation, on y trouve l'égalité hommes-femme tous les sujets de développement concernant les territoires d'outre- mer se trouvent dans des 17 Objectifs de développement durable, oui madame la sénatrice ainsi les Terres et les terribles événements climatiques qui ont affecté les anti et, notamment, Saint-Martin Saint-Barthélemy en septembre, nous en cruellement rappelé. L'urgence à agir. Le budget du ministre du ministère de l'Outre-mer a largement contribué au financement des mesures d'urgence, notamment par le biais du Fonds de secours mon budget sera abondé en conséquence parce que vous savez que la somme a largement été débordé de 3 1000033 pardon millions. D'euros on a eux ont fr et à la fin, dès la fin de cette année, j'ai par ailleurs, annoncé à la. Saveurs de cette discussion budgétaire, la création d'un fonds pour la réhabilitation des logements privés, axée sur les risques sismiques et cycloniques de 5 millions d'euros dès 2018. L'actualité ne nous permet plus d'attendre, je l'ai déjà largement celle qui a participé au à la préparation de la COP 21, souhaite que les territoires d'outre-mer, soit des exemples en matière notamment d'adaptation. fois, il va falloir que l'on puisse emmener effectivement cette dynamique, les collectivités du Pacifique bénéficient d'un mécanisme de prêts à taux 0, vous l'avez rappelé pour accompagner leurs projets environnementaux, mon souhait est double, Monsieur le Sénateur, enjeu ciblés, plus encore qu'on ne le fait actuellement, nos crédits à l'adaptation, changements climatiques. Tout simplement parce que nous parlons tous d'atténuation mais rarement d'adaptation et je souhaite aussi que se font ces avantages qui s'est étendue à l'ensemble des territoires d'outre-mer. Je ne veux pas y travailler seul, mais avec mes collègues au sein d'un du gouvernement et avec les territoires car soyons clairs, les enjeux sont tels que c'est pas. Le budget du ministère de l'Outre-mer ou mystère d'autres maires qui pourra seul répondre à l'ensemble de ces défis, nous allons pouvoir y répondent que par un fonds qui serait interministériel et inter-agences.

La réforme des aides aux entreprises est nécessaire et le secteur du tourisme doit être largement soutenu parce que c'est un fort pourvoyeur d'emplois et de développement dans les territoires d'outre-mer, le temps des assises est nécessaire. Pour concrétiser ou pour construire ou co-construire la réponse. Le 1er, le président de la République l'a dit, nous ne verrouille pas les assises. Par des considérations budgétaires. Oui, Monsieur le Sénateur. Dany oui, Monsieur le Sénateur, passion. Il y a une possibilité d'évolution institutionnelle, le président de la République a indiqué qu'il était ouvert aux évolutions en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, et nous le ferons sont bout et nous ferons avec vous, si c'est nécessaire. Mais la réponse institutions. Elle Elle sera présente que si elle est souhaitée. D'abord que ce qu'elles soient pertinentes et ensuite souhaité. Par un consensus au plan local, la Guyane notamment organise actuellement les états généraux, nous suivons de près l'ensemble de ces débats. Sur la santé, vous m'avez aussi interrogé, vous évoquez madame la sénatrice. La crise de 2017. Depuis ses 85 millions d'euros qui ont été mobilisés sur les questions de santé et notamment pour les puisse hôpitaux. Pour Mayotte le CHU, c'est 170 millions d'euros mobilisés pour la Guadeloupe, la crise provoquée par l'incendie, il y a quelques jours, du CHU nous oblige, on nous a obligés. à une réponse rapide et demain, c'est 550 millions d'euros qui viendront pour moderniser les établissements hospitaliers. Alors il faut aller plus loin et c'est dans ce cadre que la ministre de la Santé a souhaité que la réflexion nationale. Prennent en compte également les territoires d'outre-mer. Est prête, la question de la mortalité infantile du diabète, de l'éducation à la santé. Le plan, développement des équipements sportifs en outre-mer. Il est pas supprimé Madame quand connaît. Notre déplacement chez vous. En Guadeloupe, ou plus largement également pardon à la Martinique Monsieur Lurel en Guadeloupe pour vous à la Martinique, ou encore à Saint-Martin a été l'occasion pour la ministre des Sports. Et de rappeler que son enveloppe de 10 millions d'euros pour 2028 2018 partants était bien maintenu. Et en ce qui concerne les crédits du ministère de l'Outre-mer, ça a toujours été sur la feuille que le complément étaient donc je vous rappelle 10 millions d'euros, confirmée par la ministre des Sports, plus un abonnement complémentaire. Dans le cadre de du FAI, quand ce sera nécessaire sur les différents projets. Monsieur Vignon je connais votre tragiquement pour l'outre-mer pour avoir accueilli chez moi à Saint-Pierre. Et Miquelon mais aussi avoir suivi votre parcours dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, les assises devront traduire l'espérance. Mais oui, je veux faire émerger. L'Outre-mer, des solutions parce que oui, il y a des défis, oui, il y a des difficultés mais il y a aussi des solutions qui ont été trouvés dans les territoires d'outre-mer et qu'il nous faut partager, partager entre autres mais partagée aussi plus largement. Vous êtes tous les bienvenus. élus, acteurs locaux socio-professionnels à participer à cette co-construction dans le cadre des Assises des Outre-Mer. Je souhaite que vous soyez nombreux n'attendez pas les habitations parce que sur tout les territoires, les débats se font. Et surtout, les territoires, l'information est à la disposition de l'ensemble regroupe des élus en dehors de ce qui est bien sûr organisée. Certains vous m'avez questionné sur la visibilité ou la lisibilité des territoires d'outre-mer. Est une priorité pour moi en parlant. France O et de la Cité des outre-mer, d'autres d'ailleurs en citer également ce projet de Cité des outre-mer d'abord vous dire qu'il n'est pas question pour moi de supprimer France ni d'ailleurs pour la ministre de la culture, je vais aussi vous dire qu'il est extrêmement important et je l'ai déjà dit que dans l'ensemble des territoires d'outre- mer, les chaînes premières. Puise rayonner sur l'ensemble de leurs bassins maritimes mais puissent aussi être des forces de production dans l'ensemble des pays voisins pour faire que ces chaînes premières produisent des émissions qui soient vus, non pas que sur France O mais aussi sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions, voici notre combat, voici un combat commun que nous devons avoir, parce que oui, il faut davantage vers les autres maires en métropole, hé oui, il faut que ce soit. L'ensemble de la France qui découvrent nos territoires et la richesse de ces territoires. La Cité des outre-mer, c'est aussi la question de la visibilité de la visibilité, la lisibilité des outre-mer ce projet pour moi, je suis arrivé, le ministère des Outre-Mer avait effectivement prévu une enveloppe pour rénover un bâtiment pour y installer la Cité des outre- mer un projet culturel son ministère de la culture à projets culturels sur la région des de France. Un projet culturel, effectivement, soutenu par la mairie de Paris, alors moi j'ai souhaité que nous puissions puissions travailler davantage ensemble. La région Île-de-France a déjà signalé sa volonté d'y revenir, revenir à la table de la discussion revenir penser. Le projet Colin sinon mieux. Voir les outre-mer et je crois que c'est important de dire que je tiens à ce projet. Je tiens à ce projet, mais il devra être plus collégial et ceux qui s'inquiètent et notamment les acteurs locaux, moi aussi, dit discrètement que jamais, ils ont été associés à ce projet, alors voilà ce que je veux, je voulais vous dire et j'espère avoir été effectivement rassurant pour un certain sur un certain nombre de points, je voudrais finir en disant que certains m'ont interrogé sur. Le changement de rhétorique ben oui, le changement de rhétorique, il est là, ça s'appelle la sincérité, la justice et l'audace, le changement dérange toujours, mais je l'assume et je l'assume, le projet de loi de finances pour 2018 fournit des outils essentiels, nous devons rendre à l'Outre-mer. Ce que je viens de vous dire la lisibilité et la visibilité, merci de votre attention et merci de votre vote

D'objectifs et et de performance, assigné à la à la Dome, nous proposons que du programme 138 138 vivement de crédit au programme 123 de 5 millions d'euros pour répondre aux obligations nouvelles obligations de la Dome pour permettre de prendre en compte cette nécessaire obligation pour nos jeunes pour les déplacements et la formation, la continuité sur Victoria. Merci, cher collègue, avis de la commission. Si je souscris, l'objectif de l'auteur de l'amendement de renforcer l'air de la continuité territoriale, qui connaît une baisse dans le présent projet de loi de finances, il me semble opportun de réduire les crédits du programme 138 puisqu'il finance les exonérations de cotisations sur Canal et l'aide aux frais des entreprises, une baisse de ses dépenses qui correspond à une prévision d'exécution puisque vu exonérations sont de droit serait irréaliste et ferait perdre sa sincérité au projet de budget, alors je demanderai à l'auteur de l'amendement de le retirer, dans le cas contraire, la Commission émettait un avis défavorable. C'est monsieur le rapporteur, Madame la ministre pour la avis du gouvernement. Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, votre préoccupation, je l'ai dit tout à l'heure est parfaitement légitime et et j'y suis sensible, la mobilité, la formation sont des enjeux majeurs pour nos territoires mais comme indiqué dans mon intervention, les besoins de l'agence sont intégralement couvert pour le projet, budget 2018 et l'activité de la Dome ne connaîtra aucun recul en 2018 tous les indicateurs sont en progression énorme en 2017 et nous maintenons le niveau élevé de notre participation à la donne à la dame, c'est-à-dire exactement la dépense de l'an dernier et nous serons présents pour abonder au fur à mesure les crédits si nécessaire selon effectivement les besoins, je vous demande donc de retirer retirer votre amendement, à défaut, ce sera un avis défavorable du gouvernement merci. Si madame la ministre, chers collègues souhaitent une explication de vote d'abord. je comprends bien, il est demandé donc aux collectés au fil de retirer donc cet amendement mais en fait, je profite de la tribune pour dire qu'au-delà des crédits affectés en plus ou en moins ça la donne, c'est l'image même de la donne qu'il faut réhabiliter parce que la donne est un outil et je sais de quoi je parle, j'étais exécutif pendant longtemps je travaille que cette structure aujourd'hui la Dorna plus les moyens de sa politique, il faut le reconnaître, la donne n'est plus attractives, alors que nos jeunes ont besoin d'avoir une structure qui les protège, surtout lorsqu'il se déplace, n'oubliez pas, ce sont souvent des heures, des jeunes qui sont déracinés déstructurés qui viennent, ne serait-ce que pour 3 4 6 6 6 mois et souvent lorsqu'ils arrivent en France hexagonale, il ne trouve pas le lieu pour pouvoir se faire, ne serait-ce que se loger, il reste parfois, je connais des jeunes de la dame qui sont restés parfois dans la rue pendant des jours et donc c'est ce plaidoyer que je fais pour qu'on puisse prendre en compte cette structure, on ne peut pas d'un côté dire qu'on veut faire de l'insertion professionnelle et vous savez combien le chômage touche nos outre-mer et particulièrement la Guyane, presque 50 pourcent des jeunes sont difficulté en sont au chômage, alors c'est un plaidoyer pour la donne que je fais aujourd'hui, on ne puisse pas dire en vente pour des raisons budgétaires, je peux bien comprendre de crédit et de transfert, Madame la Ministre, vous avez bien dit que vous allez prendre en compte et en considération cette structure j'attends maintenant que l'on puisse le faire de façon très concrète, je ne suis pas Saint-Thomas. Merci Monsieur Karam, est-ce que Monsieur Lurel a demandé la parole. parole. Présidente, Madame la Ministre et cher collègue, l'existence de ces amendements prouve bien l'insuffisance du budget. Ces amendements étaient présentées par la majorité soutenant et votants tout à l'heure, ce budget et il y en a d'autres, en plus des contrats aidés, il y a plus de près de 9 millions pris sur le budget de la année il y a une philosophie derrière qui est gênante, on nous dit les avions low-cost sont arrivés. Et donc on peut diminuer le budget et donc l'exécution budgétaire peut-être revu et donc à la baisse alors que le président proposé 200000 billets, on est très très loin du compte et je finis, madame la présidente, sur une chose : le président de la République, on a essayé toutes les lettres tous les engagements, a dit à l'hebdomadaire actu en Nouvelle-Calédonie que nous participerons au GP de 50 milliards maintenant c'est 57 milliards ça ferait plus de 2 milliards et qu'en plus ils pensent pouvoir mais dans les plans de rattrapage, je cite, un milliard, sans compter le milliard de la Guyane, ça vous fait 3 milliards 0 dans le budget, on aurait pu mettre des autorisations d'engagement et faire la programmation non, on attend des résultats hypothétiques des outre-mer alors que toute l'armature toute l'architecture du développement à long terme est contenue dans la loi égalité oui la rhétorique a changé, le Père Noël, la frugalité non je me sens offensé, je le dis très clairement la les les outre-mer ne sont pas des assistés on ne sommes pas des enfants, ce discours défend-il ils Sion n'est pas de mise. Merci, cher collègue sur cet amendement, chers collègues est-ce que vous souhaitez le retirer ou vous le maintenez. Rapidement, en fonction des explications fournies par Madame la Ministre, seront très vigilants et très attentif, donc nous retirons l'amendement. Merci, cher collègue. Donc il est repris. J'ai vu, est-ce que Madame Joly. Je ne connais pas Monsieur le raid. Il est repris à ce moment-là, il n'y a pas de problème, maintenant, vous avez déjà pris la parole, donc vous n'avez normalement plus le droit de vous exprimer mais vous l'avez repris. C'est fait, donc il est repris par Monsieur Lurel. Donc nous avons sur cet amendement, un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement, nous le mettons je vois

Qui s'abstient. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons maintenant à l'amendement 556 rectifier, il est présenté par Monsieur

en consacrant 5 millions d'euros qu'il convient de transférer des crédits de l'action numéro un du programme 138 vers l'action, numéro un du programme 123 consacré aux conditions de vie outre-mer. Merci monsieur Vignon, avis de la commission. Il a aussi l'intention de faire encore une fois, louable, il n'apparaît pas réaliste de faire baisser les crédits de l'action 01 du programme 138 qui finance l'exode, les exonérations de cotisations sociales et constituent donc des dépenses contraintes, je précise, même si cela reste très insuffisant, que le présent projet de loi de finances étant certains crédits dans d'impôts et des dispositifs de défiscalisation Outre-Mer aux travaux des réhabilitations, contre le risque cyclonique, alors je demanderai, là aussi, de retirer l'amendement autrement, la commission des finances, a émis un avis défavorable. Merci, cher collègue, Madame la Ministre votre avis. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Bignan votre moment reprend effectivement une proposition qui a été débattu à l'Assemblée nationale et qui souhaite étant de les crédits du logement du ministère et que ceci soit fléchées, surtout sur la rénovation des bâtiments et leur adaptation au changement climatique cet amendement a été retiré à l'Assemblée nationale, parce que comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, dans mon discours, j'ai pris l'engagement d'y mettre pour l'année 2018, 5 millions d'euros et nous verrons avec le temps et l'évaluation de ce nouveau dispositif, comment nous pouvons l'abonder dans les années à venir, merci de retirer votre amendement dans le cas contraire, ce sera un avis défavorable. Je le retire. Très bien, merci Monsieur l'amendement 556 rectifier et retiré, nous passons à la présentation de l'amendement 188 rectifier qui est présenté par Monsieur Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement propose d'affecter 4 millions de d'euros supplémentaires au programme 138 à l'autorisation d'engagement, les crédits de paiement afin de pouvoir créer une dotation au CCI d'outre-mer, celle-ci est destinée à compenser l'impact de la baisse de ressources fiscales de 17 pourcent prévus par l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 plusieurs raisons justifient cette dotation d'abord la sensibilité particulière des tissus économique des drônes à l'action des CCI, du fait d'une part plus importante des ventes d'entreprise unipersonnelle nécessitant un accompagnement plus prononcé et, d'autre part d'un dynamisme entrepreneurial plus important ensuite la perte progressive depuis 2010 de concessions sur la gestion des grands équipements qui a durement impacté le budget des CCI ultramarines faisant passer leur volume budgétaire de 300 millions d'euros dans le cas de Rome en 2010 à 117 millions d'euros en 2015, enfin, parce que des économies plus difficile à réaliser dans ces 6 pays compte tenu de la taille des territoires et de l'absence d'établissements frais régionaux qui pourraient être fusionnées établissement puis publique de l'État, les chambres de commerce et de ministres, ils sont les représentants élus du secteur économique et remplissent des missions de service public vital à l'activité économique comme l'accompagnement des créateurs d'entreprise, la formation professionnelle, l'accompagnement et à l'international nationalisation, les centres de formation des apprentis consulaires, etc, une nouvelle baisse aussi substantielle de de leurs ressources de fonctionnement aboutir et par conséquent nécessairement à une dégradation sensible de la qualité du service public prodigués aux entreprises ultramarines et à des suppressions d'emplois, faute de pouvoir isoler les CCI d'outre-mer dans le mécanisme de plafonnement des taxes affectées prévue à l'article 19 du projet de loi de finances, il est proposé que le ministère des Outre-mer compense l'impact budgétaire à due concurrence, cela prendra la forme d'un transfert de 4 millions de d'euros de l'action de du programme 123 vers l'action du programme 138, il est en effet possible de financer cette subvention par un phasage dans le temps, différent du paiement de contrats liant l'État et les territoires fort cette année de plus de 152 millions d'euros mal et de plus de 153 millions d'euros en CP. Merci, cher collègue, l'avis de la Commission, monsieur passion. On est toujours dans la même configuration, il s'agit de transfert de crédits là au détriment de la politique contractuelle de l'État en outre-mer, là aussi, je demanderai à monsieur vous allez de retirer son amendement autrement, la commission des finances, a émis un avis défavorable.

celle de territoires d'outre-mer qui sont extrêmement fragiles et elles sont essentielles au service des entreprises mais je le répète ici : le ministère des Outre-mer n'a pas vocation à contribuer au financement des CCI c'était des établissements publics dans le môme n'assure absolument pas la tutelle mais je veux aussi rappeler que le ministre de l'action et des Comptes publics l'a redit la contribution demandée à l'ensemble du réseau sera limitée à la seule année 2018 et que il y a aussi un dispositif de péréquation qui va être mis en place pour effectivement soutenir les CCI, les plus fragiles, alors j'espère que ce dispositif de péréquation viendra aider les plus fragiles des CCI et donc les CCI d'outre-mer, je vous demande de retirer votre amendement dans le cas contraire, c'est un avis défavorable. Alors, Monsieur Mohammed Oui, fort de ces explications de madame la ministre, et dans la mesure où mon intention était vraiment de porter l'attention sur cette problématique des CCI je retire mon amendement. Merci, cher collègue, l'amendement 188 rectifier et donc retirés, nous passons à l'amendement 513 rectifier qui est présenté par Monsieur

Merci dans la présidente, madame la ministre, chers collègues, effectivement, j'ai bien entendu dans le discours de Madame la Ministre tout à l'heure, l'intérêt très vif qu'elle porte sur les questions de jeunesse son souhait également de voir se développer les échanges, notamment à travers la mise en oeuvre du du fait Bex qui fut instituée par la loi d'orientation de de 2000 et qui a été revisité ou améliorer lors de l'examen du dossier sur l'égalité réelle, l'année dernière dans le projet de loi sur l'égalité réelle des outre-mer et donc je me suis volontiers associés à cet amendement comme un certain nombre de collègues du groupe de l'Union centriste de Gérard Poadja qui, bien entendu, je souhaite que l'ensemble des populations françaises puissent bénéficier des échanges comme cela se fait naturellement aussi sur le territoire européen à travers des programmes européens du TP Rasmus mais ici c'est bien de permettre à l'ensemble des populations françaises de pouvoir en bénéficient, or jusqu'à présent, il apparaît que les populations de nouveau de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en serait exclus, donc il y a pas de raison qu'elle ne puisse profiter de de ces mesures que l'on souhaite tous voir mises en oeuvre et c'est pourquoi cet amendement a été présentée avec une imputation de crédit qui puisse permettre d'accompagner les projets de des jeunes notamment qui sud et territoire de Polynésie française, et de Nouvelle-Calédonie. Merci, cher collègue, avis de la Commission, monsieur passion. En dépit de l'objet de l'amendement, qui est d'étendre les compétences du feu, mais aussi sur la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ceci restera impossible car son intervention dans ce territoire resterait contraires à l'article 40 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'autre mère donc défavorable de la commission, car il faut une modification législative. Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, la vie de de la commission le le signal étant ne fait Bex à la Calédonie et à la Polynésie nécessite donc une modification législative dans les délais sont incompatibles avec votre préoccupation, par contre j'en avait déjà pris l'engagement auprès de la députée Sanquer, il est important que la Polynésie la Calédonie puisse être soutenue aussi dans l'ensemble de leurs projets éducatifs, sportifs et vous avez su me convaincre vous savez effectivement combien la jeunesse est importante, alors je m'engage ici à ce que ces 100000 euros soit mis au service des projets non pas dans le cas du FedEx mais hop des projets qui se rend à mon ministère dans l'année 2018 ans que ces 100000 euros, nous les mettre en au bénéfice de ces 2 territoires mais je vous demande effectivement parce que on peut pas le faire dans ce cadre-là, de retirer votre amendement merci beaucoup. Monsieur Canivet, au vu de ces précisions apportées par Madame la Ministre, tirez-vous votre amendement. Madame la présidente, au vu de la volonté nettement exprimé par Madame la ministre et que je salue, que je remercie, effectivement, nous allons le retirer en souhaitant que, enfin, les populations de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, puisse être accompagné tancer dans leurs déplacements, de même nature que celle des autres territoires d'outre-mer, merci. Bien, merci Monsieur Quenneville amendements. 513 rectifier et donc retirés, nous allons procéder au vote des crédits de la mission outre-mer figurant à l'État B. je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mets donc on voit les crédits de la mission. qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient Les crédits de la mission sont adoptés, j'appelle en discussion : les articles 57 quater 57 qu'inquiet 57 sexy, ses 57 cette qui sont rattachés pour leur examen au crédits de la mission outre-mer et j'ai une demande de parole de monsieur Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain me scientiste à vous la parole. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, la mission outre-mer du projet de finances pour 2018, de prime abord, le budget pour cette mission semble en augmentation

néanmoins You regarder de plus près, on constate que le programme 123 conditions de vie outre-mer subit une baisse de dotation que je qualifie d'importante au regard des situations compliquées, difficiles de nos territoires de mon train de 73 millions d'euros en à moins de et près de 53 millions d'euros CP, moins 7 pourcent cela d'autant plus inquiétant que cette baisse concerne la LB provoquant la diminution des constructions de logements sociaux dans nos territoires, à l'inverse des gouvernements précédents, par exemple en 2016 le nombre était fixé à 6953 dont 2802 logements très sociaux, d'ailleurs, l'article 3 de la loi et Rome prévoyait la construction de 150000 logements dans les outre-mer dans les 10 ans suivant sa promulgation, le gouvernement ne s'est engagé que sur 5870 logements locatifs sociaux et très sociaux, auxquels s'ajoutent 3550 opérations de réhabilitation du parc existant, ce qui est très insuffisant, donc sur la vie de milliers de familles mais impact important également sur l'activité des PME de la construction, cette baisse concerne aussi la continuité territoriale, moins 1,3 alors que le gouvernement s'était engagé à favoriser en 2018, les conditions d'augmentation du nombre de billets d'avion et aidés, cette baisse concerne également les collectivités territoriales, avec une diminution drastique de leur budget, moins 40 millions en a eux et 24 millions en CP, cette baisse concerne un autre le Champ sanitaire il sociale avec une baisse de 10 millions et de 2,1 millions en CP, alors même que nos territoires ultramarins dans le rassemble la difficulté avec des risques sanitaires spécifiques importants dans un contexte socio-économique dégradé, cette baisse concerne enfin l'insertion économique de la coopération régionale, moins 5 pourcent alors même qu'il faudrait au contraire augmenter largement ce montant afin de permettre à nos territoires de lutter contre la concurrence des îles voisines, proposant une fiscalité avantageuse, couplée à une détaxe des produits de navigation, j'ajouterai et je terminerai là-dessus que la PPL relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des Outre-Mer mer dans leur environnement régional pourtant voté en 2016 est parue au Journal Officiel du 6 décembre 2016 qu'on écrit au chaud, dans l'attente de décret d'application concernant certaines dispositions importantes, ce qui ont ralenti considérablement, pour ne pas dire annulent totalement la portée et l'ambition de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue. Je mais maintenant on voit l'article 57 quater, qui est pour. Qui est contre.

Merci, monsieur le rapporteur général vous soucier de la célérité de la séance à monsieur le président de la commission excusez-moi. Je mets au voilà retirerais le 57 cette Thiès même j'appelle en discussion l'amendement tendant à insérer un article additionnel, qui est rattachée, pour son examen au crédit de la mission outre-mer. Il s'agit donc après l'article 57 sceptiques de l'amendement 557 rectifié présenté par monsieur Vignon. Merci madame la présidente, j'ai compris des explications et des engagements de Madame la ministre danser les interventions au cours de notre discussion que l'objet de cet amendement pourrait figurer parmi les travaux et les préoccupations des assises qui me paraissent probablement plus adapté qu'un rapport à l'échéance de 1900 de 2019 en voie de conséquence, je retire l'amendement.

La présidente, simplement pour dire aux membres de la commission des finances, qui sont encore nombreux dans l'hémicycle que nous avons, dès maintenant, une réunion pour examiner des amendements de 2ème partie, nous en avons 350 à l'heure du jour. Vous avez de l'occupation pour cette soirée. Je vais maintenant suspendre la séance, elle sera reprise à 22 heures 10. Pour l'examen de la mission recherche et enseignement supérieur, la séance est suspendue.